La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, nous n'avons pas reçu d'observation. Il y en a-t-il en séance. Je n'en vois point. Le procès verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur, une délégation conduite par monsieur Hendrik Wüst, ministre-président du Land de Rhénanie. Du Westphalie. Et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne chargé des relations culturelles franco-allemande. La délégation est accompagné par notre collègue Ronan Le Gleut, président du groupe d'amitié du Sénat et par Monsieur, Hans Dieter Lukas, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en France à souligner l'importance de la coopération étroites et de longue date entre le Sénat et le Bundesrat au service de la relation franco-allemande. Nous aurons l'occasion de réaffirmer solennellement cette amitié en 2023 ont célébrant le 60ème anniversaire du traité de l'Élysée, la dimension culturelle devrait y occuper une place renouvelé, alors que l'apprentissage et la pratique de la langue de part et d'autre, tendent à se faire moins fréquent, nous devons réfléchir à de nouvelles initiatives permettant de conforter des expressions culturelles convergentes. Sans cultures partager la relation franco-allemande perdrait de sa singularité de façon plus générale, il est crucial que nos deux assemblées Oeuvres à la nécessaire solidarité entre les États membres de l'Union européenne

appelle de notre part une réponse qui soit à la fois commune et solidaire afin de préserver l'unité de la zone Euro et la force de nos 2 économies dans la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, en votre nom à tous, mes chers collègues permettez-moi de souhaiter. Ah monsieur Hendrik Wüst et à sa délégation la plus cordiale bienvenue au Sénat. Madame

Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La séance est retransmise en Direct sur Public Sénat et sur notre site internet au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun et chacune d'entre vous, mes chers collègues, observé au cours de nos échanges, une des valeurs essentielles, ici au Sénat, le respect, le respect des uns et des autres, et celui du temps de parole je vais immédiatement donner la parole au président François Patriat. Pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vous avez la parole Merci monsieur le Président, gardez votre téléphone pour vous, merci monsieur le Président Madame la première ministre, Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question fera écho à vos propos, monsieur le Président, puisqu'elle portera sur l'énergie et le prix de l'énergie qui préoccupe beaucoup nos concitoyens qui les inquiète, l'inquiétude et les chez les particuliers, l'inquiétude et chez les entrepreneurs chez les agriculteurs l'inquiétude, elle est aussi chez les maires et dans les collectivités locales. Je mesure aujourd'hui l'effort qui a été fait par le gouvernement au cours de ces derniers mois pour faire face à ce défi, ils ont été les réponses ont été nombreuses, elles ont été efficaces, je pense au bouclier énergétique, je pense au prix de l'énergie, je pense à la charte des fournisseurs qui a été signée ce matin même. Cela a permis d'une part, de juguler l'inflation, ce qui nous permet d'être en Europe ce qui ont le mois d'inflation aujourd'hui ce qui a permis de préserver le pouvoir d'achat nous compenser nous qu'on que ces mesures à court terme ne suffiront pas, il faudra la participation de tous, il nous faudra un changement d'attitude, il nous faudra de la sobriété, il nous faudra a vanté de nouveau le pays le Conseil européen avec Madame Pannier-Runacher qui s'est tenu cette semaine vendredi ah les ministres de l'énergie est arrivé déjà à certaines conclusions positives, notamment la conclusion de faire en sorte d'une contribution, une contribution sur les producteurs de pétrole et sur les producteurs d'énergie aujourd'hui, nous ne pouvons rester là, vous avez évoqué les pistes, monsieur le président, l'essentiel se jouera pour partie au Conseil européen de la fin de cette semaine et la lance ce Conseil européen ne faudra évoquer le plafond des prix il faudra évoquer le prix de l'électricité, celui du gaz deçà vont déjà les efforts que le gouvernement a fait pour y parvenir et qu'il entend y faire aujourd'hui je rappelle mes chers collègues, que l'effort consenti pour les boucliers et autres pour les collectivités, les entreprises et les particuliers aura coûté 100 milliards en 3 ans à notre pays quelles sont Madame la première ministre les pistes que vous pourrez évoqué vendredi prochain pour arriver au but que nous en venons de relever ce défi énergétique, je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à. Madame Élisabeth Borne Première ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, François Patriat. Je mesure parfaitement l'inquiétude des entreprises et des collectivités, face à la flambée des prix de l'énergie, de nombreuses communes, malgré des efforts de sobriété important se demande si elles pourront payer leurs factures et maintenir ouvert tous leurs services publics dans les prochains mois. Monsieur le Président Patriat ces communes, ces élus, vous les connaissez bien et les membres de mon gouvernement et moi-même avons échangé avec de nombreux élus locaux et avec les représentants de leurs associations. Tous portent le même message et mon gouvernement le porte avec eux, cette situation n'est pas tenable, nous devons agir et nous agissons alors nous agissons d'abord à la racine pour faire baisser les prix. Les prix ne retrouveront pas les niveaux artificiellement bas de la crise Covid mais ils ne peuvent pas non plus rester à des niveaux artificiellement au tirée par la spéculation, nous devons ramener les prix de l'électricité à des niveaux cohérent avec les coûts de production et pour cela, nous agissons d'abord au plan européen. Nous y travaillons et nous avançons bien vous l'avez mentionné la Commission européenne a ouvert la porte lors du conseil de l'énergie, vendredi dernier à l'élargissement du dispositif qui a permis de diviser le prix de l'électricité par 3 en Espagne, le président de la République s'est entretenu cette semaine avec le chancelier allemand et avec la présidente de la commission et ours ou la femme der Leyen a annoncé ce matin que la Commission ferait des propositions pour le plafonnement du prix du gaz lors du Conseil européen, ce vendredi, au niveau français, à d'autres mécanismes pour ramener les prix à des niveaux raisonnables mais nous agissons aussi pour protéger les consommateurs, le bouclier tarifaire dont j'ai annoncé mi-septembre la prolongation en 2023 et la mesure la plus protectrice d'Europe, la hausse de la facture de l'énergie pour les ménages, mais aussi pour les très petites entreprises et pour les petites communes sera limitée à 15 % ensuite je prends un engagement devant vous, aucune collectivité ni aucune entreprise ne sera laissé dans une impasse, je pense en particulier aux collectivités les plus exposés, comme celles qui connaissent des activités saisonnières ou qui gère de gros équipements, les ministres de l'Économie et de l'énergie ont réuni ce matin, les fournisseurs d'énergie, les engagements pris vont permettre qu'il n'y ait plus d'entreprises ou de collectivités 100 fournisseur d'énergie des offres seront faites à chacun, et la Commission de régulation de l'énergie va publier des indicateurs de prix pour que chacun puisse vérifier que les offres ne sont pas abusive par ailleurs s'agissant des entreprises, nous allons améliorer les aides exceptionnelles pour les gros consommateurs d'énergie, s'agissant des collectivités, elle bénéficie d'ores et déjà d'acompte pour soutenir leur trésorerie et le fait, filet de sécurité mis en place pour traiter les cas les plus difficiles, sera renforcé, le gouvernement présentera prochainement des propositions, donc vous voyez, Monsieur le Président, Patriat nous protégeons nos compatriotes nous protégeons nos collectivités, nous protégeons nos entreprises et nous veillerons à ne laisser personne sans solution, je vous remercie.

le 3 mars 2017 Emmanuel Macron affirmait publiquement un principe : tout ministre mis en examen devra quitter le gouvernement, engagement qui fut repris par Édouard Philippe Premier Ministre et qui fut appliquée : François Bayrou s'en rappelle, quelques jours après la prise de fonction de celui-ci comme garde des Sceaux. Quelques années plus tard, il y a 2 jours, nous apprenons que le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti ici présent et renvoyé devant la Cour de justice de la République pour des faits commis pendant l'exercice de ce mandat actuel comme ministre de la justice et rien. Simplement la réaffirmation de la confiance que vous lui donner. Madame la première ministre comment et quel motif a présidé au fait que ce principe présidentielle été reniée désormais. Pour vous répondre, l'appareil. Alors ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement Monsieur Olivier Véran. Vous avez la parole monsieur le Ministre. Moi aussi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, mesdames et messieurs les sénateurs, bonjour madame la sénatrice de La Gontrie, merci pour votre pour votre question, j'ai envie de vous dire puissiez-vous être aussi prompt à à venir dédouaner et accompagné à une personne qui, une fois mises en examen, auraient été innocenté que vous l'êtes aujourd'hui dans cet hémicycle, a demandé son exclusion pour le simple motif qu'elle est mise en examen et donc, par définition, loin d'être condamné, madame la sénatrice, il est souvent fait référence à une jurisprudence, celle du gouvernement Balladur qui avait donné lieu à l'éviction systématique de tout ministre mis en examen, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtise, mais il me semble que sur les quatres Ministre qui à l'époque avait été contraint à la démission parce qu'ils avaient été mis en examen, un seul avait été condamné trois auront donc été privé injustement en tout cas aux yeux de la justice, de la capacité qu'ils avaient de servir l'intérêt général et l'État, je vous dis madame la sénatrice gardons nous gardons-nous de jeter un opprobre systématiques sur les serviteurs de l'État sous prétexte qu'il ne partagerait pas nos idées politiques car vous savez que le nuage radioactif qui découle de telles attaques va en réalité irradié sur l'ensemble de la classe politique et de l'ensemble des serviteurs de l'État et qu'en définitive, c'est la démocratie qui se attaqués et affaiblis. Vous avez madame la sénatrice en tant que législateur, dans votre grande sagesse modifier un terme dans la loi en changeant le mot prévenu par le mot mis en examen, si vous regardez les minutes des débats au Sénat à l'époque, c'est intéressant, il était précisé que le mot prévenus semblait trop indiquait que la personne était coupable ou responsable par définition de ce qui lui était encore encore à peine reprocher alors que mis en examen, voulait vraiment dire ce de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'on allait regarder s'il y avait il y a lieu ou non de prononcer un acte de culpabilité, donc personne à ma connaissance, n'a été condamné, je dirais même qu'il y a un renvoi en cassation, qui a été fait dans le cadre du ministre Dupond-Moretti, ce qui veut dire qu'à l'heure à laquelle je vous parle, il est même plus factuellement, mis en examen, puisque la démarche a été suspendu en attendant la ville, la Cour de cassation, j'espère, madame la sénatrice avoir répondu à votre question. Madame de La Gontrie. Madame la première ministre plusieurs points tout d'abord, je note que le ministre qui a répondu au nom du gouvernement désavoue le président de la République et désavoue le Premier ministre, Édouard Philippe, dont acte. Ensuite je crains et je le dis avec solennité, je crains que vous n'étiez pas très bien compris ce qui est en train de se passer, nous parlons d'éthique gouvernementale, nous parlons du fait que tous ici, nous sommes considérés par les citoyens français comme des personnes qui ne sont pas honnêtes, nous avons besoin, nous avons besoin de réaffirmer l'éthique en politique, je citerai simplement ce qu'a dit François Bayrou lorsqu'il a démissionné du gouvernement, et ce sera je pense la réponse la plus efficace, il a dit je pars car j'ai choisi de ne pas exposer le président de la République et le gouvernement que je soutiens, c'est exactement ce qui est en train de se passer, sachant qu'un ministre de la Justice, renvoyé devant la Cour de justice de la République pendant l'exercice de ses missions, c'est totalement inédit, et cela va alimenter encore plus le populisme dans le de notre collègue Jean-Pierre Camby 16 pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président que présent Madame la première ministre monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne, elle aussi, la situation de nos communes face au coût de l'énergie, déjà fortement impacté par l'inflation 2022, les collectivités, le sont encore en 2023, avec une prévision au-dessus des 4 % la loi de finances rectificative pour 2022 a mobilisé une enveloppe de 430 millions pour les accompagner, mais nous savons déjà que cette enveloppe sera insuffisante même porté à un milliard d'autant qu'elle doit être aussi affectée à la compensation de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, par ailleurs, sa mise en oeuvre inquiète fortement les élus locaux, les qui répartition entre les différents niveaux de collectivités ne sont pas connues les modalités opérationnelles restent le critère de la baisse de l'épargne brute ne pourra être connue qu'avec le compte administratif 2022 c'est-à-dire au mieux en juillet 2023 comment gérer d'ici là, l'impact de la crise énergétique sur la trésorerie de nos collectivités, si la situation reste là, les élus seront confrontés à des choix cornéliens, augmenter les impôts diminuer les investissements ou Ferré, fermer certains équipements, on a évoqué les piscines, mais qu'en sera-t-il des salles accueillant les clubs sportifs ou les socio-culturel, voire pire, nos écoles, comment préserver tout ça sans mettre en péril les finances locales qui, rappelons-le, à la différence de celle de l'État doivent être équilibrées, les collectivités ont déjà largement contribué à l'effort national, il est temps de le renvoyer l'ascenseur à minima, les dotations versées aux collectivités doivent être indexées sur l'inflation, comme le réclame à bon droit, l'Association des maires de France, concrètement, monsieur le ministre, quelles mesures d'urgence à moyen terme et même pour l'hiver 2023 2024, entendez-vous prendre pour concrétiser la solidarité avec les communes, dont d'ailleurs, s'enorgueillit le président de la République à chacune de ses visites au congrès des maires de France. Jérôme Monsieur le Président Madame la première ministre monsieur le sénateur, comme cesse d'abord dans la continuité des propos qui ont été tenus par là. Première ministre il y a quelques instants, l'action, elle est globale, elle se fait d'abord à une échelle européenne pour que, avant de répondre précisément à votre question, il y a un effort coordonné pour baisser les prix et que les mécanismes de bouclier ne conduisent pas alimenter une rente que par ailleurs nous sommes en train d'essayer de récupérer avec le dispositif qui est conçu à l'échelle européenne, et qui s'applique déjà pour partie à l'électricité dans ce pays, ensuite, en ce qui concerne l'année en cours ce matin. Le comité des finances locales a été saisi du projet de décret qui est la traduction de ce qui a été voté dans cet hémicycle, l'enveloppe des 430 millions d'euros, dont vous avez parlé pour, précisément, à la fois préciser les règles du jeu est-ce que vous évoquez, sur le fait qu'il y aura un décalage par les comptes administratifs nous incite à penser que des dispositifs d'avance sur une partie du dispositif serait disponible pour pouvoir accompagner ce cette année transitoire plus largement. Je souhaite puisqu'on parle des collectivités locales au sens large, toute de suite expliqué qu'on a globalement 3 catégories : d'abord on a celles qui sont protégés par les bouclier tarifaire successifs qui ont été décidées de 4 % puis de 15 c'est toutes les communes qui ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions d'euros de budget, ensuite on a les départements et les régions qui sont confrontés à l'inflation, hein, d'autres éléments, mais qui ne sont pas impactés par les prix de l'énergie dans les mêmes proportions que le bloc communal qui lui est particulièrement concerné : il est d'autant plus que les communes qui sont au-delà du seuil que j'évoque, abrite le plus souvent, les équipements publics dont vous parlez, premières actions, on s'efforce de baisser les prix 2ème action nous prévoyons des dispositifs de soutien dans le cadre du PLF qui vous sera présenté et pour la première fois depuis 13 ans, l'enveloppe de DGF qui est proposé est proposé à la hausse, c'est une première depuis 13 ans, je sais, je n'ignore rien que certains aimeraient que ce soit davantage je signale néanmoins que ses premiers 210 millions d'euros, marque une rupture par rapport à des choses qui avait été indiqué enfin la première mini-vient de vous le dire, nous sommes en train en ce moment de finaliser le travail qui va nous permettre d'expliquer comment, face à une situation que nous considérons comme n'étant pas tenable, nous accompagnons les collectivités qui sont exposés en insistant auprès de vous que nous avons aujourd'hui communes qui sont encore couvertes par des tarifs d'énergie qu'elles ont négocié pour des périodes plus et d'autres qui sont déjà entrés en zone d'Exposition et qui se retrouvent confrontés au dilemme d'avoir des tarifs plus élevés que ce que leur financent leur permettent, nous y travaillons, vous aurez très bientôt la réponse. Monsieur le commissaire, vous avez quelques secondes. Tim ce ministre, je vous rappelle qu'il y a peu, vous étiez encore maire de cette belle ville danger Aurélie ou accepter de voter un compte administratif en déficit, la quiétude des élus locaux, aujourd'hui, va se transformer en colère en juin 2000 23 au moment des votes des comptes administratifs à 3 mois du roulement du Sénat, je vous laisse imaginer les conséquences, je vous remercie. La parole est maintenant au président Guillaume Gontard pour le groupe écologiste solidarité et territoires, vous avez la parole monsieur le président. Merci, merci Monsieur le Président Madame la première ministre à écouter à l'instant monsieur Véran, il est nécessaire et peut être utile de répéter deux fois une citation d'Emmanuel Macron je cite donc dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement, s'il est mis en examen, le principe, le principal danger pour la démocratie et la persistance de manquements à la probité parmi des responsables politiques, le président Macron a conservé sa conduite 6 semaines entre mai et juin 2017, le temps d'obtenir une Marie-Jo aurité absolue à l'Assemblée nationale depuis les affaires se succèdent à un rythme effréné, la banalisation et maintenant de mise, allant même jusqu'à la nomination au gouvernement de personnes lourdement accusé la république exemplaire et de devenue la République des affaires cette semaine un nouveau cap a été franchi avec la mise en examen du secrétaire général de neiger une première et le renvoi du garde des sceaux devant la Cour de justice de la rue de la République une première également alors Madame la première ministre connaissent tant la probité qui est la vôtre, allez-vous enfin l'appliquer à votre gouvernement. Pour vous répondre, la parole est à Madame la première ministre, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Gontard, comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'assemblée hier, j'ai pris acte de la décision rendue lundi de renvoi d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Comme chacun ici, je suis attaché à la séparation de l'exécutif, du législatif et de l'autorité judiciaire. Je ne commenterai donc pas cette décision, en revanche, je veux rappeler 2 éléments fondamentaux pour notre État de droit. Le 1er c'est l'indépendance de la justice, c'est un des piliers de notre démocratie. Et le second, c'est la présomption d'innocence elle aussi protège chacun elle aussi est primordial dans un état démocratique. Ces principes n'appelle ni commentaire ni exception. Dès lors, une seule question se pose cette situation affecte-t-elle le fonctionnement du ministère de la justice, ma réponse est claire et elle se fonde sur plusieurs mois de travail avec le ministre, alors oui, le ministère de la justice se réforme, se transforme, oui, le ministère de la justice avance et voit ses moyens atteindre des niveaux inédits, oui des réformes profondes s'engage notamment suite aux états généraux de la justice. L'engagement du ministre est résolu solide et indéfectible et pour les dossiers ou Éric Dupont-me de Moretti est un justiciable comme les autres ou pour ce qu'il a pu connaître en tant qu'avocat, nous avons mis en place un dispositif de déport il était exigeant, il est efficace, il me conduit à piloter en Direct une une série de sujets je vous remercie. Merci madame la première mini, je pense que vous n'avez pas bien compris, le sujet n'est pas ici la présomption d'innocence, le sujet c'est le respect de la parole donnée, qui plus est de la parole présidentielle, le sujet c'est de ne pas ternir l'image du gouvernement de la France, le sujet c'est de disposer de ministres à temps plein au service des Françaises et des Français, le sujet c'est la sérénité qui incombe à la décision de justice, à fortiori quand le justiciable et le garde des Sceaux, c'est la préservation de l'indépendance de la de la justice Emmanuel Macron nous avait promis l'exemplarité politique de mise sous François Hollande mais ils nous ramènent aux pratiques délétères des présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, alors que la crise démocratique et plus profonde que jamais, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir alors que les fascistes l'ont conquis de l'autre côté des Alpes, la responsabilité qui est devant l'histoire est considérable Madame la première ministre, il est encore de temps de prendre la bonne décision. La parole est à notre collègue Dany Wattebled pour le groupe, les indépendants républiques et territoires. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis 30 ans, la France fait face à la perte de son industrie, faute de politiques adéquates, nous en avons enfin pris conscience ces dernières années, elles ont commencé à prendre les mesures pourtant face à l'explosion du prix de l'énergie, cette menace est de nouveau d'actualité. Le mégawattheure de gaz naturel redescend difficilement sous la barre de 200 euros, les prix de électricité s'envole après 10 ans d'excédent, la balance commerciale de la zone Euro a lourdement a Tous les secteurs sont concernés, du verre à l'aluminium en passant par le ciment ou encore l'acier. Aux difficultés des collectivités, des agriculteurs et bien sûr des familles évoquée depuis des mois, s'ajoute celle des entreprises, elles organisent leur activité dans les prochains mois à la baisse. Les PME annonce des fermetures au licenciement s'ajouteront des fragilités importantes sur des secteurs clés et des importations obligatoire en provenance d'autres continents. Nos souveraineté une menacé sur bien des aspects, notamment industriels et alimentaires certaines Pelo ils sont à Khan, cela risque de nuire non seulement pour d'achat mais aussi à la puissance économique, c'est un choc majeur de comité pour l'Europe, l'écart n'est plus entre pays européens mais entre l'Europe et le reste du monde, ce qui laisse craindre de nouvelles délocalisations. Alors que l'urgence est à la soudure européenne les discussions sur le découplage du prix du gaz et d'électricité, rencontre des difficultés : une action unilatérale fragilise l'autre ensemble. Je comprends la volonté de nos amis allemands, avec leur bouclier anti-inflation, mais au-delà c'est amitié, nous ne pouvons pas continuellement subir leurs choix en matière énergétique, monsieur le Ministre quelles actions comptez-vous mener pour éviter cette catastrophe économique, tant au niveau français qu'au niveau européen. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics Monsieur Attal, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Wattebled, comme l'a indiqué la première ministre tout à l'heure, l'essentiel de la mobilisation du gouvernement aujourd'hui du président de la République, c'est d'agir pour faire baisser les prix de l'énergie sur le marché européen, la première ministre a rappelé les échanges, les réunions extrêmement importants qui se sont tenues, la réalité c'est que nous avons une responsabilité, nous avons un objectif, c'est d'empêcher que la crise de l'énergie se traduise par des difficultés économiques supplémentaires cet objectif, il nous anime en réalité depuis plus d'un an maintenant, et nous avons d'ores et déjà pris des mesures avec le bouclier énergétique avec des mesures plus spécifiques pour soutenir le secteur industriel que vous évoquez cette année avec notamment les mesures sur la reine, ce sont 45000 emplois industriels qui ont été sauvées cette année en 2022 dans 150 établissements par les mesures que nous avons prises, il faut donc continuer à agir hein en refroidissant, le marché de l'énergie avec les propositions que fait la France et que porte la France pour découpler le prix d'électricité du prix du gaz avec les mesures qui ont été annoncées par Bruno Lemaire ce matin, c'est le premier objectif et le 2ème objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui sont particulièrement fragilisée particulièrement consommatrices d'énergie, nous avons pour cela, il vous l'avez voté cet été, une enveloppe de 3 milliards d'euros, qui permet de soutenir les entreprises qui ne sont pas au tarif réglementé, elles peuvent se rendre sur le site impôts Point gouv Point FR il y a un simulateur et elles peuvent recevoir une aide jusqu'à 50 millions d'euros, la première lecture que nous avons eue, c'est que les critères étaient trop restrictif, nous avons déjà élargi une première fois, nous travaillons au niveau européen pour pouvoir élargir davantage ces critères et nous travaillons par ailleurs à d'autres mesures qui pourraient venir soutenir les entreprises, donc le message que je veux passer, c'est que depuis un an nous avons agi et permis à nos entreprises de tenir et et que notre action va se poursuivre et s'amplifier pour leur permettre de tenir parce qu'agir pour les entreprises, c'est agir pour les Français, c'est permettre à nos concitoyens de conserver notre emploi et c'est permettre à notre économie de rester dynamique. Merci, la parole est à notre collègue Étienne Blanc pour le groupe Les Républicains. Le président et voici quelques jours la semaine dernière avec le groupe d'amitié France- Arménie du Sénat, nous nous sommes rendu à Erevan avec notre collègue son président Gilbert Luc de vinasse nous avons effectué ce déplacement alors que l'Azerbaïdjan se livrait à ça, énième attaque contre le peuple et contre le territoire arménien, quelques jours auparavant, Madame von der Leyen s'étaient rendus à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan et la elle avait signé un accord gazier pour assurer la sécurité des livraisons de gaz au profit de l'Europe, la concordance de ces 2 événements ne saurait être fortuite pour le peuple arménien alors Madame la première ministre ma question est simple aujourd'hui, le gouvernement français se sentent-ils solidaires de cet accord que l'on peut juger indigne et puis l'Arménie a exprimé elle exprime régulièrement son souhait d'obtenir des livraisons d'armes de défense la France accepte-t-elle aujourd'hui d'être le fer de lance d'un dispositif permettant à l'Arménie, de disposer de ces armes pour assurer sa protection, la protection de son peuple et de son territoire, la France préside le Conseil de sécurité de l'ONU une demande prégnante de l'Arménie et d'obtenir de l'ONU, la présence d'une force d'observation et d'interposition sur sa frontière avec l'Azerbaïdjan, pouvez-vous aujourd'hui prendre au nom de monsieur le président de la République, l'engagement que la France déploiera des efforts incessants pour que cette force d'interposition se mettent en place, c'est la condition de la protection de l'Arménie et de son peuple

Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs, monsieur le sénateur blanc, vous le savez, la France est pleinement solidaire du peuple arménien, elle a toujours été, vous l'avez dit, elle a toujours été parce que nos histoires ont été liés depuis que notre pays a accueilli les rescapés du génocide arménien de 2015. elle est aux côtés du peuple arménien les solidaire du peuple arménien le restera, je sais ce que nous parvenions à un règlement négocié et pacifique du conflit qui l'oppose à l'Azerbaïdjan, les armes ont assez parlé, Monsieur le Sénateur, les incursions armées de l'Azerbaïdjan et les frappes menées contre le territoire internationalement reconnue de l'Arménie, constitue une violation de la charte des Nations unies, elles doivent cesser, nous l'avons dit je le répète ici même, nous nous mobilisons aussi pour obtenir la libération des prisonniers arménien prisonniers de guerre et je peux vous faire savoir que 17 d'entre eux ont été libérés hier par l'Azerbaïdjan alors la France avec l'Union européenne est engagée dans un processus de dialogue entre les 2 pays qui se poursuit en ce moment même, et que le président de la République poursuivra demain avec un certain nombre de ses collègues européens parce que c'est l'attachement à la paix et au droit international qui guident notre action et c'est ainsi que sera garanti le droit de l'Arménie à vivre libre, nous avons aussi réunis, monsieur le sénateur, le Conseil de sécurité sous présidence française à 2 reprises les 15 et 16 septembre parce que oui, le Conseil de sécurité peut avoir un rôle, vous avez raison, mais comme la priorité immédiate est de faire baisser les tensions et que pour cela il faut établir un constat objectif de la situation, la frontière nous oeuvrons concrètement à obtenir l'envoi rapide d'une mission d'établissement des faits de l'OSCE et je vais demander au président en exercice de cette organisation, il y a quelques jours à peine, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à madame Annick Billon pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole madame la présidente. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la première ministre dans notre rapport sénatorial porno l'enfer du décor avec mes 3 collègues corapporteur Alexandra Borchio Fontin Laurence Cohen et Laurence Rossignol nous avons pour la première fois dans l'histoire du Parlement révéler les dessous sordides de cette industrie de la pornographie, une industrie qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année dans des conditions opaques, une industrie qui a fait de la marchandisation du corps et de la sexualité des femmes un Business à l'échelle mondiale, la consommation de porno aujourd'hui et massive, elle représente plus d'un quart de tout le trafic vidéo en ligne dans le monde, le site Pornhub cumule à lui seul plus de 40 milliards de visites annuelles et près de 220000 vidéos vues chaque minute dans le monde, notre rapport dresse un tableau très sombre mais réaliste des pratiques de cette industrie violence systémique envers les femmes, exploitation de leur précarité économique et sociale, actes de torture et de barbarie, les 2 affaires judiciaires en cours en France, en témoigne : elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg, nous appelons à sortir de toute vision datée faussé et édulcoré du porno Le porno aujourd'hui ce sont majoritaires militairement des contenus violents dégradants, humiliants tous ces contenus sont facilement et massivement accessible aux mineurs, 2 tiers des enfants de moins de 15 ans et et un tiers de moins de 12 ans ont déjà vu des images pornographiques, la délégation porte unanimement 23 propositions pour lutter contre les violences pornographique et leurs conséquences, ma question est la suivante Madame la première ministre, comment comptez-vous vous emparer de ses propositions.

Merci monsieur le président, madame la présidente, Annick Billon, je vous remercie pour votre question et je tiens à saluer la qualité du travail que vous avez effectuées avec vos collègues, Laurence Rossignol, Alexandra Borchio vous feront hein et Laurence Cohen, votre rapport est extrêmement utile parce qu'il a permis de mettre un coup de projecteur sur les dérives d'une industrie qui, pour reprendre vos mots est une machine à broyer les femmes, une industrie qui a banalisé les violences sexistes et sexuelles oui le porno est un enfer pour les femmes, votre rapport propose des solutions concrètes pour protéger nos enfants, mais pour protéger aussi les actrices de cette industrie, certaines de vos recommandations rejoignent le travail d'ores et déjà engagées par le gouvernement, avec mon collègue pape Ndyaye Ministre de l'Éducation nationale, nous nous sommes saisis dès notre arrivée au gouvernement du chantier de l'éducation à la sexualité, il est grand temps que la loi de 2001 soit appliquée dans nos écoles, je pense aussi aux travaux pilotés par Jean-Noël Barrot et Charlotte Caubel sur le contrôle parental sur les smartphones, mais nous pouvons aller plus loin et votre rapport alimentera grandement les travaux que nous mènerons prochainement avec mes collègues de la justice, de l'intérieur de la culture du numérique et de la protection de l'enfance, nous nous rencontrons, vous le savez, le 18 octobre et je sais que nous avancerons ensemble de manière constructive, je vous remercie. vous avez la parole. de ce qui attend nos collectivités comme nos concitoyens et nos entreprises en matière de facture énergétique et cela malgré les nombreuses alertes formulées notamment par toutes les les associations d'élus, les 430 millions d'euros, du projet de loi de finances rectificative que vous évoquez ont été arrachés cet été par les parlementaires que nous sommes et moins de 8000 communes vont malheureusement bénéficié du fait des critères que vous avez retenu quant aux fournisseurs dont dont dont vous vous réjouissez qu'ils aient signé ce midi une charte. hier encore. Il menaçait des communes de les couper, d'énergie, si elle ne payait pas les tarifs qui s'apparente, certains élus locaux l'ont dit à du raquette les sommes en jeu sont telles qu'il ne suffira pas d'éteindre l'éclairage public ou de baisser d'un degré le chauffage dans nos écoles et on risque en effet de vivres des coupures de service public dans nos territoires le comble, c'est que nos collectivités sont en train de repousser des investissements qui permettrait précisément de réaliser des économies d'énergie, allez-vous enfin entendre ce cri d'alerte et examiner les propositions qui sont sur la table par exemple le retour aux tarifs réglementés de l'énergie, de, de, de vente de l'énergie pour les collectivités. Pour vous répondre la parole comme ministre délégué chargé des comptes publics. et des tensions et des inquiétudes de nos collectivités que nous consacrons l'essentiel de notre temps, je le disais il y a un instant à agir face à cet emballement des prix de l'énergie, ma collègue Agnès Pannier Runacher pourrait vous en parler, elle termine ses soirées et ses nuits à Bruxelles pour négocier les avancées sur le marché de l'électricité commence ses journées comme ce matin avec les fournisseurs, en France, précisément pour lutter contre les pratiques que vous évoquez, donc oui, nous en avons pleinement conscience, et je le redis, la première priorité, c'est ce à quoi nous sommes en train d'aboutir, c'est de réformer le marché européen de l'électricité pour faire baisser les prix, la 2ème priorité c'est de soutenir et d'accompagner les collectivités locales, mon collègue Christophe Béchu rappeler un instant que nous avons saisi aujourd'hui le comité des finances locales du projet de décret qui fait suite aux dispositifs de filet de sécurité que vous avez adoptée et même enrichi enrichi au Sénat, c'était notamment le travail du rapporteur général Husson, ce que je peux vous annoncer, c'est que les collectivités locales pourront faire une demande d'acompte dès la semaine prochaine et que celui-ci pourra leur être versé entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, on parle ici d'une prise en charge jusqu'à 70 % de la hausse des prix de l'énergie ou de l'alimentation pour les collectivités ou ou jusqu'à 50 % de la hausse de la masse salariale liée au à l'impact du point d'indice, donc il y a cette action qui est menée, le tarif réglementé s'applique pour 30000 des 36000 communes, celles qui ont moins de 10 salariés ou moins de 2 millions d'euros de budget pour les autres, nous avons fait le filet de sécurité cette année nous allons plus loin avec le PLF en prévoyant Christophe Christophe Béchu la rappeler aussi une revalorisation de la DGF de 210 millions d'euros de sorte que 70 % des communes verront leur DGF augmenter l'année prochaine et nous continuons à travailler par ailleurs et je pense que c'est aussi encore un enjeu qui nous réunira dans l'examen du PLF à de nouveaux dispositifs qui pourrait s'inspirer aussi du filet de sécurité pour soutenir là encore les collectivités face à ces difficultés liées au prix de l'énergie, vous le voyez, nous sommes mobilisés sur la question du prix pour le faire baisser et sur la question, l'accompagnement des collectivités pour continuer à les renforcer Non, Monsieur le Ministre, toutes les collectivités n'ont pas accès aux tarifs réglementés, notamment pour le gaz. Et ce tarif réglementé va bientôt disparaître pour tout le monde en juillet 2023 et les questions qu'il n'y en ait plus pour personne, vous pourrez faire signé toutes les chartes que vous voulez si vous nous démunis c'est si vous démunis c'est la puissance publique de moyens d'agir, il ne se passera qu'une accélération des fins de phénomène que nous connaissons aujourd'hui. Merci.

Monsieur le président, Mesdames, messieurs les Ministres, chers collègues, femme vie liberté ces 3 mots se propage à travers le monde en soutien aux courageuse iranienne qui brûlent leur voile pour réclamer l'abolition d'une loi qui les oblige à se couvrir, symbole de la soumission et l'oppression des femmes dans une société patriarcale face à un pouvoir théocratique dont elle ne supporte plus le carcan le gouvernement va-t-il enfin admettre que le voile est un étendard politico- religieux quand en Iran le voile semble être la Pierre angulaire du régime des mollahs je regrette encore votre attitude d'opposition à tous les amendements que nous avions déposé dans le cadre de la loi séparatisme et que vous avez qualifié d'amendement textile textile alors qu'aujourd'hui, clairement, les entraves à la laïcité dans nos écoles augmentent de manière inquiétante et que les abayas, les cas Miss le risque dans les lycées, signe de l'influence islamiste et particulièrement des Frères musulmans, qui se diffusent dans l'esprit d'une partie de notre jeunesse, quand le gouvernement va-t-il enfin avoir un discours et des directives très claires sur ce sujet. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Et du service national universel, madame, elle est vous avez la parole madame la ministre. Merci monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice stage Bruno, on connaît votre engagement pour la laïcité, madame la sénatrice, mais la loi, confortant les principes républicains, porté par Gérald Darmanin et ma collègue Marlène Schiappa ont permis des avancées réelles et nous permet de porter en réalité des coups aux atteintes de la laïcité, cependant, madame la sénatrice, votre question elle porte réellement sur la laïcité à l'école et ces atteintes oui aujourd'hui, Madame la sénatrice, il y a des atteintes à la laïcité au sein de nos établissements scolaires et c'est pour ça que nous nous luttons pied à pied, comment déjà en toute transparence, en faisant appliquer toute la loi de 2004, parce que plus que jamais les signes religieux ni les tenues qui pourrait être considéré comme incident le jeune ont leur place au sein de nos établissements scolaires alors c'est le fruit d'un travail qui avait été déjà porté par Jean Michel Blanquer et qu'on continue à porter, c'est pour cela que nous souhaitons objectiver ce phénomène, la réalité c'est que nous avons besoin de chiffres, le ministre pas prêt PAP NDiaye a décidé de chaque mois, rendre publics ces chiffres au sein de notre de nos enceintes madame la madame la sénatrice, la clarté, la clarté, nous permet de nous appuyer sur le vade-mecum de la laïcité, qui rappelle que une tenue peut être considéré comme un signe religieux par destination, si elle est porté de manière régulière et que le jeune ou l'étudiant refuse de l'enlever, madame la sénatrice, vous savez que pour nous, l'école, hé bien, c'est un sanctuaire, ce sanctuaire est un sanctuaire républicain et nous accepterons aucune atteinte aux valeurs de la République, c'est pour ça qu'il y a les équipes qui soutiennent les chefs d'établissement, madame la sénatrice, ainsi que les enseignants, nous appliquons la loi de mille quatre, toute la loi de 2004 avec transparence et clarté. Madame la sénatrice. Il n'est plus, il n'est plus temps de faire semblant, notre pays se fracture sur ce sujet ces dernières années et vous y avait contribué, refusant tout discours de fermeté des enseignants sont abandonnés ou livrés à eux-mêmes et parfois se censure sur leur programme, face à des exigences communautaristes de plus en plus forte, le monde du sport fait face aux mêmes difficultés l'ambiguïté des discours et l'absence de directives claires ont engendré des situations de plus en plus ingérable et de moins en moins supportée par la grande majorité des Français lorsqu'un ministre ose dire que les problèmes peuvent être réglés en faisant appel au bon sens et à l'expérience des équipes pédagogiques, cela revient à dire : débrouillez-vous, on ne négocie pas avec la laïcité émancipatrice de la jeunesse, le voile et la vitrine et islamistes qui savent tirer parti de notre tolérance et de notre faiblesse aujourd'hui les femmes iraniennes nous démontre chaque jour au péril de leur vie, faisant face à la police des moeurs qu'il est de notre devoir d'avoir enfin du courage. Merci

Merci monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre diplomatie revendique d'avoir des partenariats privilégiés avec l'Afrique, si l'actualité la plus récente oblige à en douter, je vous concède néanmoins qu'il existe bien des échanges humains, culturels, éducatifs économiques intemporel la décision prise par le président de la République en conseil de défense, il y a un an, de réduire de 50 % le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et algériens et de 30 % pour la Tunisie touche précisément ce qui tisse et entretiennent ces Liens, cette politique du chiffre qui se veut être la démonstration de votre volonté de réduire l'immigration emporte de conséquences délétères, elle est d'abord vécu comme une punition collective par ceux qui ne présente aucun risque migratoire qui se rend en France pour certains depuis des décennies, à des fins familiales ou professionnelles, les perdants se sont quand à humilié et on exprime une aigreur et un ressentiment dans la presse nationale se faisait encore l'écho ce matin ce sont ensuite des appels d'offres perdu parce que l'investisseur étranger n'obtient pas le VISA nécessaire, il se tourne vers un autre pays plus accueillants, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie en tire aujourd'hui des bénéfices économiques et vous en remercie de toute évidence, les mesures mises en place depuis un an, se révèlent inefficaces, les États concernés n'ont pas accepté de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière, l'immigration illégale n'a toujours pas cessé quant aux effets politiques et électoraux que vous en attendiez les dernières élections ont montré la vanité de votre démarche, il est temps de laisser à nouveau le soin au personnel expérimenté de nos consulats d'instruire les demandes dont ils sont saisis toutes les demandes et, ce faisant, refuser celles qui doivent l'être, il est temps de négocier des accords bilatéraux en matière d'immigration accord sans lesquels le tissu affectif et charnel de la relation qui nous lie à l'Afrique s'estompera sans lendemain, qu'en pensez-vous Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Europe. Mais les affaires étrangères Madame Colonna. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénatrices madame la sénatrice Conway Mouret 3 pays du Maghreb, madame la sénatrice, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont fait l'objet depuis septembre 2021 2 mesures restrictives sur la délivrance des visas, ces mesures de restrictions ont été décidées par le gouvernement, vous l'avez rappelé madame la sénatrice en réponse au constat d'une forte baisse du nombre de laissez-passer consulaires délivrés par ces pays dans le cadre des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des étrangers en situation irrégulière sur notre territoire par le ministère de l'Intérieur, je tiens à souligner que les discussions récentes entre le ministre de l'Intérieur français et des pays concernés en matière de coopération migratoire sont positives, il y a une réelle amélioration de la situation et qu'elle se poursuive de façon constructive, le ministre de l'Intérieur, comme moi-même, nous nous en réjouissons nous progressons encore tout récemment, il y a quelques jours à peine avec le Maroc et nous souhaitons pouvoir continuer d'avancer, afin de mettre un terme à cette situation, je tiens d'ailleurs à rappeler que les mesures restrictives qui avait été mise en oeuvre, l'ont été avec le souci de préserver au maximum les publics prioritaires, notamment les étudiants, les entrepreneurs, les artistes ou d'autres, et enfin, au-delà du sujet spécifique de ces mesures et de leur évolution en cours ou à venir, je ne les connais pas l'enjeu des délais de traitement des demandes de VISA dans nombre de nos consulats, ils sont parfois trop long c'est vrai nous l'entendons, de tous côtés, mais ils sont tout simplement après 2 années, contrainte par la pandémie de Covid 19, donc moi mystère et mobilisé pour les réduire, j'ai décidé que des renforts seront envoyés dans les pays qui en ont le plus besoin et je créerai rapidement un centre de soutien spécifique dédié à ces à ces missions, je vous remercie. Madame Beaudoin Morel. Il y. Je crois qu'au au vu du de la montée du sentiment anti-français sur le continent africain, je crois qu'il est urgent lorsque la politique migratoire touche aux relations entre États, je crois qu'elle ne peut pas être le seul fait du ministère de l'Intérieur. Donner la parole à notre collègue Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains. merci, monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la première ministre puisqu'elle fait suite à une déclaration du président de la République qui a un pacte de nombreuses politiques publiques de la question migratoire à celle de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale, au logement, le combat pour la ruralité son développement sa modernisation son attractivité autre au centre des préoccupations du Sénat sur tous les bancs de cet hémicycle, alors que la reconquête de cette qui a cruellement manqué de vision politique pendant des années, est aujourd'hui possible, nous avons été nombreux à être sidéré par les déclarations du président de la République devant les préfets, il y a quelques jours en effet, le président a proposé une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment, je cite, dans les espaces ruraux, qui eux sont en train de perdre de la population et où nous devrons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges dans ces régions, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans les zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, a-t-il ajouté, je vois merci donc Madame la première ministre de bien vouloir préciser devant la représentation nationale, votre vision de la ruralité comme de l'immigration d'ailleurs suite à ces déclarations et les intentions du gouvernement pour les mettre en oeuvre, y a-t-il des projets de quotas territoriaux, y a-t-il un conditionnement du maintien des services publics à l'accueil de migrants si oui lesquels je vous remercie. Ah c'est Madame Cayeux pardonnez-moi. la politique migratoire de la France, c'est l'un des axes prioritaires du ministère de l'Intérieur, des débats sont d'ailleurs prévues dans les semaines à venir au Sénat et à l'Assemblée nationale avant la présentation d'un projet de loi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin en début d'année prochaine, nous le savons, notre politique migratoire doit évoluer pour cela, nous devons être plus ferme avec celles et ceux qui n'ont pas leur place sur le sol français et dans le même temps mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à y rester, l'intégration des étrangers en situation régulière et lui, un enjeu majeur de notre politique migratoire et c'est l'honneur de la France, mais le système actuel qui conduit à une trop forte concentration sur certains territoires n'est pas satisfaisant, il suffit d'en parler aux élus locaux concernés, qui se tournent régulièrement vers l'État pour les accompagner, face à ces situations humainement compliquée à gérer, nous devons donc mieux organiser les flux et les accueil de migrants, pour mieux les intégrer le mécanisme de répartition territoriale existe déjà, il fonctionne et fait ses preuves pour les demandeurs d'asile, nous l'avons d'ailleurs mis en oeuvre à grande échelle avec l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine, une grande partie d'entre elles, qui avaient afflué en quelques jours dans les Oeuvres de Paris, Strasbourg et Nice, une fois l'accueil d'urgence garantie, nous leur avons proposé d'être hébergé partout sur le territoire et cela a fonctionné cette politique, il faut donc aujourd'hui la développé notamment à travers des mécanismes incitatifs, c'est le travail que nous conduisons, là encore, en étroite concertation avec les territoires, les associations, les élus locaux qui sont mobilisés pour répondre aux enjeux d'intégration, d'emploi, de formation et d'attractivité, je vous remercie. Je vous remercie, madame la ministre, je ne pense pas que vous ayez répondu à la préoccupation que j'essayais de vous faire partager la ruralité n'est pas un sou, territoire ni pour les immigrés, ni pour ceux qui y vivent d'ailleurs le problème de l'immigration n'est pas celui d'une répartition territoriale mais d'un contrôle d'une maîtrise et de l'application des textes n'entrera ruralité pardon accueille déjà de nombreux étrangers et en particulier les réfugiés ou les exilés d'Ukraine, mais c'est pas du tout le sujet que que je sur lequel je vous interroger et ceci de manière choisie et humaine, la ruralité n'a pas effectivement aujourd'hui le coeur en berne, mais nous nous refusons à devenir une réserve où on les Parker et au moment où nous nous battons pour la prise en compte de quelques sujets majeurs pour notre ruralité Services Publics École santé Ozanne nous renvoyer cette vision de la ruralité et cruel et méprisant, il semble que pour certaines ne soyons destinée qu'à accueillir les migrants pour soulager les banlieues vous l'avouez presque et les éoliennes pour éclairer les urbains, la ruralité souterrain sous territoire de la France, c'est non et je pense que c'est pas le message qui a été envoyé par les Français au moment de l'élection présidentielle, je vous remercie.

Bamako Bangui Yaoundé Dakar N Djamena et samedi dernier, Ouagadougou partout en Afrique, le sentiment anti-Français grandit et se manifeste de plus en plus violemment les contestataires exigent d'une part, le retrait des institutions françaises, de la gestion du franc CFA et d'autre part, s'oppose à la présence militaire de notre pays sur leur continent, les réseaux sociaux massivement utilisés dans une guerre de l'information de la manipulation amplifie, bien entendu, ce phénomène la présence sur le continent africain de puissances comme la Chine ou la Russie contribue à changer la donne, Russie, qui se présente comme une alternative face à l'impasse militaire française au Sahel, via une société paramilitaire privée que nul n'est besoin de nommer d'ailleurs en parlant de ces 2 pays, ironie de l'histoire, nous avons vendu l'immeuble du ministère de la coopération, a des Russes qui eux-mêmes l'ont ensuite revendu à l'État chinois qui a installé son ambassade, certains y voient un symbole sur notre politique vis-à-vis de l'Afrique, bref, il y a, et vous le savez mieux que quiconque une spirale exponentielle là et d'actes anti-français sur place, les milliards d'euros d'aide publique au développement ne change pas la donne, car ce jugement est irrationnel et le malaise extrêmement profond par maladresse, peut être, par manque de communication assurément, nous ne parvenons pas à convaincre ou tout simplement à rassurer les populations locales sur nos louables intentions en Afrique il y a 20 ans, les slogans anti-français, du Style on en a marre aujourd'hui le slogan récurrent et France dégage, nous sommes donc en droit de nous inquiéter sur la nature du slogan de demain Madame la Ministre, comment interrompre ce processus de dégradation de l'image de notre pays, dégradations qui impactent directement nos entreprises présentes sur place ah qui, parfois, on laisse 48 heures pour quitter le territoire et qui impacte aussi naturellement nos 250000 expatriés présents sur ce continent.

c'est vrai, monsieur le sénateur, la France est victime d'une scandaleuse campagne de désinformation en Afrique, dans laquelle certains se laissent entraîner et qui produit des effets, nous prenons ce phénomène nous allons-y répondre, mais nous n'allons pas y répondre en recourant aux instruments de ceux qui cherchent à nous nuire, nous allons tout simplement dire et répéter la vérité, la vérité c'est que la France a doublé son aide publique au développement depuis 2017 et que celle-ci est très largement concentré dans les pays d'Afrique les plus fragiles, la vérité c'est que nous agissons concrètement dans la lutte contre le changement climatique pour la santé : pour le renforcement des systèmes agricoles, la vérité c'est que nous soutenons la culture, le sport, la jeunesse, l'éducation, les entrepreneurs, la vérité, c'est aussi que nous nous interdisons toute ingérence comme à nouveau au Burkina Faso, ces derniers jours alors malgré cela, oui, nous sommes la cible de campagnes de désinformation, elles sont orchestrées professionnel peut être organisé, je ne reviens pas sur vos propos, nous y répondrons en mettant mieux en valeur ce que le partenariat avec la France apporte aux pays qui le souhaitent, c'est le sens du programme de renforcement de nos capacités diplomatie publique en Afrique lancée depuis cet été, depuis cet été, seulement au sein de mon ministère, de rappeler les les paramètres du partenariat avec la France un partenariat d'égal à égal, respectueux, un partenariat avec les États, comme avec les sociétés civiles et qui peut s'appuyer aussi, nous le ferons sur les diasporas présente également chez nous, je vous remercie. Monsieur de billets, vous avez quelques secondes, la parole est à notre collègue Charles Guené pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, Mesdames et messieurs, le Ministre, mes chers collègues, madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales en juillet dernier lors du projet de loi de finances rectificative le Sénat améliorer le filet de sécurité proposées pour les communes et les groupements, les plus fragiles, en le portant à 430 millions d'euros, enfin de leur permettent de résister à l'inflation et au dégel de ceux du point d'indice. Vous nous aviez alors précisé que ce filet de sécurité bénéficierait à 22000 communes sur les 35000 que compte notre pays, les collectivités ont de plus en plus de doutes quant à l'efficacité de ce filet non je précise le CFL a refusé les termes ce matin et elle goûte assez peu les fuites de notes confidentielles parvenu fort opportunément à la presse, affirmant qu'elle serait en pleine santé, pouvez-vous nous assurer qu'au terme de ce processus, ces 430 millions d'euros parviendrons bien aux collectivités locales comment expliquez-vous que le chiffre évoqué en juillet 2 22000 communes soit réduit désormais à moins de 9000 selon les propos les propos tenus devant notre commission des finances à moins de 10 jours. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée. En charge des collectivités territoriales Madame Cayeux. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Charles Guené. Si on veut mettre les choses au clair au début de l'année 2022 les finances des collectivités se portait plutôt bien, même si cette situation générale dissimule a déjà des disparités influence inflation que nous connaissons va dégrader leurs finances en 2000 22 et et pèsera encore plus sur les Budgets en 2023, de manière plus ou moins forte selon les catégories de collectivités et la part des dépenses d'énergies dans leur budget, or il est essentiel, nous le savons tous que les collectivités préserve des marges de manoeuvres financières pour qu'elle puisse mettre en oeuvre des services publics de qualité et qu'elle puisse investir massivement dans la transition écologique, le gouvernement est pleinement conscient que l'État a besoin des collectivités locales et doit donc être à leurs côtés, c'est dans ce sens que nous avons construit le projet de loi de finances pour 2023 avec Christophe Béchu et Gabriel Attal après avoir consulté, tant l'ensemble des associations d'élus dans une méthode de concertation qu'elle semble avoir salué, nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir ensemble d'ores et déjà un filet de sécurité pour les communes les plus par l'inflation en 2022 a été votée dans le cadre de la loi de finances rectificative son décret d'application a été présenté ce matin en comité des finances locales, vous y étiez, monsieur le sénateur, selon nos estimations, plus de la moitié et les 3 quarts des communes et les 3 quarts des groupements seront éligibles, il conviendra évidemment d'attendre la clôture des comptes 2022 pour savoir qui bénéficiera effectivement de la compensation toutefois dès la parution du décret un acompte pourra être demandé pour qu'il puisse être versée avant la fin de l'année une demande devra être adressées avant le 15 novembre au service de l'État, ce filet pourra d'ailleurs et Christophe Béchu l'a dit tout à l'heure, aspirer un nouveau dispositif de soutien pour 2023 si le Parlement le décide, lors des discussions budgétaires. Madame la Ministre, après les augmentations qui plombe leurs finances s'ajoute désormais un effort supplémentaire est supérieur à celui que l'État s'impose à lui-même, qui sera demandé aux collectivités sur leur budget de fonctionnement, celui-ci devra diminuer de 0,5 pour 100 de moins que l'inflation soit un effort de 9 milliards tout ceci les conduira à diminuer leur investissement alors qu'elle soutienne à elle seule près de 70 % de la l'investissement public, or, contrairement à l'État, les collectivités ne peuvent se laisser aller à la facilité de voter un budget de fonctionnement en déficit, ni de le financer par la dette, contrairement à l'État, elles ont fait des efforts de gestion pour reconstituer leur auto-financement et aujourd'hui vous prenez argument de ses efforts pour les sanctionner, c'est leur bonne gestion que vous vous apprêtez à cent, à sanctionner cette méthode n'est pas la bonne, d'abord parce que le changement des règles permanent rend de plus en plus difficile une vision à long terme pour les élus locaux, ensuite parce que les collectivités ne mérite pas d'être les boucs émissaires d'un État incapable de s'engager, comme elle dans une véritable rationalisation des de sa gestion, ainsi qu'en témoigne le PS. à notre collègue Martine Filleul, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, toutes les enquêtes convergent pour dire que cette rentrée universitaire va être la plus chère de ces 20 dernières années, l'UNEF chiffre la hausse du coût de la vie étudiante à 400 euros avec les frais d'inscription qui explosent et le prix des pâtes, base de l'alimentation des étudiants qui augmente de 21 % en un an, 56 % des étudiants ne mangerait pas à leur faim 56 % à Lille, un tiers des étudiants vit déjà sous le seuil de pauvreté oui en France, les étudiants ont faim et l'inflation sonne comme un coup de grâce, pour eux, oui, en France, les étudiants ont froid, ils vont subir un nouvel hiver dans les logements du Crous délabré, encore moins bien chauffé cette année oui en France, les étudiants ont peur le traumatisme du distanciel resurgit des universités comme celle de Strasbourg prévoit une fermeture pour faire des économies d'énergie, peur également de format sup algorithmes opaques, il est honteux de la sélection en master, véritable épée de Damoclès, le gouvernement fait des annonces, mais elles sont sans commune mesure avec l'ampleur, la gravité et l'urgence de la situation, alors Madame la ministre, ma question est simple : les étudiants sont-ils encore une priorité pour ce gouvernement et quelle université voulons-nous pour demain. Pour on vous répondre, la parole est. Ah, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Madame Sylvie Retailleau. Mais la parole. Merci monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice d'abord je voudrais vous remercier de remettre ce point ah, merci, pardon, vous avez pas vu, j'étais de dos, ce qui s'est moi je voudrais vous remercier en cette rentrée avec le contexte de l'inflation, c'est une vraie question avez je vais directement répondre à votre dernière question, oui, les étudiants Castres au coeur de la priorité de notre gouvernement clairement au coeur, les étudiants et notre jeunesse, en partie déjà avant l'été par des mesures d'urgence qui sont appliquées actuellement je voudrais quand même vous les rappeler parce qu'il est bon que tous les connaissent le premier, vous avez parlé de l'augmentation des frais d'inscription, nous avons gelé les droits d'inscription, et ceci depuis plusieurs années, comme les gels des loyers des Crous ont été aussi gelé le second, c'est l'augmentation des 4 pour 100 de la revalorisation des bourses pour les boursiers, puis ensuite le 3 et demi pour les APL, dans le cadre des étudiants boursiers ou les étudiants qui ont aussi bénéficié d'aides annuelles du Crous ou tous les étudiants APL une aide exceptionnelle de solidarité de cent euros enfin le la suite du repas à un euros pour toute l'année universitaire, ce repas à 1 euros c'est cent euros d'économie par mois pour un étudiant, c'est plus de la moitié des étudiants qui sont touchés par ces mesures d'urgence à la rentrée et je voudrais passer un message, parce que je suis d'accord avec vous, c'est important, qui est aujourd'hui en précarité, il s'adresse au Crous et pour avoir accès au repas un euros et des être très vite rapidement et des aides d'urgence pour les problèmes énergétiques, le message est clair pour toutes les établissements pas au détriment des étudiants, pas de remise à distance des enseignements et pas de blocage de gros projets d'investissement de nos établissements, en particulier pour la rénovation thermique énergétique et pour le plan de sobriété les messages ont été passés et les établissements seront accompagnés au cas par cas pour que justement cela ne se reproduise pas, je vous remercie. Madame la Ministre, merci de votre réponse, mais malheureusement changer quelques paramètres, comme vous le suggérez n'est pas suffisant, je vous donne quelques exemples : 77 % des étudiants sont exclus de l'aide au repas, hein, un pour 100 et la majorité des boursiers un euro, et la majorité des boursiers perçoit le zéro bis, soit la somme dérisoire de 100 euros mensuels, il faut, madame la ministre, une refonte complète du système des bourses, comme le président Macron s'y était engagé en 2017 car le système des aides sociales aux étudiants est à bout de souffle, on ne peut pas plus longtemps faire l'économie de ne pas investir dans la jeunesse, merci. Merci monsieur le président, ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Monsieur le Ministre, ce matin vous avez ordonné l'évacuation du campement du crack, située dans le square force valent à Paris, le prolongement de la colline du crack cette colline de l'enfer annoncé comme une opération d'envergure dans la lutte contre la drogue dans la capitale, une question demeure : Monsieur le Ministre, où sont-ils allés où vont-ils aller seront-ils soignés, les opérations de ces dernières années ont montré que les consommateurs et leurs dealers changer d'endroit rapidement, souvent d'ailleurs, peu de temps avant le passage des forces de l'ordre cette situation reste un drame humain considérable pour ces centaines de personnes qui se droguent sous nos yeux à ceci s'ajoutent des scènes d'une violence inouïe, qui se déroule tous les jours dans la capitale, comme par exemple l'agression d'un bébé de policiers d'un pharmacien d'une opticienne d'une femme poussée sur sur les rails du métro et sans oublier tout dernièrement l'agression extrêmement violente d'un homme de 92 ans, roué de coups par une toxicomane, à Paris, c'est une évidence, le plan crack est un échec, le problème n'est pas traitée juste déplacé du 19ème au 18ème arrondissement ou inversement, alors Monsieur le Ministre que comptez-vous faire pour éradiquer définitivement le trafic et la consommation du crack à Paris. On nous réponde, la parole est au ministre de l'Intérieur, que le ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice en effet ce matin tôt, une à peu près un millier de policiers étaient dans le 19ème arrondissement de Paris pour procéder à la destruction après réquisition des services de la ville de Paris on pourrait appeler ça une ville je mets des guillemets parallèle : celle de la colline du crack, comme vous l'avez évoqué notamment du score de Forgeval mais également pour pouvoir interpeller les personnes qui passent leurs nuits, là vous savez qui sont à peu près 200 la nuit et à peu près entre 600 et 700 le jour tout dépend évidemment d'un certain nombre d'aléas, puisque nous avons compté jusqu'à 17 points de deal du krach et je voulais dire et dire que cette année, depuis le 1er janvier il y a eu 772 affaire faites par la police parisienne et dont 584 personnes interpellées ce qui montre à chacune et à chacun le travail qui était déjà fait auparavant, mais après m'en avoir couvert pardon auprès de Madame la première ministre, j'ai décidé cette opération qui permettra de laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut, des centaines de policiers à Paris entre la place de Stalingrad jusque les 2 villes d'Aubervilliers de Pantin pour empêcher vivement la reconstitution de ces villages, il s'agit pas de les déplacer, mais il s'agit évidemment de mettre fin à ce village de drogue ainsi ouvert il y a eu ce matin 211 contrôle de personnes 52 personnes étaient sous l'infraction à la législation sur les étrangers, en gros, il était irrégulier sur le territoire national, ils ont donc été conduits, ils sont en train d'être reconduit dans les centres de rétention administratif où nous parlons, nous avons réservé 70 places de pour pouvoir justement permettre de mettre ces personnes dans l'écrin et pouvoir les expulser du territoire national, 63 ont été mis à l'abri, notamment des femmes, particulièrement vulnérables 39 interpellations, dont 17 fiche de recherche monsieur le garde des Sceaux 6, infraction à la législation sur les stupéfiants, 11 personnes qui avaient des armes et un pistolet automatique d'ailleurs été retrouvé ce matin très tôt 5 hospitalisation d'office madame la sénatrice, l'État a pris ses responsabilités pour mettre fin à ceux des autres que les Parisiens ne pouvait plus accepter, il faut désormais qu'en lien avec bien sûr la santé, les collectivités locales, vous le savez bien, prennent aussi leurs responsabilités, c'est le sens des appels que nous avons eue avec madame la maire de Paris que j'ai prévenu hier, c'est le sens du travail que d'un 1er ministre et moi-même, appelons avec mon collègue de la Santé partenarial avec la région Île-de-France France avec la Ville de Paris pour que l'Ordre sont maintenus, bien évidemment, mais que le suivi sanitaire soit particulièrement maintenues également. Madame Dumas. Merci, monsieur le Ministre, bon je prends note de ces éléments qui sont censés répondre à l'inquiétude et à la colère, surtout des habitants des riverains, mais aussi à l'impatience des élus parisiens avec les élus du groupe changer Paris sous la présidence de Rachida Dati nous prendrons d'ailleurs une initiative lors du prochain conseil de Paris à cette occasion, nous comptons sur le plein soutien du préfet de police Laurent N'uñez d'autant que l'exécutif parisien a montré toutes ces dernières années son incompétence, son inefficacité en la matière, alors Monsieur le Ministre, votre responsabilité est grande, ne laissez pas perdurer dans notre capitale le plus grand marché à ciel ouvert de crack en France. La parole est à notre collègue Jean-Marc Boyer pour le groupe Les Républicains. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au ministre des Transports, il est 17 millions d'habitants du territoire auvergnat et du Massif Central, se désespère d'être les enfants pauvres des mobilités de la République, au point que, sur une carte et The Crown de la France, Marseille se retrouve au nord de Clermont-Ferrand en temps de trajet vers Paris, les ministres passent et les trains sont toujours très en retard sur la ligne Clermont Paris depuis de nombreuses années et de manière récurrente des incidents et des retards importants pénalise fortement la desserte de nos territoires auvergnat, cette situation était déjà inadmissible, elle devient totalement incompréhensible et révoltante, les retards ont été jusqu'à 17 heures oui 17 heures de retard en juillet dernier, monsieur le Ministre, comment pouvez-vous venir sur notre territoire, il nous dire la même chose, mot pour mot, que votre prédécesseur, il a 3 ans, sur le plan financier sur les travaux tant attendu en effet des améliorations nécessaires de la ligne n'avance pas, le calendrier n'est pas respectée et pire vous exigez désormais une étude environnementale qui retardera encore les travaux de 2 ans, alors qu'il manque déjà 130 millions d'euros pour l'électrification de la ligne, alors Monsieur le Ministre : envisagez-vous de respecter le calendrier initial et les financements des travaux prévus pour 2025.

car elle a connu historiquement d'importantes difficultés c'est exact et vous avez rappelé un épisode du mois de juillet qui a été particulièrement désagréable, j'ai changé à ce moment avec le maire et je me suis rendu dès le mois de septembre, en effet, à Clermont-Ferrand. Parce que cette ligne est importante, c'est la raison pour laquelle l'État engagé un effort absolument exceptionnel, ces dernières années qui est maintenu et qui est déployé, je veux le rappeler car aucun autre projet à par une autre ligne d'équilibre du territoire de même importance celle, Orléans, Limoges, Toulouse, qui les relie à Paris fait le le le fait l'objet d'un tel investissement, 2 milliards d'euros financé par l'État pour la modernisation, la régénération du réseau et pour la art le renouvellement intégral du matériel roulant, je le confirme, mais c'était le sens de ma visite à Clermont-Ferrand, ces engagements seront tenus il y a, en effet, je n'ai pas caché, des difficultés de calendrier l'autorité environnementale a exigé ce n'est pas le gouvernement, nous respectons les procédures législatives prévues par l'autorité environnementale, elle s'impose à nous tous et je déplore que cela ajoute une procédure, mais c'est ainsi, et nous devons le respecter néanmoins les délais qui seront seront ces délais supplémentaires qui seront ajoutés à l'a dit, à la suite de cette décision, autorité l'autorité environnementale seront précisées, je les partagerai en toute transparence d'ici la fin de l'année, mais ils n'empêcheront pas le déploiement notamment de l'intégralité du nouveau matériel roulant quant à la rénovation du réseau, elle est en cours de réalisation, et j'insiste, nous tiendrons là aussi nos engagements et nos financements il y a un dernier point qui est lié à la situation industrielle que vous connaissez, à la fois sur Paris, Orléans, Limoges, Toulouse et sur Paris-Clermont-Ferrand ce renouvellement est assuré par l'entreprise CAF qui produit en France et qui connaît des difficultés industrielles comme beaucoup d'entreprise je recevrai la semaine prochaine, le PDG de cette entreprise pour préciser les délais de livraison, en faisant un clin d'oeil bienveillant à ma visite du 15 septembre que je n'avais pas annoncé de d'éléments nouveaux, ma responsabilité c'est de tenir les engagements et de réduire les calendriers, nous le ferons et surtout en attendant d'améliorer la qualité de service, je m'y engage, et nous instaurons un comité de suivi mensuel qui s'installera à partir de la fin du mois d'octobre, avec tous les élus de toutes les sensibilités, j'espère que tout le monde y participera pour améliorer en termes de connexion de propreté de régularité qui s'est améliorée depuis le début de l'année, le fonctionnement de cette ligne, nous y sommes totalement engagée et je me rendrai de nouveau avant la fin de l'année à Clermont-Ferrand pour assurer suivi. Monsieur le Ministre, votre réponse est est décevante et n'est pas à la hauteur des attentes du territoire à ce désastre ferroviaire s'ajoute le le désengagement d'Air France qui a réduit ses vols pour Clermont-Ferrand de 8 allers-retours à 3 aller-retour aujourd'hui quel mépris pour notre territoire qui n'est pas à moins de 2 heures de la capitale en train pour cela, le TGV Paris-Orléans-Clermont Lyon doit aussi redevenir une priorité pour l'avenir économique du Massif Central, seul territoire dont desservi par une ligne à grande vitesse le président Rémy Pointereau de l'association LGV POCL il travaille très sérieusement alors Monsieur le Ministre, face à ce constat désespérant, je vous le demande avec gravité engagé avec tous les partenaires un véritable plan de désenclavement ferroviaire et aérien du centre de la France et du Massif c'est un cri, c'est une urgence. Nous en avons fini avec les questions au gouvernement, je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mercredi 12 octobre je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 pour les débats d'actualité sur le thème : atteinte aux droits des femmes et aux droits de l'homme en Iran, on a trop de la séance est suspendue pour 10 minutes.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat d'actualité sur le thème : atteinte aux droits des femmes et aux droits de l'homme en Iran. Madame la Ministre, mes chers collègues par ce débat, retenu par le président du Sénat sur le fondement des propositions des groupes politiques, le Sénat souhaite rappeler la mémoire de Mahsa Amini, décédé le 16 septembre dernier en Iran après avoir été arrêté pour une mèche de cheveux qui dépassaient de son voile et celle de 10 Najafi exécutés par la police parce qu'elle réclamait sa liberté en tant que femme et iranienne. Et puis. Nous souhaitons lors de ce débat, rendre hommage à l'ensemble des victimes de la répression du puissant mouvement de contestation en Iran et à toutes ces femmes et ces hommes qui revendique aujourd'hui leur liberté et nous saluons unanimement le courage. Je vous rappelle que dans ce débat, la faculté pardon s'il le juge nécessaire de prendre la parole immédiatement après chaque orateur. Pour une durée de minutes l'orateur disposera alors d'un droit de réparties d'une minute, le temps de réponse du gouvernement à l'issue du débat est limité à 5 minutes, Madame la Ministre, vous pourrez donc, si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura exprimé son expression. Dans le débat, la parole est à madame Annick Billon.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le 16 septembre dernier la mort de Masha Amini, âgé seulement de 22 ans après son arrestation par la police des moeurs pour avoir porté une tenue non appropriée, nous a profondément choqué depuis l'Iran connaît une contestation populaire d'une ampleur inédite des femmes, des hommes, la jeunesse iranienne manifestent chaque jour dans les villes d'Iran pour exprimer leur colère, le mouvement de contestation entre maintenant dans sa 3ème semaine et ne faiblit pas, tout comme la répression sanglante organisée par le pouvoir en place, les dernières nouvelles qui parviennent à sortir du pays malgré les coupures internet organisée par le gouvernement font état d'une centaine de morts et de plus d'un millier d'arrestations arbitraires, la police n'hésitent plus à entrer dans les universités pour réprimer les étudiants soupçonné d'apporter leur soutien à la lutte pour le droit des femmes, la persécution des femmes en Iran, perdure depuis de nombreuses années et si l'on a pu espérer quelques améliorations de leur statut sous Hassan Rohani, l'élection du président Ebrahim Raïssi a mis un terme aux espoirs de progrès en faveur du droit des femmes, dans son dernier rapport annuel sur l'Iran Amnesty International et sans concession la discrimination envers les femmes sont nombreuses, mariage, divorce employes succession ou encore accès aux fonctions pu politique les inégalités perdurent les droits des femmes et des filles sont bafoués par le régime iranien, par exemple, l'âge légal du mariage est toujours fixé à 13 ans et les pères peuvent obtenir des autorisations pour marier leurs filles à un âge encore plus jeune, le port du voile imposé par la loi est synonyme de harcèlement quotidien d'un d'invisibilisation des femmes de détentions arbitraires, d'actes de torture et d'autres mauvais traitements de la part des gardiens de la révolution. Ces contestations qui se sont levés à la mort de Masha Amini ne reflète pas seulement le recul du droit des femmes, mais dénonce tout un régime et ses abus femme vie liberté, nous devons faire notre ce magnifique slogan des manifestants et manifestantes qui ont le courage de défier le pouvoir en place pour mettre fin aux terribles discrimination dont sont victimes les femmes iraniennes, la communauté internationale, si elle est attachée à la défense des droits des femmes doit envoyer un signal fort et unanime pour soutenir cette contestation historique Madame la Ministre quelles actions en faveur de la contestation populaire iranienne, le gouvernement compte-t-il mettre en place ce sujet fera-t-il l'objet d'échanges lors de la réunion informelle des chefs d'état de l'Union des sanctions semble être en discussion, qu'en est-il. Et pour conclure, que penser de l'élection de l'Iran à la Commission de la condition de la femme de l'ONU en 2021 alors que la persécution des femmes en Iran, il est systématique, l'Iran a-t-elle vraiment sa place dans cette instance internationale dont le but est la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, faisons notre ce slogan femme vie liberté. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame, Esther Benbassa. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues en Iran depuis la mort de mars à un mini-interpellé il y a 3 semaines par la police des moeurs parce qu'une mèche dépassé de 100 foulard, la contestation ne retombe pas, elle touche l'ensemble du pays, la répression est féroce, le nombre des morts et des personnes arrêtées monte chaque jour et les revendications dépassent la seule question du port du voile ce sont désormais le Guide suprême et le régime qui sont remis en question, de son côté que fait la France, notre président se drape dans un silence opportuniste, on ne touche pas trop à l'Iran utiles en cette période de guerre à l'Est avec le probable retour sur le marché international de ce grand vendeur de pétrole que l'Iran lors de son entretien à New York avec le dirigeant ultraconservateur iranien Ebrahim Raïssi en marge de l'assemblée générale de l'ONU, le président de la République a juste demandé une enquête transparente sur la mort de Marsa, les échanges se concentrant sur le dossier nucléaire iranien. Actuellement, les manifestants, femmes et hommes s'organise, parti ce qui est à la fois leurs forces et leurs faiblesses cette spontanéité fait que des cinéastes, des athlètes, des musiciens, des artistes expriment leur solidarité le pouvoir annonce qu'il s'en prendra aux célébrités qui ont soufflé sur les braises, le réalisateur Asghar Farhadi 2 fois oscarisé lui a invité tous les artistes, cinéastes, intellectuels, militants des droits civiques du monde entier à exprimer leur solidarité et l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi d'insister : il faut envoyer un signal fort en en France, une cinquantaine de personnalités d'artistes femmes ont déjà hier diffusé une vidéo où elle se coupe une mèche de cheveux en soutien aux femmes iraniennes j'appelle tout le milieu artistique français et les personnalités à rejoindre largement cette mobilisation quant à nous, les politiques au-delà des protestations d'usage ne devons-nous pas faire pression avec vigueur et conviction sur les l'exécutif pour pour qu'il sorte de sa frilosité. Mobilisons nous évitons surtout d'instrumentaliser la lutte des Iraniennes pour régler nos différends intérieur sur la question du voile en France, l'enjeu de nos engagements et la la liberté et les droits humains, je regrette qu'il n'y a pas assez de monde. Aujourd'hui où il est nécessaire de se mettre d'accord et faire des actes symboliques, pour montrer notre soutien aux Iraniens et aux Iraniens merci. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Guilaine Pantel pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Dans un 1er temps au nom du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, nous tenions à remercier les organisatrices et organisateurs de ce débat d'actualité oh combien fondamental pour quiconque se réclame de l'humanisme. à plus ou moins 5 heures d'avion de Paris, la mort de la jeune Mahsa Amini à 22 ans le 16 septembre dernier a déclenché un grand mouvement de libération des femmes et de contestation contre le régime autoritaire de la République islamique d'Iran, la disparition de la jeune fille d'origine kurde est le fruit d'une arrestation violente de la police locale des moeurs et ayant pour motif un port de vêtements inappropriés, le journal de d'opposition en exil Irak International a révélé un scanner de son crâne mettant en évidence une fracture osseuse une hémorragie et un ODM cérébral compatible avec un passage à tabac, se rappelle de cette tragédie est fondamental pour prendre la mesure de la mécanique infernale d'oppression instaurer dans ce pays. Voilà donc où nous en sommes, ou lorsque l'on parle d'atteinte aux droits des femmes et aux droits de l'homme en Iran aujourd'hui un état totalitaire et répressif selon plusieurs organisations non gouvernementales, les femmes, les personnes LGBT et les membres de minorités est technique, pardon, ethniques ou religieuses font face à des violences et à une discrimination quotidienne dans toutes les sphères de la société. Avec naturellement l'approbation et l'encouragement des autorités politiques et religieuses dans les relations sont particulièrement poreuse. Les observateurs constatent également des atteintes au droit et à la vie à la liberté d'expression, d'association et de réunion, l'interdiction de partis politiques indépendants de syndicats et d'organisations de la société civile, la censure et des médias sont monnaie courante. Du côté du système judiciaire, l'égalité devant la loi, la séparation des fonctions le secret de l'instruction, les droits de la défense la présomption d'innocence, la possibilité de voie de recours et le principe du contradictoire, ils sont totalement piétiner. Aussi la peine de mort, il est pratiquée impunément à l'issue de procès grotesque. Face à ces données et au contexte de mobilisation citoyenne évoqué au début de mon intervention, nous ne pouvons qu'éprouver une certaine stupeur au regard des informations qui nous parviennent au compte-gouttes, en effet, bien que l'accès aux réseaux sociaux soit devenu presque impossible en Iran depuis le début de la contestation des images et des vidéos édifiante parviennent à franchir la censure et souligne le danger auquel les manifestants s'opposent en descendant dans la rue. Mais au-delà du caractère émotionnel que cela provoque à juste titre, notre pays se doit d'être à la manoeuvre pour promouvoir les valeurs que nous portons fièrement dans notre devise républicaine, le 1er réflexe doit être un message d'unité et de solidarité dans le combat pour les droits des femmes à disposer de leur corps à arborer leur chevelure à interrompre une grossesse non désirée à circuler librement à accéder au marché du travail, et bien d'autres, il s'agit de combat universel des femmes contre par un patriarcat qui tue, mutile et blesse psychologiquement le 2ème réflexe doit s'inscrire dans une stratégie diplomatique au niveau européen et international, pour apporter un soutien plus concret aux populations hein d'Alger. Pour ce faire, nous devons, avec une très grande précaution, des mesures restrictives car elles peuvent produire l'effet pervers d'appauvrir les plus fragiles. à titre d'exemple, l'accorde une protection ici ou dans d'autres pays européens nous semble être cohérent avec des risques avérés de persécution cette protection dans s'exécuter jusqu'à ce qu'il y a une mise en conformité du droit interne iranienne avec le droit international. En outre, la saisie du Conseil des droits de l'homme et des Nations-Unies paraît adéquate pour ouvrir une enquête indépendante sur place afin de recueillir des preuves des agissements du régime à l'encontre de son peuple et d'engager des poursuites en temps utile. Ce recueil de preuves d'exactions peut aussi être facilitée, via une stratégie d'offensive numérique Anne accompagnera les initiatives permettant à la population de retrouver un accès normal à Internet et de communiquer avec le reste du monde. Pour conclure simplement mon propos, je dirais que, quelles que soient les mesures engagées par notre pays la France leur finalité doit être l'humaine d'abord et femme vie liberté.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers. Collègues le 16 septembre pour avoir mal porté son voile dans les rues de Téhéran, une jeune femme, Mahsa Amini est morte aux mains de la police des moeurs pour avoir mal porté son voile la futilité confondant des raisons. Qui ont mené à son décès de Laurent que plus révoltant plus avilissant pour ceux qui s'en sont rendus coupables ce drame vient rappeler au monde s'il en était besoin, la réalité de ces millions d'Iraniennes qui vivent sous le joug de la révolution islamique, il expose aux yeux de tous la brutalité des sbires de ce régime anachronique qui considère littéralement au travers de la il y a que la vie d'une femme ne vaut que la moitié de celle d'un homme. Mais il souligne également le profond mépris des mollahs pour les minorités du pays dont les cultures non depuis longtemps plus droit de cité en Iran car Mahsa Amini en plus d'être une femme avait un autre tort : celui d'être sa mort aura été l'étincelle qui a fait s'embraser la contestation qui couvait, d'abord dans sa région natale du Kurdistan puis presque immédiatement à Téhéran à Mechhed 2ème ville du pays, et comme une traînée de poudre dans tout l'Iran, la mobilisation n'a cessé depuis cette révolution des femmes comme certains n'hésitent pas la nommer, engendre des scènes que nous aurions tous cru impensable il y a encore quelques semaines, des Iraniennes qui descendent en masse dans la rue, tête nue sous les acclamations de la foule des Iraniennes qui se coupe les cheveux qui brûle ce voile qui a coûté la vie à l'une des leurs. Et qu'illustre plus que tout autre symbole le statut d'infériorité dans lequel a voulu les enfermer un Islam rigoriste. Et théocratique des femmes iraniennes qui sont, il est fondamental de le souligner aujourd'hui soutenus et accompagnés par les hommes iraniens le rappel qui s'exprime au cri de femme vie liberté et plus qu'un cri de colère s'ans Roger, bien sûr, mais c'est aussi un projet, car ce sont des valeurs ces valeurs qu'elles incarnent là-bas avec un courage étourdissant et que nous défendons ici parfois bien timidement face aux coups de boutoir, qu'elle ne cesse de subir ces dernières années, alors qu'elle peut être l'issue de ce mouvement, nous nous rappelons les grandes manifestations de 2017 puis de 2019 qui déjà avait violemment remis en cause le pouvoir en place il y a dans les émeutes d'aujourd'hui qui sont à la fois d'une ampleur plus importante et d'une nature plus profonde le vacillement d'un régime contesté dans son essence et les prémices de son effondrement, une certitude, c'est né à moins rapidement imposé la réponse des autorités sera féroce et ne fera pour reprendre les mots du chef du système judiciaire iranien preuve d'aucune indulgence, elle s'est déjà traduite par des milliers d'arrestations, des dizaines de morts et des centaines de blessés et pour ajouter à l'intolérable, elle menace désormais la stabilité régionale en projetant la violence au-delà du territoire iranien, Téhéran a ainsi pris prétexte de la crise pour frapper à coups d'artilleries de drônes et de missiles balistiques, les locaux des partis d'opposition Kurdes réfugiés de l'autre côté de la frontière irakienne est accusé de souffler sur les braises de la contestation contre le régime, le gouvernement iranien vient en outre de lancer un avertissement sans équivoque à ceux qui, dans les médias, ont pris fait et cause pour le mouvement qu'il s'agisse de journalistes, d'acteurs de musiciens ou de sportifs, on pense notamment à ses joueurs de l'équipe nationale de football qui avait asséné publiquement cette phrase lourde de sens, les cheveux de nos filles sont recouverts dans un seul cette répression est avant tout une meurtrissure faite au peuple iranien, mais elle est aussi une nouvelle insulte aux valeurs de liberté, de dignité que nous avons en partage avec les manifestantes et les manifestants d'Iran nous ne pouvons donc rester sans réaction et nous tenir à l'écart de ce qui est plus qu'un simple soubresaut de l'histoire, même si nos moyens d'action, il faut bien le reconnaître, sont très limitées, il est probable que l'Union européenne adopte des sanctions, comme elle le fait régulièrement, chaque nouvelle violation grave des droits de l'homme en Iran malgré leur absence prévisible d'effet concret, il est indispensable que de telles mesures soient prises car nous ne pouvons plus nous contenter des nécessaire condamnation de principe Émile jusqu'à présent la France Madame la Ministre, devra jouer un rôle majeur dans ce processus européen, mais aussi dans la mobilisation internationale en oeuvrant à ce que toutes les instances compétentes des Nations-Unies se saisisse d'urgence de la situation iranienne, cela ne suffira sans doute pas infléchir le cours des événements et encore moins la nature profonde du régime iranien, mais il est essentiel que ce dernier mis sous pression à l'intérieur le soit également à l'extérieur, il est surtout fondamental que les Iraniennes puisse sentir qu'elles ne sont pas seuls, qu'elle sache que le monde les regarde et qu'il est à leurs côtés, il faut en d'autres termes faire nous. Pour le précepte du philosophe Ali Charia, cité par le prix Nobel iranien de la paix Chirine Ebadi, dans son ouvrage La cage dorée, si vous ne pouvez éliminer l'injustice au moins racontez là à tous, je vous remercie.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le temps des dictateurs est revenu. Les démocraties au terme d'une lutte implacable avait vaincu au XXe siècle, les 2 totalitarisme aux dizaines de millions de morts. Certains les croyait disparu à jamais sous nos yeux l'international des tyrans se reforme le boucher de Moscou le génocidaire des Ouïgours en Chine, le Docteur Folamour de Corée du Nord, le massacreur de femmes de Téhéran et quelques autres se sont regroupés, leur seul but : se venger abattre l'Occident, mettre à bas la liberté, et d'abord celle des femmes. Le pire est que, comme aux siècles précédents, ils ont des alliés dans nos propres pays les adorateurs de Poutine, indifférent au massacre des Ukrainiens, les complices de Chick qui se moque des Ouïgours et de Taïwan, les alliés de Khamenei, expliquant au moment où les iranienne Mehr que le voile essayant en un mot, les populistes de tous bords qui partagent une idée fixe avec les despotes la haine de la démocratie. Depuis le début de la révolte en Iran et jusqu'à la manifestation de dimanche dernier à Paris, ces professionnels de l'indignation ceux qui battent le pavé chaque semaine pour crier que la police tue ou dénoncer le racisme systémique en France avait disparu, où étaient-ils lors des 2 premiers rassemblements en soutien des femmes iraniennes en week-end, sans doute, comme lors des manifestations pour l'Ukraine leur compte Twitter qui dénonce chaque jour le patriarcat et l'islamophobie sont devenus muets, pas un mot de soutien pas un appel contre la monarchie et sa police des moeurs pendant qu'à Téhéran, les femmes meurent sous les coups et les balles, il préfère dénoncer le virilistes du barbecue, faire l'éloge d'un gifle heures ou juger les harceleurs dans des comités de transparence qui sont l'oxymore le plus grotesque inventé depuis la dictature du prolétariat, quelques-uns d'entre eux ont réapparu dimanche dernier lors du rassemblement place de la République à Paris, les Iraniens et les Iraniennes. Présent leur en donner une grande leçon de laïcité en signifiant à Madame Rousseau, qu'elle n'était pas la bienvenue, ils ont rendu clair pour tout le monde cette évidence, on ne peut en même temps être pour le voile à Paris et défendre celles qui brûlent leur voile à Téhéran en sifflant madame Manon Aubry. En sifflant madame Manon Aubry, ils ont signifié qu'un parti ne peut, en 2019 marcher avec les islamistes, et en 2022, soutenir les victimes de la république islamiste en un mot, ils nous ont montré qu'on ne peut être à la fois communautaristes et universalistes, il faut choisir en Iran des femmes risquent leur vie pour se débarrasser du voile ici les intersectionnelle se présente le présente comme une liberté, écoutons ce que leur répond Chantal de heures le voile n'est pas un objet cultuel mais un objet politique, c'est le produit phare de l'islamisme, et c'est désormais une affirmation anti-occidentale et anti-démocratique, fin de citation ce morceau d'étoffe Bourguiba l'appeler l'épouvantable chiffon aux naïfs qui croient que se voiler est un choix oh des coloniaux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, il faut rappeler que la lutte contre le voile n'est pas une oppression néo-coloniale, mais que les grands dirigeants musulmans qui avait compris que la soumission de la femme était l'une des causes principales du déclin de leur pays l'ont tous combattu Atatürk le 1er qui l'a interdit dans les années 20 en Turquie Reza Shah dans les années 30 en Iran Bourguiba plus tard en Tunisie, Nasser en Égypte s'en moquer publiquement devant le grand mufti d'Al-Azhar ce combat qu'ils avaient gagné a été perdue depuis la révolution islamique de 1979 les femmes iraniennes reprennent toujours de ce flambeau contre les mollahs les ayatollahs les dictateurs les talibans et leur police des moeurs, c'est un coup de poignard dans le dos de ses combattantes confond ce certaines néo-féministe en condamnant toute critique du voile au prétexte de ne pas nourrir l'islamophobie, un coup de poignard dans le dos, lorsque Sandrine Rousseau déclare que le voile peut être un embellissement ou que Rokhaya Diallo ose affirmer que la liberté peut être aussi dans le hijab combien faudra-t-il de morts à Téhéran pour que l'héroïsme des Iraniennes les forces à ouvrir les yeux et les oreilles pour qu'elle cesse de danser le Moonwalk de Michael Jackson, en faisant semblant de faire avancer la cause des femmes tout en la faisant reculer le 21ième siècle s'annonce aussi dangereux que le précédent, il est temps de s'en rendre compte, ceux qui croient que nous ne sommes pas en guerre ou qui, pour se rassurer, se force à le croire, font une erreur tragique car les dictateurs et les ayatollahs, eux, savent qu'ils sont en guerre contre nous, puissent les admirables femmes iraniennes-les héroïques soldats ukrainiens et les courageux dissident chinois nous convaincre de nous rallier à leur crient Liberté je vous remercie. Merci, cher collègue, et la parole est à maintenant hein Madame Mélanie Vogel. Monsieur le président, chers collègues, je vais me permettre de commencer par quelques mots qui ne sont pas de moi pour danser dans la rue pour toutes les fois où nous avons peur de nous embrasser pour ne plus avoir honte d'être pauvre pour l'enfant qui, jusque dans ses rêves doivent fouiller dans les poubelles pour respirer un air pur pour les arbres qui meurt pour ses larmes qui ne cesse de couler pour les étudiants pour leur avenir pour les enfants afghans pour cette petite fille qui rêve d'être un garçon pour femme vie liberté ces paroles sont celles d'une chanson de gerber naïf pour emprisonner quand il a publié une chanson qui n'a pas composé qu'il n'a pas composé puisqu'elle est formée à partir de tweets postés courageusement par celles et ceux qui se dressent en Iran contre l'oppression, elle démontre une chose, une chose qui est insupportable pour le pouvoir en place ce qu'il se passe en Iran aujourd'hui est profondément différent de ce qui a pu se passer lors des dernières révoltes parce que, précisément, ce n'est pas une révolte, on a déjà vu dans le passé une partie de la société iranienne plutôt la jeunesse des villes courageuse engagée se mobiliser, nous avons aujourd'hui à faire et quelque chose d'une toute autre dimension, on a là un mouvement de masse, guidés par des femmes qui est en train d'agréger tout ce que la société iranienne compte de personnes qui veulent être libres et vivre dignement les femmes oui, les femmes d'abord, puis les hommes aussi les minorités ethniques, politiques, religieuses, sexuelles de genre : les jeunes qui ne voient pas d'avenir, les pauvres qui ne peuvent pas survivre dans un pays où l'inflation et de plus de 40 % les universitaires qui ne peuvent pas enseigner les paysans qui ne peuvent pas cultiver leurs champs à cause de la gestion désastreuse de l'eau, toutes celles et ceux qui, au fond, veulent simplement respirer vivre, aimer le féminisme, la lutte féministe déploie en ce moment même en Iran et je pèse mes mots, sa puissance révolutionnaire, ce qui est en train de se passer en Iran n'est pas une révolte, c'est une révolution, une révolution pour la démocratie, pour la justice contre la tyrannie religieuse, une révolution pour les femmes, pour la vie et pour la liberté et une révolution, ça ne se calme pas, ça ne se passe pas une révolution, une révolution, ça se fait, ce sont donc les femmes qui entraîne et entraîneront un jour ou l'autre je ne sais pas quand la chute de ce régime, ce sont les femmes qui en luttant pour leurs droits pour leur liberté trace en ce moment même le chemin des droits et des libertés tout court, ce sont les femmes qui en réclamant l'égalité pour elles peuvent conquérir l'égalité tout court, ce sont les femmes aujourd'hui, on entend souvent, en France et ailleurs dans le monde que les féministes mènent des combats marginaux que les luttes des femmes sont secondaires qu'il y a mieux à faire, et plusieurs gens que la vraie, la grande la sérieuse politique, c'est autre chose, les Iraniennes qui, au prix et au risque de leur vie brûlent leur foulard dans la rue, danse dans la rue, hurle à la fin de la dictature, les Iraniens font en ce moment même la démonstration puissante bouleversante et irréfutable que dans notre monde, ce sont les combats des femmes qui sont l'avant-garde des combats pour toutes et tous, les valeurs pour lesquelles se battent les Iraniennes et les Iraniens réprimé dans le sang, ne sont pas des valeurs occidentales importée des États-Unis ou d'Israël, ce sont des valeurs bien ancrées en Iran, ce sont leurs valeurs et nous les partageons aussi face à cette révolution face à cette répression dans le sang, face à ces morts pour la liberté, nous devons bien sûr relayé leur voix, bien sûr, mais nous devons aussi agir, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine le 24 février le soir même, les dirigeants européens se réunissaient et s'accorder sur un 1er train de sanctions après l'invasion, entre en vigueur dès le lendemain, le 25 février nous sommes au 19 jours de cette révolution, cela fait 19 jours qu'un régime est en train de massacrer son peuple et aujourd'hui pas grand chose, les négociations sur le nucléaire iranien continue comme si de rien n'était, il n'y a pas au niveau européen, de nouvelles sanctions on entend qu'on pourrait être en train d'en préparer pour la prochaine réunion du conseil des ministre des Affaires étrangères, le 17 octobre le 17 octobre c'est un mois après, ce n'est pas possible, il faut agir et comme cet après-midi, nous ne pouvons que débattre entre nous parler, je vous propose de faire au moins une chose que nous pouvons faire ici au Parlement français, sans rien craindre écoutez faire écouter quelques instants 7ème ne révolutionnaire qu'en Iran, on n'a pas le droit d'entendre librement.

je vous remercie.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le 16 septembre dernier une jeune femme de 22 ans est morte alors qu'elle était aux mains de la police des moeurs iranienne pour port de vêtements inappropriés. Depuis cette date, les femmes et la jeunesse iranienne se soulève massivement dans la rue et dans les universités pour crier une révolte légitime en réponse l'appareil sécuritaire iranien réprime ces manifestations avec brutalité, si nous sommes toutes et tous se réunit aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est parce que cette arrestation, la mort de Mahsa Amini et la répression de ces manifestations nous choque profondément et que nous les déplorant alors d'aucuns pourraient penser que débattre de l'atteinte aux droits des femmes et aux droits de l'homme, à 5000 kilomètres de Téhéran, comme nous le faisons aujourd'hui est inutile et vain je pense tout le contraire, car c'est la liberté dont il est question. Je veux croire que la liberté n'est jamais acquise, je veux croire que la liberté ne se décrète pas, mais qu'elle s'exerce et qu'il est important que l'on en débatte encore ici aujourd'hui si ce débat nous permet de condamner la mort de Mahsa Amini et la répression violente des manifestations qui s'en est suivi, il est surtout l'occasion de rappeler que le combat pour la liberté que le combat contre les violences faites aux femmes est loin d'être gagné aussi la France doit-elle utiliser toute l'influence dont elle dispose pour promouvoir l'universalisation de la Convention d'Istanbul au Conseil de l'Europe, qui représente aujourd'hui l'instrument international le plus abouti dans cette lutte indispensable contre les violences faites aux femmes, sans doute faut-il aussi avec nos partenaires européens envisagé la possibilité de recourir au régime de sanctions de l'Union européenne en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, en tant que sénatrice des Français de l'étranger, comment ne pas évoquer les quelques 1500 de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui en Iran, parmi eux plus de 80 % sont des binationaux, or vous le savez peut-être, mais l'Iran ne reconnaît pas la double nationalité, autrement dit ces binationaux qui sont retenus ne peuvent pas bénéficier de l'assistance consulaire de la France, le contexte actuel fait que cette communauté binational qui est naturellement très sensible à la question des droits de l'homme et des droits des femmes et, particulièrement, exposées. Elle court le risque d'une arrestation. D'une détention arbitraire et d'un jugement inéquitable, ces derniers jours la presse s'est d'ailleurs fait l'écho de l'annonce du ministère iranien des Renseignements, affirmant que 9 ressortissants étrangers auraient été arrêtés, dont au moins un Français. Je veux ici relayé la vive inquiétude de la communauté française en Iran et dire que la France doit tout mettre en oeuvre pour protéger ses ressortissants, notre groupe condamne fermement l'arrestation et la mort de Mahsa Amini, ainsi que la répression violente des manifestations qui a lieu aujourd'hui en Iran, il soutient vivement cette demande de liberté des femmes iraniennes, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à Madame Marie-Arlette Carlotti. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chères et chers collègues, le sang coule en Iran, et c'est d'abord le sang des femmes, la révolte que connaît l'Iran depuis 3 semaines, porte le nom de Mahsa Amini, morte le 16 septembre après avoir été arrêtée à Téhéran, parce que son voile couvrait mal ses cheveux, elle avait 22 ans et son visage martyr est devenu le symbole puissant de l'iniquité et de la brutalité du régime iranien, les images qui nous parviennent, nous serre la gorge, elle qui arrachent leur voile pour le jeter au feu, elle qui coupent leurs cheveux et qui brave la police des moeurs et elle qui entonnent Bella ciao ce Champ déjà émouvant lui-même quand il évoque le courage et l'esprit de résistance devient complètement bouleversant lorsqu'il est entonné par les iranienne dont les soeurs descendent dans la rue pour dénoncer l'obscurantisme du régime, au risque d'y laisser leurs propres vie en février 79 même, avant même l'instauration de la République islamique d'Iran, l'ayatollah chromé ni déjà la liberté de la femme comme le principal obstacle à son projet politique en les uniformise en par l'obligation d'abord du port du voile, puis par un manteau puis par un code couleur, on a voulu réprimer leur identité, les transformer en nombres d'elles-mêmes les priver de leur statut social et le les les relégués aux confins de la vie publique et depuis l'élection de l'ultraconservateur Ibrahim Raïssi en juin 2021 depuis que l'aile la plus dure, a mis la main sur le système, la situation des femmes s'est encore dégradée pendant toutes ces années d'horribles crimes ont été commis contre les femmes, le vitriol pour refus de mariage, la décapitation pour soupçon de flirt la lapidation pour délit d'adultère, la femme a été sacrifié au nom de l'honneur, l'honneur de l'homme, l'honneur de la famille de la société de l'État, mais elles n'ont jamais baissé les bras, aujourd'hui elles sont aux avant-postes du soulèvement, car elle ne supporte plus ce voile qui les entrave et au fil des jours ça te révolte féministe a pris une autre dimension, celle de la contestation du régime théocratique le soulèvement a d'abord touché des étudiants parce que ce sont toujours eux qui sont les plus prompts à réagir, puis il a gagné toutes les catégories sociales, toutes les villes toutes les provinces et les protestataires aujourd'hui descendent dans la rue, au nom de Mort au dictateur et en ce sens je crois moi aussi que le mouvement est assez différent de ce qui s'est passé en 2017 et 2019 désormais le renversement du régime des mollahs et réclamé et leur système corrompu corrompus, alors qu'il y a entre 50 et 80 % de la population, selon les territoires qui vit en dessous du seuil de pauvreté, les femmes sont opprimés en Iran, mais pas seulement les femmes, tout le monde, tout le monde : les avocats sont emprisonnés les manifestations d'enseignants sont réprimer la liberté d'association entraver la liberté de la presse n'existe pas, le rapporteur spécial de l'ONU, a dénoncé la situation des minorités, il se dit alarmé par le nombre d'exécutions arbitraires en partie Culié envers les Baloutches et les Kurdes, la République islamique qui a pourtant hérité d'un empire pluriethnique, cet employé a repris à réprimer toutes les revendications régionales, elle défend un centralisme autoritaire réfractaire aux minorités et elle développe comme contre toute forme d'opposition, la violence d'État dans les prisons iraniennes on côtoie toutes les composantes de la société civile, les militants politiques, les syndicalistes et les enseignants, les cinéastes, des journalistes, vous en avez parlé et depuis l'arrivée au pouvoir de Raïssi c'est l'escalade, encore plus, des arrestations arbitraires, la population est excédée par les privations de toutes sortes et Aspire à plus de liberté, alors le régime, c'est que, une nouvelle épreuve l'attendent : Tôt ou tard, ça va être la succession du guide suprême cet octogénaire à la santé chancelante, qui trouve quand même suffisamment d'énergie pour condamner la communauté internationale et nous accuser d'ingérence dans ce contexte, ils sont peu rempli peu enclin à discuter la police répond par la violence, elle recourt, semble-t-il, aux armes létales et à chaque manifestation, elle le tu, moi je ne sais pas ce que va devenir ce mouvement de révolte est ce qui va porter la révolution, je ne sais pas attends les leaders des oppositions de toutes les oppositions ont été emprisonnés, tués, poussé à l'exil, mais ce que je sais, c'est que ces femmes font preuve d'un incroyable courage et que l'on se doit nous, responsables politiques, d'être à la hauteur, nous avons été un peu lâche pendant ses 43 ans, d'oppression, la France et l'Union européenne doivent parler plus fort, Madame la Ministre, pour dénoncer cette répression sanglante, vous avez proposé le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, où en est-on est-ce que ça va se réaliser alors que le régime se sert des négociations sur le nucléaire iranien pour obtenir le silence de la communauté internationale, en tout cas moi ce que je sais, c'est que la France doit rester dans son rôle, c'est-à-dire la défense de ceux qui se battent pour la liberté, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est au président, Pierre Laurent, pour cinq minutes également. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, femme vie liberté depuis 3 semaines, c'est le cri de colère et d'espoir qui retentit dans les rues iraniennes ce cri de dignité et d'humanité, je veux évidemment le saluer avec émotion au nom de tout notre groupe, cet appel à la liberté, nous devons le soutenir de toutes nos forces le 16 septembre Masha Amini a été odieusement assassiné par la brigade des moeurs cet instrument d'oppression du régime des mollahs, elle est devenue le symbole de la révolte populaire son Crime : avoir mal porté le foulard symbole de la soumission imposée aux femmes par le pouvoir théocratique à la tête de la République islamique d'Iran depuis 1979 les femmes iraniennes n'ont cessé d'être exposés aux violences sexistes et patriarcales aux violences d'un régime politique et religieux obscurantistes qui a fait de la domination des femmes, un instrument de la domination sur toute la société, la situation s'est encore empiré depuis l'arrivée aux affaires de l'ultra-Ebrahim Raïssi en 1000 en 2021 ainsi des médias iraniens révéler encore récemment l'intention de recourir à l'Intelligence artificielle pour identifier les les femmes non ou mal voilées les sévices et les humiliations frappe toute la société iranienne, elle s'exerce contre femme violemment et aussi contre de larges fractions du peuple contre la population kurde contre la jeunesse qu'on prend toutes les forces du mouvement ouvrier au profit exclusif des cercles dirigeants du pouvoir et d'oligarchie prédatrice qui les soutiennent face aux femmes qui jettent avec courage leur foulard qui les brûlent qui se coupe les cheveux face à la Jeunesse, femmes et hommes qui se joignent au mouvement, la répression, et cette fois encore, féroce, on dénombre des dizaines de morts, des milliers d'arrestations arbitraires ce soulèvement des femmes iraniennes est un signal de courage et d'espoir pour les femmes du monde entier en lutte contre les oppression sexiste et patriarcale religieuses ou non, pour les femmes kurdes en lutte dans tous les pays de la région, notamment dans la Turquie voisine pour les femmes d'Afghanistan, d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe pour les femmes, filles victimes du viol utilisé comme une arme de guerre sur toute la planète pour les femmes victimes des réseaux mondiaux de prostitutionnel mis à nu par le remarquable rapport du Sénat pour les femmes du monde, en lutte contre toutes les violences sexistes et contre les attaques qui s'amplifie contre le droit à l'IVG, notamment en Europe et aux États-Unis, oui, la lutte des femmes en Iran est partie prenante de ce mouvement mondial pour libérer toute l'humanité des dominations sexistes et patriarcales elle a notre plein soutien, les femmes en Iran ne secoue plus seulement leur voile, elle secoue aujourd'hui le régime politique répressive d'une théocratie obscurantiste qui étouffe la civilisation de ce grand pays de 84 millions d'habitants depuis 10 ans, des mouvements de contestation des politiques sociales du régime ont déjà secoué le pays en 2009 2017, 2018, 2019 aujourd'hui se joignent au mouvement des femmes d'autres secteurs de la société pour dénoncer la dictature politique de ce régime, le peuple iranien ne veut plus de ce carcan dictatoriale l'Iran connaît de profondes mutations sécularisée son peuple a cessé d'élever son niveau de l'éducation, en particulier chez les femmes, quand ses structures politiques, elles se sont fossilisés la paix du monde a besoin d'un Iran qui retrouve la voie de la démocratie et de la justice sociale, force est de constater que la mise au ban de l'Iran par les États-Unis avec le retrait unilatéral en 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien et les sanctions américaines ah et non combattu la radicalisation répressif du régime qui se déchaînent, aujourd'hui contrôlée femmes tout le peuple iranien paye cher une terrible crise économique auquel s'ajoute le lourd tribut du Covid 19 : un jeune sur 4 est au chômage la moitié de la population a plongé dans la pauvreté, madame la Ministre, la solidarité avec les femmes d'Iran. Nous devons l'inscrire tout autant dans la lutte mondiale pour l'émancipation des femmes, contre tous les obscurantismes comme dans la lutte pour un nouvel ordre mondial juste, dans lequel le peuple d'Iran puisse trouver la voie d'un développement démocratique juste solidaire en paix avec ses voisins, la France doit agir clairement dans ce sens, comme le dit le proverbe iranien quand la corde de l'injustice grossit outre mesure, elle se déchire puisse toutes ces injustices se déchirer et le plus tôt sera le mieux.

Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la mort de Mahsa Amini quelques jours après son arrestation pour port de vêtements inappropriés et l'élément déclencheur d'un mouvement plus global de contestation du régime en place son nom est devenu un symbole de ralliement pour tout le peuple iranien désireux de vivre dans un état de droit, depuis la révolution de 1979 ces femmes et ces hommes subissent les pressions d'un pouvoir autoritaire et répressif, comme le rappelait ma collègue Annick Billon et beaucoup d'entre vous l'instauration de leur constitution les a privés d'une grande partie de leurs droits les plus absolu et fondamentaux cette mainmise des autorités sur leurs droits et renforcé par le recours à la censure, l'accès aux médias et réseaux sociaux, il est très restreint, cet été, le Parlement a précipité la préparation d'une proposition de loi pour ériger en infraction, la production et la diffusion d'outils permettant de contourner la censure ainsi des milliers de personnes ont été interrogées poursuivi ou détenu et des centaines d'autres sont emprisonnés, simplement pour avoir exprimé leur conviction, parmi eux, des journalistes, des artistes, des avocats ou des enseignants comme la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdel cas condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale ou aux chercheurs suédo- iranien Ahmad Reza Jalali, condamnés à mort, la violence est admise et systématique et la peine de mort est devenue un instrument de répression des dissidents et minorité aujourd'hui les contestations provoquée par la mort de Mahsa Amini ne cesse de prendre de l'ampleur, les universités sont devenues le théâtre de violents affrontements, enseignants et étudiants, ils sont particulièrement exposés des vidéos témoignent de la violence des répressions et arrestations, alors que les étudiants scandaient les étudiants préfèrent la mort à l'humiliation, la répression est menée jusqu'au coeur de la prestigieuse université Sharif à Téhéran, selon des témoins cités par le site d'information indépendant Iran-Wire dimanche dernier, des étudiants ont été battus, d'autres ont essuyé des tirs lors de l'intrusion des forces de police qui ont bouclé le bâtiment armés de paintball de gaz lacrymogène et de fusils à pompe, plusieurs jeunes seraient blessés si une partie des étudiants alors pu quitter l'université, d'autres sont restés bloqués à l'intérieur des témoins attestent avoir vu des arrestations de plusieurs dizaines d'étudiants et professeurs des vidéos circulent montrant des jeunes cagoule noire sur la tête, embarqués dans des fourgons de police. étudiants et professeurs de nombreux pays ont exprimé à la suite de ces mouvements inqualifiable, leur colère et exige la libération de leurs camarades détenus par la police, notre inquiétude est grande pour tous ceux et toutes celles qui manifestent et se soulève aujourd'hui en Iran, l'ONG Iran Human rights fait état d'un bilan particulièrement lourd, plus de 90 morts tandis que le ministère des Renseignements iranien revendique l'arrestation de 9 ressortissants de pays européens dont la France, pour leur rôle dans les manifestations. l'avocate pardon iranienne et prix Nobel de la paix Shirin Ebadi a récemment soutenu qu'il revient aux pays occidentaux de réduire leurs contacts avec l'Iran parce qu'un pouvoir qui est sourd aux demandes de son peuple, doit être boycotté, d'un point de vue politique, c'est aussi le sens de notre demande aujourd'hui dans une dans une totale unanimité des différents groupes du Sénat. La parole est à Madame Valérie Boyer. Pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis 2 semaines après la mort de la jeune Masha Amini en Iran, des femmes courageuses, avec l'appui de certains hommes poursuivent leur évolution au péril de leur vie, mais alors que nous, à juste titre le courage c'est iranienne, je profite de ce temps de parole pour vous dire à quel point je regrette que nous ne parlions pas davantage des femmes arméniennes actuellement torturés, démembrés violée, tuée et filmés par les Azéris fiers de leur forfait, je pense en particulier à Anoucha pétillant et à toutes les autres cette barbarie se fait dans l'indifférence générale et il ne peut y avoir de hiérarchie de l'horreur le sang des Arméniens cool comme celui des Ukrainiens ou des Iraniens ne les abandonnons pas pour autant alors que la France Emmanuel Macron veut servir d'exemple en matière de respect de droits des femmes, qu'en est-il, nous avons l'Union européenne et le Conseil de l'Europe qui enchaîne des campagnes de communication pro-voile sans protestation de notre gouvernement, que ce soit avec le slogan la liberté dans le hidjab ou avec des affiches de petites filles voilées, doit-on y voir la marque de la Turquie d'Erdogan, toujours membre du Conseil de l'Europe ou d'organisations islamistes comme les Frères musulmans qui tentent depuis des années, d'imposer des programmes de recherche d'agir sur nos institutions, comment accepter ce détournement de fonds publics, des institutions démocratiques utilisé pour normaliser, non pas une liberté religieuse mais un enfermement dans le sexe, une négation de la personne un interdit de liberté à l'interdit d'égalité un interdit de fraternité, l'Europe, si prompte à remettre en question les valeurs ne peut être le cheval de Troie de l'Islam politique, pourtant vous pratiquez toujours la politique du Mans, en même temps, vous nous dites agir mais aucune sanction n'a jamais été envisagée contre l'Union européenne ou le Conseil de l'Europe, ni à l'encontre d'associations qui font en France, la promotion du voile ou même d'organismes publics qui pose avec des femmes voilées, aucune enquête pour savoir d'où viennent ces promotions indigne, pire encore, depuis que les Iraniens ne se révolte, nous entendons de nouveau dans notre pays, cette petite musique, liberté de ne pas porter le voile, liberté de pouvoir le porter à l'heure où les femmes iraniennes bravent l'interdit certains dans notre pays devrait méditer l'exemple de ces militants de la liberté, comme si le voile ne sera en France qu'un vêtement ou un embellissement ou une liberté 6 Masha Amini a été tué ce n'est pas pour un simple bout de tissu accepté cette fois s'en mode c'est conforter le communautarisme dans notre pays, c'est choisir le camp des oppresseurs, c'est soit lire le camp des islamistes, c'est abandonner les femmes d'Iran, d'Afghanistan, d'Arabie qui sont obligées de se voiler, mais aussi celle d'Algérie, de Tunisie au d'ailleurs qui le font au nom de la présence sociale comme celle de nos quartiers ne nous leurrons pas : la bataille du voile est l'expression la plus visible de la volonté des intégristes de marquer leur territoire et de soumettre les femmes comme les hommes, cette forme de purification vestimentaire en est le marqueur aujourd'hui nous voyons dans dans notre pays non pas des zones de non-droit, mais des zones d'un autre droit ou l'islamisme s'affiche en uniforme et organise à véritables contrôle social d'ailleurs pendant que les Iraniennes héroïques arrachent leur voile pour sentir le vent dans leurs cheveux, des adolescentes rebelles détenus islamistes dans nos écoles, mais le ministre de l'Éducation nationale préfère déplorer à l'étranger, l'absence de débat nuancé sur les questions ethno-raciale et découvrent ce que nous dénonçons depuis des années, l'école n'est malheureusement plus le sanctuaire de notre République, mais devient le théâtre de revendications communautaires, pire encore, de menace islamiste, comment ne pas penser à Samuel Paty l'école construit l'Islam détruit d'islamisme détruit pour reprendre Vincent Trémolet de Villiers hier c'était là qu'on faisait des Français aujourd'hui, c'est à l'école, que la France se défait votre faiblesse et votre inaction inquiète les Français, mener la bataille contre le voile islamique, c'est mener la bataille pour l'humanité, pour la liberté car en enlevant aux femmes leur identité, leur visage, on leur enlève leur humanité et pourtant vous vous êtes toujours opposée aux propositions que nous avons formulé, je pense notamment aux propositions, nous avons fait dans la loi séparatisme et vous nous avez même accusé de déposer des amendements, textile, quel mépris, je pense à l'interdiction du voile des accompagnatrices scolaires pour les mineurs, ou encore le burkini il est de notre responsabilité de dire haut et fort que nous ne pouvons accepter qu'en France comme ailleurs qu'une petite fille porte ce signe d'infériorisés Sion, parce que c'est de ça dont il s'agit, nous le devons aux Français, nous le devons à nos jeunes filles, nous le devons à celles et ceux qui prennent le risque de leur vie pour leur liberté, nous ne devons aussi à celles et ceux qui se réfugier en France pour cette liberté, nous le devons à toutes ces femmes à travers le monde qui risquent leur vie avec courage pour refuser de porter le voile femme vie liberté un beau slogan en France comme ailleurs car, pour reprendre ce que disait Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté ni de liberté, son courage alors aujourd'hui ayant du courage et de la cohérence, c'est-à-dire refusons bien évidemment et soutenons les femmes, les femmes iraniennes mais refusons aussi ses marques d'infériorisés sont dans notre pays. Voilà 43 ans que les Iraniennes et les Iraniens qui avaient fait tomber la dictature du Shah vivent sous une autre dictature 43 ans que les mollahs ont confisqué des révoltes populaires et les aspirations démocratiques de 78 et 79. 43 ans que nous accueillons nos amies féministes démocrates syndicalistes kurde homosexuels 43 ans que nous lisons leur livres que nous voyons leurs films et que nous faisons ce que nous pouvons pour qu'on ne s'habitue pas à la répression au pendaison au déguisé aux décapitations et aux persécutions 43 ans, que la République islamique d'Iran impose à son pays et au monde, scène des femmes et ça haine des juifs, alors aujourd'hui nous pleurons d'émotion. Nous tremblons de peur, chaque matin, nous regardons les vidéos que au péril de leur vie des Iraniennes et des Iraniens ont capté pendant les manifestations dans les universités, dans les collèges, dans les rues. C'est une révolution féministe. Qui a émergé aujourd'hui en Iran une révolution féministe qui entraîne une insurrection générationnel et qui mobilise le soutien d'une grande partie de la population. Les femmes qui sont l'obsession des islamistes. Sont aussi leur première menace parce que leur combat est universelle, parce que ce sont elles qui sont le ferment de la rébellion, parce que, en fait, les Iraniens ne s'y trompe pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout, les Iraniens ne s'y trompe pas, personne n'est libre dans un pays où les femmes ne le sont pas. Alors, beaucoup de nos collègues avant moi ont eu des mots très beau, très fort pour dire leur leur solidarité avec le peuple iranien pour dire leur crainte du lendemain ces jeunes, de voir ces jeunes gens que l'on connaît par j'évoquais tout à l'heure, les vidéos et un jour, on les voit et le lendemain, on apprend qu'ils ont disparu, que leurs corps a été rendus à leur famille, tout le monde tremble du moment où la répression sauvage peut s'abattre sur eux. Mais je voudrais en toute courtoisie dire à certains de nos collègues et je peux me permettre de dire parce que personne ne m'a jamais prise en défaut lorsqu'il s'agit de caractériser le voile islamique la le hidjab tous ces oripeaux pour ce qu'ils sont des outils politiques. D'un projet religieux et politiques qui tous portent. La l'oppression et la domination des femmes en ne que nous ne devons pas poursuivre nos discussions franco-française, voire même franco-européenne aujourd'hui en saisissant le prétexte de la révolte en Iran, nous aurons l'occasion d'en débattre encore, ne vous inquiétez pas. Pierre Laurent, d'autres ont cité les femmes d'Afghanistan les femmes d'Arménie, cité par Valérie Boyer tout à l'heure, en fait, les femmes à peu près partout dans cette planète à peu près partout pour dire aussi que les fous de Dieu, ne sont pas tous islamistes, il y a aussi des fous de Dieu dans bien d'autres pays qui ne sont pas des pays islamistes les fous de Dieu sont à la Cour suprême aux États-Unis à priver les femmes de leur droit d'avorter les fous de Dieu sont dans les Favel à Rio à drainer les voix des classes populaires en faveur d'un dictateur d'un fasciste, pardon, je me tromper, ce n'est pas un dictateur d'un fasciste Bolsonaro qui menace non seulement son peuple et la planète alors combattre des fous de Dieu, c'est notre responsabilité partout sans choisir les dieux.

Merci monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues Malala Yousafzai il avait 15 ans lorsque les talibans lui ont tiré une balle dans la tête alors qu'elle se rendait à l'école, Amina Ali avait 17 ans lorsque des mercenaires de Boko Haram l'ont enlevé avec 219 autres jeunes filles alors qu'elle était au lycée Marzin un mini arrêté par la police des moeurs avait 22 ans lorsqu'elle est morte dans les geôles iraniennes alors qu'elle avait laissé s'échapper quelques mèches de cheveux de son voile toutes avaient en commun de vouloir vivre libres dans des états ou le pouvoir religieux, militaire ou politiques le leur interdisait parce qu'elles étaient des femmes, la mort de Mahsa Amini nous bouleverse, comme elle a bouleversé son pire elle a suscité une vague de courage admirable chez des femmes et des hommes que tout menace à ce jour plus de 60 personnes ont donné leur vie après que Marsa et perdu la sienne et ils sont des milliers à la risquer dans les rues d'Iran au nom de la plus haute idée qu'ils se font de la dignité humaine dans notre pays où les allégorie de la Liberté prennent si souvent les traits de femmes le cri des Iraniennes résonne avec un écho particulier en Occident, nous savons combien le chemin vers cette liberté ardue lent et exigeant jamais garanti, bien qu'il habite notre philosophie depuis des siècles, nous savons également ce que la lutte pour les droits des femmes suppose de cette même exigence Silvio tonneau et cette promesse faite au monde cette assurance qu'il se battra toujours pour que chacun, quel qu'il soit puisse vivre sans crainte pour son existence et que jamais une femme ne meurent du simple fait d'être femme alors l'Occident se doit profondément d'être cohérent face à un état qui a fait de l'oppression des femmes un marqueur de sa politique, il en va de ce que nous sommes l'histoire récente de l'Iran nous montre que rien n'est acquis, il nous incombe d'oeuvrer pour que de telles menaces ne prennent jamais racine sur notre territoire la radicalité qu'elle soit religieuse ou politique n'a sa place ni des dans les principes qui nous fonde ni dans les traités qui nous régissent ni dans les lois que nous élaborons, nous devons aux femmes iraniennes de ne pas laisser se répandre chez nous, ce qu'elles veulent tant voir disparaître chez elle, Madame la Ministre, le radicalisme politique et religieux qui s'attaque aux droits de l'homme en Iran s'embarrasse peu des frontières. nous savons bien qu'il pèse aussi à moindre degré en Europe et dans notre pays on ne peut indéfiniment chérir les causes dont on déplore les conséquences le temps mis pour expulser Hassan Iquioussen l'augmentation du nombre de signalements d'atteintes à la laïcité à l'école que le ministre-pape Ndyaye confirmé la semaine dernière, ou encore la campagne de communication du Conseil de l'Europe, la liberté dans le hidjab ne sont que que quelques exemples d'un entrisme inquiétant opérée, parfois avec le concours passif de l'État, Madame la Ministre, cet événement tragique, interroge notre cohérence la condamnation unanime que nous portons contre cet acte ne suffit pas, il revient à votre gouvernement de défendre les principes qui nous fondent et qui nous porte vous engagez-vous à propager les voix, la voix des Iraniennes les valeurs de liberté et d'égalité dans les instances nationales, européennes et internationales en luttant notamment pour que les principes radicaux qui régissent aujourd'hui des systèmes étatiques oppressives comme l'Iran, tendent à disparaître, vous engagez-vous partout où notre pays s'investit à oeuvrer pour qu'aucune forme de soutien, ni économique, ni morale, ni politique ne soit offert aux partisans de telles idéologies vous engagez-vous à envoyer un signal clair à Malala Yousafzaï à Amina Ali à Marsa à mini celui que jamais nous ne tendrons la main de quelque façon que ce soit à ce qu'il a voulu les détruire le courage des Iraniens et des Iraniennes appelle aujourd'hui le nôtre, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Catherine Colonna Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les les sénateurs merci de ce débat merci de vos interventions très largement convergentes entre les convergentes aussi avec nos propres lignes même si chacun s'exprimera à sa façon. Vous l'avez tous dit le 16 septembre dernier Mahsa Amini est morte à 22 ans sous les coups de la police des moeurs de la République islamique d'Iran, il avait arrêté au prétexte qu'elle aurait mal porté son voile Une vie détruite et pourquoi, pour une mèche de cheveux dépassant d'un voile, quelques jours plus tard, une autre jeune fille puis tant d'autres étaient victimes de la même violence lorsque la répression du régime s'abattit brutalement sur les manifestantes et les manifestants partout en Iran de sa caisse, la ville natale de Mahsa Amini à la ville sainte de Qom de Machhad à Téhéran de Chiraz à Ispahan ou à Karaj. Tant de vies détruites parce que ces jeunes femmes oser revendiquer leur liberté parce qu'elles osaient affirmer que leur dignité ne valait pas moins, mais autant que celle d'un homme, c'est aujourd'hui un même cri qui retentit femme vie liberté c'est ce cri que le régime cherche à étouffer par la censure et par la violence, à ce jour, les ONG ont fait état de plus de 100 victimes, sans doute, le chiffre est-il supérieur et de plus de 1000 arrestations de militantes et de militants d'avocats et d'avocate de journalistes de citoyens, de femmes et d'hommes unis par la même volonté d'émancipation. Femme vie liberté c'est ce cri aussi que la diaspora iranienne Anton en déco de Paris à San Francisco, de Londres à Rome ou à Erbil. Dès le 19 septembre la France a condamné avec la plus grande fermeté les violences ayant entraîné la mort de machin et mini et la violence utilisée contre les manifestants, comme je l'ai rappelé hier à l'Assemblée nationale, nous avons appelé les autorités iraniennes à respecter le droit de manifester pacifiquement, respecter le droit au rassemblement et aussi à respecter l'exercice de leur métier par les journalistes, nous l'avons fait officiellement et j'ai fait moi-même auprès de la presse aussitôt en marge de l'assemblée générale des Nations unies, ou ici en France, à plusieurs reprises. Les autorités iraniennes ont considéré qu'il s'agissait d'une forme d'ingérence que de rappeler les principes fondamentaux des droits de l'homme, elles ont cru bon de le faire savoir notre ambassade sur place, j'ai donc décidé de faire convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris car il n'y a pas en ce moment d'ambassadeur d'Iran, il a été reçu vendredi dernier au Quai d'Orsay, il lui a été dit clairement ce que nous pensons des méthodes iranienne. Mesdames et messieurs les sénateurs, ce qui se joue dans les rues de Téhéran et dans les autres villes iraniennes, c'est la liberté, il y a d'un côté, la répression, une répression brutale que nous condamnons dans les termes les plus forts, une répression menée contre des femmes et des hommes qui manifestent pour le respect de leurs droits et de leur dignité, une répression que nous avons dénoncé à plusieurs reprises et que tu nous continuerons à dénoncer, je peux vous rassurer, Monsieur le Sénateur, évidemment, sur ce point, nous le faisons au conseil de droits de l'homme à Genève, nous le faisons dans toutes les enceintes internationales et nous le faisons dans chacun de nos échanges bilatéraux, quel qu'en soit le niveau. Rappelons aussi que l'Iran a lui-même souscrit aux principes fondamentaux que nous défendons ici le principe du Pacte relatif aux droits civils et politiques des Nations-Unies, auquel elle a adhéré en 1975 et je précise, en réponse à Madame la sénatrice Billon, que l'Iran a en effet été élu à la commission des Nations unies sur la condition de la femme, c'est la règle majoritaire au sein de chaque groupe géographique auquel nous n'appartenant pas au demeurant cet organe est utile car il produit des documents de référence sur la situation des droits des femmes dans les pays et permet donc de mieux savoir ce qui se passe chez eux. En face, les autorités il y a une aspiration à la liberté et je dis en face, face aux auteurs de la répression mais je devrais dire partout car cette aspiration à la liberté, nous la voyons partout s'exprimer les femmes d'Iran veulent vivre libres et un grand nombre d'Iraniens les suivent désormais des villages kurdes d'Iran aux métropoles du Baloutchistan de la Caspienne au golf les femmes d'Iran veulent vivre libres, les femmes diront veulent que leurs droits soient garantis les femmes d'Iran Aspire à ce que leur égale dignité soit respectée, le courage des femmes iraniennes force l'admiration et nous oblige, nous soutenons leurs aspirations et nous continuerons à les soutenir, mesdames et messieurs les sénateurs. Nous sommes en première ligne pour agir avec nos partenaires européens, notre réponse doit être à la hauteur de l'enjeu et en ce sens, nous avons lancé dès la semaine dernière avec nos partenaires européens des travaux afin de sanctionner les auteurs de la répression, il s'agira de geler les avoirs et de geler, d'interdire donc le droit de voyager aux individus identifiés comme responsables des violences, il nous espérons madame la sénatrice Carlotti, que ce soit fait d'ici 8 à 10 jours, nous sommes 27, dois-je vous le rappeler, madame la sénatrice Vogel permettez-moi aussi de préciser que les négociations sur le retour au Pitiot et se sont conclus par la présentation d'un texte que l'Iran n'a pas pour l'heure, accepté en d'autres termes, elle ne se déroule donc pas, quoique la conclusion d'un accord aurait un fort intérêt pour empêcher l'Iran d'accéder au seuil nucléaire, ce qui sera vraie de de loin préférable, chacun en conviendra. Nous resterons totalement mobilisé aux côtés des Iraniens, des des Iraniens qui se battent pour leur droit à la dignité, car vous le savez, hélas, les violations des droits de l'homme en Iran n'ont pas attendu les événements récents nous continuerons d'appeler l'Iran à mettre fin aux discriminations et à toutes les formes de violence envers les femmes et les filles à interdire les mariages précoces et à permettre l'accès des Iraniennes à leurs droits en matière de celle de santé sexuelle et reproductive quand il s'agit pas que de l'obligation de porter le voile l'oppression que subissent les femmes iraniennes et brutal, inscrite dans les lois de la République islamique autant que profondément enracinée dans les moeurs du régime. Aucune société, nous le savons, ne peut se développer sereinement, si elle n'assure pas l'égalité des droits, l'égalité entre femmes et hommes, l'égalité entre femmes et hommes qui est une condition du développement qui est même le gage d'une société libre, un élément fondamental de la justice indispensables à nos vies. Ce combat essentiel n'est donc pas notre seul combat parce qu'une société injuste avec les femmes, et tout simplement une société injuste pour tous, nous continuerons à dénoncer des arrestations arbitraires, des cinéastes, des militants des droits de l'homme, des femmes et des hommes engagés pour la défense de la liberté d'expression, d'étudiants, de journalistes, nous continuerons, dénoncé les exécutions auxquelles il est procédé, y compris les exécutions de mineurs, et nous le faisons, et nous le ferons, parce que c'est notre responsabilité, nous le faisons, et nous le ferons, parce que nous avons le droit moral et politique de défendre les valeurs qui sont les nôtres oui mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous disons tous ensemble, la femme est l'égale de l'homme en Iran comme ailleurs, je vous remercie. Je vais suspendre la séance pour quelques instants afin de afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point à l'ordre du jour et la stratégie maritime national. La séance est suspendue.

La séance est donc reprise l'ordre du jour appelle le débat sur la place des outre-mer de la stratégie maritime nationale débat demandé par notre délégation aux outre-mer la parole et tout d'abord aux orateurs de la délégation qui a demandé ce débat et qui ont se sont partagés le temps de parole nous commençons par madame Annick Petrus, au nom de la délégation aux outre-mer.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2017, la France s'est dotée d'une stratégie nationale pour la mer et le littoral. Conçu pour une durée de 6 ans qui a été acté par décret les outre-mer en 97 % de l'espace maritime français, la délégation aux outre-mer du Sénat a souhaité évaluer cette politique publique qui se situe à la croisée de tous les grands enjeux actuels les enjeux géopolitiques et sécuritaires, bien sûr, mais aussi les enjeux de valorisation économique, énergétique et scientifique les enjeux de communication avec la question des transports maritimes et du câble a et sous- marins, sans oublier les enjeux climatiques et environnementaux avec mes autres collègues rapporteurs Philippe Folliot et Marie-Laure Phinéra Horth nous faisons globalement le constat paradoxal et préoccupant, suivant l'autre stratégie nationale pourtant indissociable des outre-mer ne les associe pas à la hauteur de nos atouts et de leur potentiel, c'est pourquoi nous estimons que pour la prochaine stratégie en cours de préparation, la méthode et les orientations devront être radicalement revue si nous voulons construire la puissance maritime à laquelle la France peut légitimement prétendre pour cela nous formulant dans notre rapport 20 propositions articulées autour de 3 axes majeurs : premièrement remplace replacer les Outre-mais au coeur de notre stratégie maritime nationale, selon nous, les orientations de cette stratégie doivent absolument être rehaussé et faire l'objet d'un grand débat devant le Parlement, précédé naturellement par une concertation dans les territoires concernés deuxièmement consolider notre souveraineté maritime pour crédibiliser les ambitions françaises avec des moyens adaptés, notamment au plan militaire et technologie, faire de la stratégie maritime, le moteur de la transition économique des outre-mer afin d'être un levier de développement pour nos territoires encore insuffisamment tournée vers la mer, c'est du dernier volet vont être développés à présent par mes deux collègues à qui je cède la parole. Merci, cher collègue est, en effet, la parole est à monsieur Philippe Folliot, pour les trois minutes suivantes. Monsieur le président, monsieur le président de la délégation, monsieur le préfet, pardon, Monsieur le Ministre, mais dis mes chers collègues. Sur ces enjeux de souveraineté relative donc à la stratégie maritime nationale et à sa déclinaison dans les outre-mer si vous me le permettez, monsieur le Ministre, et si finalement on avait mis un point d'interrogation à la fin de la présentation donc de notre rapport, je voudrais simplement répondu par mot congrue. Parce que nous sommes face à une situation qui est une situation au niveau de laquelle les outre-mer ne sont pas à la hauteur des enjeux qui devraient être les leurs au regard du fait que 97 % de notre zone économique exclusive, ça été rappelé et je tiens à saluer du resto mes 2 collègues qu'au rapport trices de ce rapport pour dire que nous avons un certain nombre d'enjeux de difficultés en matière de souveraineté tout d'abord, dans ce cadre, nous avons en mémoire les échanges que nous avons eue avec notamment des cols des marins-pêcheurs de Guyane, qui nous ont fait part de la façon dont ils étaient agressés dans leur quotidien, nous avons pu constater aussi un certain nombre de difficultés qui sont tout à fait réel et prégnante au regard de l'exercice de la souveraineté, vous savez Monsieur le Ministre, mieux que quiconque, nous sommes face un trou capacitaire par rapport aux moyens qui sont les nôtres, de contrôler et de surveiller notre zone économique exclusive, tout un chacun sait aussi les difficultés qui peuvent être les autres sur certaines parties totalement oublié, je pense à la passion qui Bertone qui sont complètement laissées à l'abandon de de ces enjeux et de toutes ces difficultés par rapport à à ces questions, nous devons simplement nous poser une question Monsieur le Ministre est-ce que pour notre pays, c'est quelque chose d'important ou pas l'absence de réponse depuis de nombreuses années au regard des moyens affectés par rapport à cela, prenons que l'exemple des forces de souveraineté, celles-ci sont passées d'un peu plus de 8000 effectif en 2008 à à peine 7000 aujourd'hui. Face aux enjeux qui sont les enjeux géopolitiques du moment face à des éléments de stratégie dont on parle à tout bout de Champ Endo pacifique indopacifique ce sont des mots aujourd'hui et derrière ces mots, il est urgent que notre pays décline une stratégie avec des actes et ces actes ne pourront être portées qu'au travers de cet appui que peut représenter, et cet atout exceptionnel que peut représenter nous outre-mer par rapport à cela il y a un un élément et c'est un petit peu le sens de ce que nous avons souhaité avec mes collègues, par rapport par rapport à cela, c'est un peu aussi le fond, j'allais dire du travail de notre délégation aux outre-mer, c'est qu'il y ait une réelle prise de conscience de ces enjeux et qu'il y a une réelle volonté d'y répondre jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas espérons que demain il en soit différemment, je vous remercie. à qui je donne la parole. Pour les trois minutes finales. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis ravi de prendre la parole, ici devant vous, afin d'évoquer la situation de nos territoires ultramarins ce rapport, tout comme les autres, publiées par la délégation sénatoriale met en lumière des problématiques qui sont souvent propre aux outre-mer et parfois malheureusement méconnu sur le plan national, j'en veux pour preuve la situation des porcs dans nos régions grâce à leur position stratégique ses infrastructures pourraient devenir des pôles importants pour le transport mondial, pourtant, à l'exception de Port réunion qui figure parmi les 4 meilleurs ports français, les autres mérite homme sérieux effort de modernisation, au travers de la réforme portuaire de 2012 marquée par la création des grands ports maritimes, le législateur a grandement améliorer le fonctionnement des ports toutefois ses poumons économiques sont en manque de moyens permettant de s'adapter à l'explosion du trafic par porte-containers en Guyane par exemple les navires sont déchargés essentiellement avec les grues de bord faute de portique ou de grue sur les quais, la lenteur de ces opérations, impacte le coût du fret et par conséquent grèvent le budget des ménages guyanais, nous devons garder à l'esprit que ces ports permettent de sécuriser l'approvisionnement des biens de consommation et des matériaux de construction pour des populations qui sont extrêmement dépendante de l'extérieur très riche et instructif, le rapport de la délégation préconise de nombreuses pistes comme un port flottant extérieur pour le plateau des Guyanes voir l'évolution du statut du port Longoni de Mayotte, lorsqu'un certain nombre de freins auront été levé, chers collègues, nous avons le devoir de rester vigilant car ces ports demeure la principale et parfois l'unique porte d'entrée de nos territoires, j'entends profiter de cette tribune pour évoquer un autre dossier sensible : la pêche, les professionnels guyanais ont profité de ces auditions pour exposer une situation catastrophique, ils doivent faire face à une baisse importante de la production en raison d'une pêche qui est illégale, non déclarée et non réglementée cette activité intensif et généralement le fruit de navires étrangers venus du Brésil ou du Surinam, nonobstant les efforts de la marine nationale les moyens doivent être réajustés pour accroître la pression sur les navires étrangers actuellement, l'État ne consacrent que 120 jours à cette lutte dans les eaux guyanaises contre une présence de 300 jours dans le canal du Mozambique, une différence de traitement qui interpelle les professionnels car ils doivent faire face à des pêcheurs étrangers de plus en plus violents même les actions, maire de la marine nationale sont comparés à des opérations de guerre, chers collègues, j'en parle ici avec émotion, car la filière a perdu il y a quelques mois à son chef de file, Georges Michel Karam, qui s'étaient battus pour la préservation de la pêche en Guyane et cette filière assurance encore l'approvisionnement de la population, produits de la mer, mais pour combien de temps encore, je vous remercie de m'avoir écouté.

Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens d'abord à saluer le travail conséquent des rapporteurs sur ce rapport et vous remercier de m'avoir invité à la question, j'ai entendu les outre-sont-ils à la hauteur des enjeux, je dirais que c'est la prise en compte des Outre-Mer partout tout le temps par l'ensemble des décideurs publics français qu'il nous faut améliorer, pas simplement sur la mer, je crois qu'il y a un enjeu là qui est fort et tout. il faut dire et redire que la France dispose du 2ème, espace maritime mondial qu'elle le doit à ses outre-mer, et plus encore la France est le seul pays au monde à être présents sur les quatre océan cette profondeur stratégique unique, confie un rôle central à la France dans le concert international, quelle que soit la taille et la puissance de notre pays le premier enjeu de la place des outre-mer dans la stratégie maritime c'est effectivement, vous l'avez dit, celui de la souveraineté. Les vastes espaces maritimes et littoraux de la France Outre-Mer sont aussi des joyaux de la biodiversité marine littoral qui s'étend du pôle Nord au pôle sud de la forêt boréale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux colonies de manchots empereurs des Terres australes en passant par le merveilleux lagon de Mayotte ces joyaux et je les connais tous sont convoités, ils font face en plus au défi du changement climatique leur préservation doit constituer une priorité absolue. Par ailleurs, les vous l'avez dit madame sont très dépendants de la mer pour assurer le développement économique et la vie quotidienne des populations. La création de valeur qui mon leitmotiv désormais en toute occasion passe nécessairement par le développement d'une économie bleue durable et résilience et par des ports en bonne santé. La souveraineté, première des priorités. Votre rapport met au 1er plan cet enjeu de la souveraineté et c'est une priorité que je partage. Si la France n'est pas capable d'assurer la pleine souveraineté dans ces espaces maritimes alors il est inutile de parler d'environnement, et encore moins de développement économique, assurer la souveraineté de nos espaces maritimes, c'est d'abord être en capacité de les surveiller par la terre par la mer et dans les airs. Comment. La France assure une présence militaire permanente dans la quasi-totalité des territoires, y compris inhabité et le canal de Mozambique il y a des enjeux de souveraineté qui qui ne font pas le cas en Guyane souveraineté sur la mer, mais dans le canal de Mozambique : les enjeux de souveraineté sont importants, d'où une présence plus forte dans le canal de Mozambique que large de la Guyane. La marine déploie depuis 2017 2 nouveaux navires. Adapter mieux adaptée aux besoins des mer c'est un renouvellement sans précédent 13 nouveaux bâtiments dédiés uniquement aux outre-mer auront été livrés au 1er janvier 2026 les moyens aériens, eux aussi, sont en cours de renouvellement mais ces moyens traditionnels doivent être complétées par des moyens alternatifs comme les drônes et le ministère des Armées, il travaille le vase zone économique exclusive, donne à la France des droits exclusifs d'exploration, d'exploitation, de préservation et de gestion des ressources, il faut les protéger contre les appétits de tout un chacun à l'extérieur mais aussi mieux les connaître. C'est le sujet du monde, deuxième partie connaissance et préservation. De la biodiversité ultramarine, on cite souvent les 97 % d'espace maritime ultramarins on parle moins des 80 %, c'est-à-dire la part des Outre-mer dans le total de la biodiversité française 80 %. Les outre-mer sont peu citer en exemple. Et s'il est un domaine où ce devrait être le cas, c'est bien celui de la protection de la biodiversité, la France prend des initiatives fortes, vous le savez, pour la protection des coraux et des mangroves, grâce à la réserve nationale naturelle nationale des Terres australes, par exemple, la France a déjà atteint l'objectif de classer 30 de ces espaces maritimes et terrestres en aires protégées, c'est un apport considérable des Outre-mer à la stratégie française. Préserver la biodiversité c'est aussi mieux la connaître les îles Eparses constituent le magnifique espace d'observation de changement climatique, enjeu de débats internationaux, je signerai bientôt avec le ministre et la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, une feuille de route qui permettra de pérenniser les efforts de recherche dans ces îles les importants moyens développés déployée par la France depuis par France 2030 pour mieux connaître les grands fonds marins ont clairement vocation à être mises en Oeuvres dans les outre-mer je pense ici au Pacifique, mais aussi à la surveillance du volcan sous-marin de Mayotte, cette connaissance et cette protection des milieux marins sont au coeur des perspectives de développement de l'économie bleue en effet l'économie bleue. Présente déjà une part non négligeable de l'économie des Outre-Mer dans les Drom elle représentant ainsi entre 5 et 10 % du PIB, c'est que économie bleue comme on dit, est principalement centrée autour du triptyque port et beaucoup reste à faire, je pense que là, une question sur laquelle je pourrais revenir sur le sujet, pêche, tourisme, qui doit s'adapter aux enjeux du XXIe siècle, c'est-à-dire changement climatique souveraineté économique, énergétique et alimentaire. Sur les ports d'abord leur fonction centrale dans l'approvisionnement des territoires doit consolider, il doit aussi accélérer leur transition énergie écologique et on développera les bateaux de croisière que ceux uniquement si tous les ports sont électrifiés, sinon il y aura des réactions qui font que ça ne marchera pas. J'ai la conviction que les grands ports maritimes ultramarins peuvent constituer des accélérateurs de la transition énergétique outre-mer par exemple en matière d'emploi de carburants alternatifs, il veut enfin s'adapter aux évolutions des normes de transport je pense d'annonces récentes de la CMA CGM sur la desserte des Antilles, mais nous y reviendrons, le secteur de la pêche et par ailleurs au coeur d'autonomie des enjeux de l'autonomie alimentaire dans les outre-mer il est absolument ahurissant que plus de 80 pour 100 du poisson consommé aux Antilles furent importées. Les pêcheurs ultramarins doivent pouvoir pêcher mieux c'est tout l'enjeu de notre combat pour le renouvellement des flottes, mais une question, et là-dessus, et j'y reviendrai d'économie bleu outre-mer, ce sont aussi des secteurs en devenir, je pense ici à l'industrie navale, je pense aux énergies marines renouvelables ou les mer ça faire preuve d'excellence comme en Polynésie et bientôt en Guyane. En conclusion, il est difficile et peut-être je parlais trop vite de résumer en quelques minutes 97 % de la puissance maritime française, je vous remercie de le faire valoir à travers cette audition à travers ce rapport, c'est fondamental, et si on en parle pas assez, c'est notre faute à tous, je dis bien à tous. La création de valeur dans les outre-mer. Mon leitmotiv, la définition d'une feuille de route économique pour chaque territoire. C'est la mission que le président de la République m'a confié. Je m'y attelle ces feuilles de route auront nécessairement une forte nuance bleu dans la mer est liée aux outre-mer et les outre-mer à la mer. L'État accompagnera les territoires dans le développement d'économie bleue durable résilience pour que c'est votre souhait, c'est le mien. Les outre-mer français soient réellement au coeur de la stratégie maritime de la France merci et je me prépare à répondre à vos côtés. Merci monsieur le ministre, et ça me donne le moment de rappeler la règle du jeu dans la suite du débat chaque orateur dispose de deux minutes maximum, y compris son éventuelle réplique le gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente, le gouvernement à la faculté, s'il le juge nécessaire de répondre à une réplique pendant une minute, l'auteur de la question disposera à son tour du droit de répondre à nouveau pendant une minute, nous commençons avec le président Artano

tous les acteurs unanimement l'absence de cohérence et parfois de coordination dont la prise de décision des infrastructures vieillissantes qui nécessitent d'être rénovés ou mais de bénéficier d'opérations de maintenance importante, les besoins sont structurels et les atouts demeurent inexploités pourtant le maintien des liaisons maritimes est vital pour l'archipel, ne serait-ce que pour le simple ravitaillement de la population, l'absence de stratégie de l'État en matière d'économie bleue est particulièrement frappante pour l'archipel et le condamne au repli la stratégie nationale adoptée en 2017, prévoyez l'élaboration d'un document stratégique par bassin, il n'a jamais vu le jour, malgré l'élaboration d'un diagnostic sur mon territoire, la création ce qu'on l'envisage la création d'un établissement public portuaire voulue par l'ancienne ministre de la mer n'est pas la réponse aux difficultés, le simple respect des institutions comme le Conseil portuaire serait déjà un minimum le rapport de la préfigure attriste émet des hypothèses de recettes plutôt inquiétante et que je ne cautionnerait jamais comme le des anneaux de plaisance possiblement exorbitants ou encore une possible taxe sur les passagers transportés par des ferries localement, tout reposant sur un équilibre financier qu'on ferait peser sur trop peu d'usagers avant même de parler de gouvernance, Monsieur le Ministre portuaire, il convient que l'État donne sa vision de la place qu'ils souhaitent en matière maritime pour notre archipel Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer, d'une part Saint-Pierre et Miquelon fera partie de cette stratégie nationale et d'autre part qu'il ne disposera d'un volet de remise à niveau ambitieux de ses infrastructures fortement dégradé. Monsieur le Ministre.

2017 entre 17 et 22 30 millions ont été investis par l'État 6 millions pour la rénovation des digues 15 millions pour la construction d'de croisière 3 millions pour engager la rénovation des Kids Miquelon et des kits de commerce à Saint-Pierre les discussions sur les autres investissements seront, nous en avons parlé étudié dans le cadre du prochain contrat de plan que nous allons bâtir ensemble. Faut-il un grand port maritime : faut-il une concession géré par l'État directement, c'est tout le sujet du déplacement que fera Saint-Pierre et nous déciderons ensemble, il ne faut pas avoir de vertu absolue sur ceci ou cela, il faut prendre le plus efficace et le plus efficace c'est quand nous mettrons d'accord ensemble dans le cadre du contrat de plan, sur ce qu'il faut faire, il y a pas de il quant à desserte maritime, c'est un vrai sujet à Saint-Pierre et à Miquelon desserte interne dessertes vers l'extérieur des certains passagers des certes en marchandises le droit en la matière est clair : le Conseil d'État l'a encore rappelé dans son avis de juin dernier à l'État, le transport des marchandises à la collectivité territoriale de transport des passagers dans le cadre des suites de la réunion du 7 septembre autour du président de la République, peut-être faudra-t-il faire évoluer cela je n'en sais rien, je découvre pas mais je commence à étudier, pour autant, le préfet engagé à ma demande, vous le savez, celle du secrétaire d'État à la mer, un travail conjoint avec vous, avec la collectivité territoriale en vue d'expérimenter sur une courte durée des possibilités plus large pour de Fred par les ferries de la collectivité de l'archipel terne, il faut effectivement, et vous le savez, travailler avec nos voisins et amis, pas toujours mais souvent et amis canadiens pour régler cette affaire, ça sera l'objet principal de mon déplacement à Miquelon, soit en toute fin d'année sont en tout début d'année. Merci pour votre précision ferroviaire, monsieur le ministre et le président Artano a encore un capital de 23 secondes, il ne faut pas gaspiller. Merci monsieur le président, oui, l'État investit 15 millions dans un port de croisière, un port de croisière qui n'a été voulue par aucun acteur local, c'est une décision du 1er ministre Manuel Valls à l'époque, ce sont des décisions qui outrepasse et qui ne tiennent pas compte des instances déjà existantes que sont le conseil portuaire, donc si vous voulez effectivement l'État investit mais ces 15 millions ils auraient pu être mis pour préserver le quai de commerce numéro 1 quai de commerce numéro 2 ou préserver les digues, ça n'a pas été le cas et je dis que plutôt que de se poser la question sur un grand port à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, posons-nous les vraies questions d'investissements structurants et qui sécurise les approvisionnements. Merci, cher collègue, et maintenant la parole est à Marta de Cidrac. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme vous le savez, cela a été rappelé dans dans les propos qui qui ont déjà qui se sont déjà exprimés la préservation environnementale du milieu marin et de sa biodiversité figurent parmi les enjeux de notre stratégie maritime, sans oublier bien sûr son importance géopolitique, géopolitique, économique, scientifique ou énergétiques détentrice du 2ème domaine maritime mondial, la France possède de nombreux atouts pour bâtir sa stratégie maritime qui passe également par une prise en compte accrue de nos spécificités ultramarines toutefois leur statut de Rup donc régions ultrapériphériques marquant l'appartenance à l'Union européenne et source d'un certain nombre de contraintes liées à Linselles à l'insularité à l'éloignement de l'Hexagone, je pense notamment aux traitements à l'exportation des déchets dans leur zone de proximité géographique rendu impossible en raison d'une législation européenne qui a du sang sur le continent européen mais interroges pour nos outre-mer or derrière ce sujet se cachent de sérieuses menaces pour l'envie, le rendement et la biodiversité et les milieux naturels, souvent uniques au monde, chacun sait à quel point les écosystèmes insulaires sont fragiles et l'histoire est là pour nous le rappeler, Monsieur le Ministre, ces problématiques sont connus et il y a urgence d'agir, et je crois que cela est partagé par beaucoup d'entre nous alors au-delà du déploiement d'une économie circulaire adapté à nos outre-mer quel dialogue allez vous engagez au niveau européen pour que nos spécificités ultramarines soit entendu à l'échelle européenne, je vous remercie. Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice, heureux de voir les Yvelines s'intéresser à l'Outre-mer, mais ça ne m'étonne pas de vous, si tout le monde faisait autant ça on progresserait c'est un vrai sujet, la gestion des déchets outre-mer, j'étais à Mayotte, il y a quelques mois et et on envoie des déchets en métropole, on est dans un système un peu ahurissant le problème des déchets outre-mer est le même que celui sur de nombreuses décharges implantées sur l'ensemble du littoral français futile ultramarins ou pas, en tout cas la hausse du niveau de la mer et l'érosion des traits de côtes croissent le risque que ces déchets se retrouve en mer, ce n'est pas acceptable. Lors du l'Océan Summit à Brest, le président de la République s'est engagé à traiter sous disant les décharges abandonnées sur les littoraux avec un 1er financement de 30 millions sur les 55 décharge prioritaires identifiés 14 sont outre-mer, c'était celle-là, donc il me revient de m'occuper, on a travaillé commencer pour celle de Lens charpentière Martinique mais le sujet n'est pas tout à fait là. Le sujet c'est d'abord européen, vous l'avez dit, c'est l'énorme, je suis en train de travailler à tenter, je vais à Bruxelles le 16 et le 17 novembre un certain nombre d'entre vous le savent, à faire application de l'article 349 du traité européen pour avoir un espèce de ratissage des normes qui ne conviennent pas, j'ai demandé à mes services de faire une liste d'une vingtaine de normes et puis je vais aller les les discuter à Bruxelles, on en reparlera lorsque vous m'interrogerez sur la pêche, donc, 1er sujet : c'est effectivement des dents 2ème sujet c'est d'être favorable au CSR partout, partout, il nous faut travailler sur les CSR, on a commencé en Guadeloupe, je ne sais pas où ça en est exactement, on y a travaillé à la Réunion, il y a des problèmes financiers, je crois, partout le CSR est une bonne est une bonne mesure, ça nous permettra de de travailler en plus sur une économie d'énergie, tout à fait intéressant après je crois aussi que, au-delà des mots, Tous les ultramarins me semble favorable à travailler sur le réemploi des objets oui c'est l'économie circulaire je compte travailler chaque fois que je vais me déplacer dorénavant à essayer de faire émerger de faire émerger une problématique d'économie circulaire et d'emplois. Je sais qu'un rapport, tu as délégation sénatoriale aux outre-mer est en cours, conduit par votre collègue Viviane Malet, il a d'importantes marges de progrès comme d'habitude. On écoutera bien on écoutera mais je voilà deux 3 axes, normes européennes CSR plus travail au cas par cas, sur un certain nombre de décharges. Madame de Cidrac 27 un de secondes à votre disposition. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ces éléments et je compte sur vous pour que vous soyez un interlocuteur exigeant auprès des instances européennes, je vous remercie. La parole est à notre collègue Joël Guerriau. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, la stratégie maritime national de répondre à une double contrainte : assurer notre souveraineté et protéger notre Patrimoine, la France doit être en mesure de contrôler ces espaces marins, il constitue un important facteur de développement, il est facile d'oublier que notre territoire s'étend à l'Atlantique nord, aux Caraïbes, à l'océan Indien à l'océan Pacifique, ou encore aux Terres australes la quasi-totalité de la zone économique exclusive, vous l'avez rappelé se situe autour de nos territoires ultramarins ces espaces Ford sont d'ores et déjà l'objet d'une compétition entre les États, particulièrement dans la région indopacifique, les contentieux territoriaux et maritimes se multiplient à mesure que le centre de gravité du monde si des places dans ces eaux et partout où se trouvent ses intérêts, la France doit maintenir une présence et des capacités crédibles des espaces maritimes sont immenses, il semble bien illusoire de penser que la France peut-elle seule développer des capacités militaires est similaire à celle de la Chine ou des États-Unis, notre pays a des moyens bien plus limités, une voix, cependant nous est ouverte, celle de la coopération avec les puissances qui partagent nos intérêts récemment enjoint à la France et Singapour ont conclu un accord militaire de soutien logistique par ses et coopération, nos 2 pays bénéficient mutuellement de leur complémentarité, la France est le seul pays de l'Union européenne et disposer de territoire en a beau dos pacifique, mais toute l'Europe, il y a des intérêts, avons-nous, Monsieur le Ministre, de nouveaux partenariats européens et internationaux envisageables pour renforcer notre stratégie maritime et de mieux protéger nos ressources en outre-mer, des quelques quelques fois de bruit comme quoi notre nouvelle porte-avions ne se ferait pas, j'espère que vous allez nous aussi nous rassurer sur ce sujet, merci. La défense de la souveraineté maritime et de la souveraineté tout court de nos outre-mer plusieurs d'entre eux, vouloir rappeler le rapport le rappelle, j'ai dit moi-même en introduction est une priorité pour ce faire, est ce que nous sommes capables d'y arriver tout seul, pour partie, c'est sûr, pour partie, c'est sûr, et le ministre des armées, qui connaît bien l'outre-mer dans la stratégie militaire pour les prochaines années, loi d'orientation de programmation militaire développe des moyens pour aller outre-mer, la question qui se pose, il doit prochainement rencontrer le ministre et le chef d'état major des armées, c'est celle de l'équilibrage entre une présence terrestre et une présence la présence terrestre est indispensable en Guyane indispensable sur les îlots du canal de Mozambique ailleurs elle accompagne ailleurs, on a le RSMA qu'il faut développer, mais on ne fera pas présence massive des militaires. Le terre des des fantassins en Guadeloupe, peut-être moins préférable et peut-être moins utile que la présence maritime. Oui, le porte-avions, j'en discuté l'autre jour avec le ministre et ex-ministre des Outre-Mer, actuel ministre des armées se fera et il se fera d'ailleurs en coopération en coopération comme les avions, hein, avec un certain nombre de pays européens, tout seul, on peut le faire à plusieurs, c'est mieux sur la coopération. Je veux dire que je me rendrai à Bruxelles le 16 et le 17. Novembre prochain pour parler de l'article 349 que j'évoquais pour parler dépêche où j'aurai l'occasion de me fâcher devant vous contre la Commission européenne, mais aussi pour parler RUP et défense globale du système, notamment. Sur la biodiversité, j'ai reçu il y a peu, Madame, l'ambassadeur ambassadrice de d'Australie, à Paris, nous avons évoqué ce sujet, elle est tout à fait en phase sur l'idée qu'il faut coopérer sur l'ensemble de ces sujets, je note d'ailleurs que, elle vient d'ouvrir un consulat général à Nouméa avec un Colonna, nous travaillons à l'ouverture de consulat général le plus possible dans les outre-français pour précisément avec des pays amis, renforcer l'idée de cette défense collective de la richesse mondiale et donc européenne et donc française que représentent les outre-mer. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur Guerriau 12 12 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, merci pour votre réponse, évidemment je tiens beaucoup à la notion de partenariat, mais aussi à ce que notre porte-avions puisse continuer à porter haut les couleurs de la France et je voudrais vraiment être rassurés sur ce sujet-là. La parole est maintenant à Joël Labbé. les outre-mer, vous l'avez dit, représentent 80 % de la de la biodiversité française et accueille 86 13 % de nos aires marines protégées, ces zones sont riche d'une biodiversité exceptionnelle, vous l'avez dit, les récifs coralliens les mangroves, dont la valeur est inestimable, mais contrairement aux recommandations de l'UICN la plupart de nos aires marines n'interdisent pas la pêche industrielle, pas même le chalutage de grands fonds véritable menace pour la biodiversité pour le climat il n'y a que dans les aires marines strictement que ces pratiques sont interdites, la France accuse un retard important sur le déploiement de ces zones lors du One Planet Summit, le gouvernement s'est donné comme objectif de protection forte de 10 pour 100 du territoire national en 2030, pendant que la protection forte des zones maritimes s'élève aujourd'hui à 39 % au Royaume-Uni et 24 % aux États-Unis, de plus, comme l'a rappelé le rapport de la délégation pour être effective, ces aires protégées doivent bénéficier de véritables moyens à ce jour, les moyens de la marine nationale ou de l'OFEV dans les outre-mer sont vraiment insuffisant par exemple pour le parc naturel marin de Martinique ou celui de Mayotte ou encore celui des îles Glorieuses, on compte seulement un agent pour 2000 kilomètres sur le ministre, alors que dans quelques semaines, débutera à Montréal la COP 15 de la convention sur la biodiversité marine de la diversité biologique, pardon, quels moyens le gouvernement compte mettre en oeuvre pour, en lien avec les collectivités, protéger la biodiversité ultramarine en rendant effective l'objectif de 10 % minimum de protection stricte de nos eaux. C'est une question qu'on n'avait pas passé donc je vais essayer de d'y répondre quand même sur l'objectif, il y a pas de souci, après vous avez les moyens à mettre en oeuvre, je rappelle que le rapport entre le territoire français et le territoire de sa zone économique est quand même extraordinaire dans le monde, hein, donc on a un problème de coopération, on le disait tout à l'heure, donc il faut y aller. Aire protégée. plus d'interdiction, c'est un objectif que je partage, la question est bien celle des moyens, ces moyens, je l'ai rappelé tout à l'heure, il se développe, on n'arrivera pas, les armées ont obtenu 3 milliards de plus cette année sur la loi de programmation militaire c'est considérable. on arrivera pas à faire 10 fois plus mais le principe de l'interdiction totale. Et à réfléchir, il vaut mieux. une exploitation raisonnée, par exemple, c'est le problème de la légitime dans les taf hein est-ce que on contrôle la pêche à la légitime la réponse, c'est que l'interdiction chaque fois en termes binaires ne me paraît pas souhaitable qu'il faut coopérer, qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables et qu'il faut savoir que ces objectifs atteindront sur la durée et que la et la réponse est dans la coopération, la France n'arrivera pas toute seule, fait le rapport entre les Terres émergées et les océans en zone économique exclusive, fixons-nous des objectifs, je répète la cas particulier, vous avez cité, le canal de Mozambique : attention, c'est un des endroits où la souveraineté terrestre c'est le seul endroit où la souveraineté reste contestée puisque nous allons signer je pense à la fin novembre, désaccord avec la les Pays-Bas sur un bout de frontière contestée à Saint-Martin. Merci, monsieur le Ministre. Notre ami l'abbé avait pris tout son temps et donc maintenant la parole est à Dominique Théophile. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous avons l'honneur aujourd'hui de mettre en lumière l'excellent rapport de nos collègues finira Petrus et Folio, sur la place des autres maires dans la stratégie maritime national permettez-moi ici de les saluer tous la qualité du travail fourni au-delà des recommandations formulées est partagée par notre groupe, le rapport met en avant la place prépondérante de la pêche traditionnelle ou artisanale en outre-mer, a fortiori en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, malheureusement, ce secteur est confronté à de nombreuses difficultés, d'une part, il doit faire face au vieillissement de la profession avec l'exemple de la Guadeloupe, où 65 % des actifs dans le secteur de la pêche sont âgés de plus de 50 ans ensuite la dégradation des conditions de travail conduit à une importante perte d'attractivité qui amplifiée par des faibles rémunérations alors de l'ordre de 500 à 600 euros. Enfin, le vieillissement de la flotte de pêche complète le panorama des difficultés auxquelles font face nos pêcheurs sur ce dernier point le soutien public à l'augmentation des capacités des moyens de pêche est en principe contraire au droit de l'Union européenne, néanmoins, le président, Emmanuel Macron, aux côtés de Jean-Claude Juncker, ancien président de la Commission européenne, s'était engagé à autoriser le financement du renouvellement des flottes de pêche dans les rues, dans le cadre de la conférence des présidents de rue pour se souvient en 2017 à Cayenne. Monsieur le Ministre, vous avez rencontré au mois de septembre, le commissaire européen de l'environnement aux océans et à la pêche afin de l'alerter sur l'urgence du renouvellement de la flotte de pêche des RUP sur l'impérieuse nécessité d'aider nos pêcheurs aussi Monsieur le Ministre, oui, oui, et vous nous faire un état des lieux de l'avancement des négociations sur le renouvellement de la flotte très attendues par la filière.

La proportion de poissons importés par rapport à la proportion de poissons pêchés autour de nous, on est sur un schéma un peu bizarre, je prends 30 secondes si le président le permet et trente secondes de plus pour Mayotte vu autre collègue oui il est là de Mayotte, on en est au point, avec les réglementations qui s'additionnent, je veux dire que suis pêcheur en pirogue utilise des engins de plage, ce qui est interdit, qu'ils aillent pêcher là où ils ont l'habitude de pêcher ça doit changer, j'ai donné instruction assez clair aux affaires maritimes en me disant que j'étais extrêmement fâché qu'il fallait que ça cesse et monsieur le préfet, ce qu'elle a dit que ça se serait très rapidement, mais sur le le sujet de la pêche et du rôle renouvellement de la flotte, je rappelle que grâce à l'action, vous l'avez dit, monsieur le président de la République, on a obtenu, on a obtenu, ça a été confirmée, sous présidence française, le fait que, on a le droit à des aides pour certaines parties de la flotte dans chaque grande tout ça a été fait et c'est légal au titre européen, mais derrière, certain nombre de fonctionnaires de la Commission et la et le commissaire européen qui est letton, on dit il faut d'abord faire un inventaire précis, ça va durer 5 ans, si on veut le faire aux normes européennes, cet inventaire va durer 5 ans, ça va nous coûter un peu d'argent, mais on va le faire avec l'Ifremer, hein, qu'il faut qu'ils s'investissent alors qu'est-ce qu'on fait en attendant j'ai effectivement rencontré le commissaire letton à la pêche. J'ai dit que je préférais les pêcheurs au poisson. Ah, il faut arrêter de considérer que les pêcheurs ultramarins. Sont juste là pour nuire. Au système l'écologie maritime, parce que pendant ce temps là, vous le savez bien, au large de la Guyane, au large de Mayotte au large de la Réunion, il y a des pêcheurs hauturiers, hein, de différents pays qui sont là, au large de la Guyane aussi qui sont là et qui ratisse tranquillement. Nous sommes donc convenus et la lettre est à la signature, parce qu'on l'envoie de le secrétaire d'État à la mer, monsieur Mervil de lui écrire et nous en étions convenus à Bruxelles. notre demande, c'est une demande précise, territoire par territoire, type de pêche, partie de pêche bateau par bateau, type de bateau par type de bateau, de manière à ce que on ait cette autorisation, j'allais dire en dérogation, hein, dans son esprit, moi je trouve que c'est réaliste en dérogation aux règles européennes qui veulent nous imposer par derrière la lettre partira je pense demain, ça a été un peu compliqué de définir, bateau par bateau, un type de pêche, partie de pêche été partie du territoire. Les services m'ont dit de l'adoucir mon Style dans la lettre que j'ai envoyée au commissaire européen, ce qui m'a pris une petite semaine de plus, mais on va le faire à partir de là, j'attends, il m'a promis que lettre serait examinée examiné par le conseil scientifique de la Commission européenne en la matière, en matière de la pêche au mois de novembre, non j'ai dit OK, j'attends au mois de novembre, ensuite j'ai trouvé une collectivité, je vous dirai pas laquelle. Qui a dit moi je fais quand même l'aide en accord avec moi et puis après on ira faire juger ça au tribunal hein, à la Cour de justice européenne, je trouve ça insupportable, je le dis, il faudra aller en Cour de justice européenne pour ça, il faut qu'il y ait une collectivité qui se mettent sur les fonds européens à soutenir la construction de bateaux, c'est ça dont il s'agit, il y a pas de bateau, il y a pas de pêcheurs et puis on verra ce que décidera donc j'ai plutôt confiance. On sait bien. La discussion a été franche comme on peut dire, avec le commissaire européen. Je saisirai tous les parlementaires européens de cette lettre et les parlementaires ultramarins pour que ils appuient partout cette demande qui me semble fondée, face à ce qui est une vraie injustice puisque, au large de Mayotte, vous allez bateaux espagnols qui ratisse tranquillement les bateaux mauricien qui ratisse et nous, on ne peut pas construire des bateaux, voilà ma réponse, elle est assez ferme, je m'en excuse. Monsieur le ministre, votre juste indignation vous a conduit à consommer une part de, de, supplémentaire que vous devrez essayer de rattraper de manière que ça reste équitable avec les parlementaires, la parole est maintenant Madame Gisèle Jourda. Merci beaucoup monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la délégation, mes chers collègues, quelle place réelle voulons-nous donner à nos outre-mer, face aux enjeux géopolitiques d'aujourd'hui grâce à nos forces de souveraineté outre-mer présente sur les quatre océan, la France et dans le club très restreint des États disposant d'une préside sans ce militaire globale, elle y figurent même à la 3ème place ces forces Rimpi ce 5 fonction stratégique protection du territoire national, prévention des conflits connaissance et anticipation, intervention, dissuasion quand vous en disant ce ne sont pas des fonctions accessoires pourtant les forces outre-mer sont placés en bas de la liste des priorités des armées avec une fatigue criante des équipements et des effectifs en précarisation presque continue depuis la fin de la guerre froide dans un environnement opérationnel contraint par de nombreux défis se profile un risque important de rupture capacitaire qui pourrait entraîner l'État à ne plus pouvoir remplir de façon opérationnelle, l'ensemble de ses missions et fonctions stratégiques, le rapport de mes éminents collègues propose un conséquence de faire des outre-mer, la priorité de l'actualisation de la loi de programmation militaire, ma question est donc la suivante : pour vous, nous compter sur vous Monsieur le Ministre, pour faire avancer cet aspect des choses est-il prévu prochainement et rapidement d'actualiser de rééquilibrer nos capacités militaires outre-mer afin de retrouver ce socle de capacité indispensable mais également pour moderniser, adapter nos forces à la géopolitique géopolitique du XXIe siècles et faire de nos outre-mer de véritables points d'appui, c'est indispensable. Pouvez-vous compter sur moi, la réponse est oui, je me bats au sein du gouvernement pour développer tout ça, je rencontre mon prédécesseur, c'est le Cornu pour que la présence Outre-mer soit renforcée et donc j'ai confiance, qu'on va y arriver, la situation n'est pas aussi dégradé, me semble-t-il, que vous le dites, ça c'est pour la marine militaire, vous avez évoqué les ports de pêche, je pense qu'il y a une question qui va m'arriver sur les ports de pêche, donc je répondrai sur les ports de pêche, sinon le président va me

je l'ai dit monsieur le Cornu hé bien en phase avec cet axe de travail : le président de la République, c'est son thème l'indo-Pacifique, je rappelle que la défense de l'Indopacifique chez aussi des territoires qui fonctionne bien bien et territoires où il y a de l'eau des territoires où il y a des ports, des territoires où il y a de l'agriculture, c'est le même message : la défense de l'outre-mer, il y a une défense militaire mais elle passe aussi par le bien-être des populations. Merci, monsieur le Ministre et le mois suivant le rapport qui faut notre débat d'aujourd'hui étaient publiés, consacré à la place des outre-mer dans cette souveraineté maritime ce ce rapport particulièrement riche évoque les différents enjeux, notamment, sécuritaires, économiques, énergétiques, environnementales et climatiques nous considérons effectivement que le combat pour la préservation des hausses des océans est important mais quelle souveraineté maritime peut avoir un sens si nous n'apportons pas un regard particulier à ces territoires ce qui saute aux yeux à la lecture de ce rapport, c'est l'absence de référence à ceux qui sont en première ligne, notamment la population et leurs élus, comment donner toute la place aux outre-mer sans répondre à leurs besoins, si nous voulons valoriser la présence de la France, il est nécessaire d'agir vite de donner des moyens humains capacitaires et de rassembler l'ensemble des acteurs pour une réelle réflexion stratégique, il est important de répondre avec les élus, au manque de moyens pour surveiller ses territoires comme par exemple en leur octroyant du matériel amphibie essentiels en cas de catastrophe naturelle de combler le manque de frégates de surveillance ou d'accélérer l'adaptation aux nouvelles technologies comme l'utilisation de drônes marins, monsieur le ministre, je vous écouté, néanmoins je m'interroge, je vous interroge sur ces points, comment mettre en oeuvre une nouvelle politique de la mer et agir en faveur d'une meilleure protection et gouvernance des océans sans ouvrir son élaboration aux populations et sans renforcer les partenariats régionaux, la question de l'ingénierie est abordée dans le rapport, ne pensez-vous pas que la mise en place d'un organe commun dédié à cette expertise serait utile, d'autant plus que la Cour des comptes nous pousse à développer les capacités propres d'expertise des collectivités d'outre- mer, que comptez-vous mettre en place pour y remédier, l'abstention a été très forte lors des élections présidentielles et législatives, ce n'est pas un bon signe, la mer n'est pas un nouvel eldorado, comme l'indique le rapport, ces références aux enquêtes prédatrice prédatrice doit être abandonnée au profit d'une conception rassembleuse respectueuse des hommes et des éléments, c'est l'essence de de mon propos est de mes questions merci Monsieur Migaud. première éléments de réponse à la suite du 7 septembre d'appel de Fort-de-France, les stratégies pour la création de valeur dans les outre-mer se construiront avec les élus, les LED sont en train de partir 2ème lettre pour montrer comment on va le faire et c'est bien dans cette différenciation responsabilisation des collectivités outre-mer que se trouve une part de la réponse, une part de réponse puisque bien évidemment la mère fait partie des objectifs et donc des stratégies Première éléments de réponse. 2ème, élément de réponse est une étude prospective sur l'économie bleue dans les Drom, comme on dit maintenant est désormais finaliser cette étude, les orientations seront partagés avec tous les territoires, en vue d'alimenter ces ces ces discussions, je voudrais vous rappeler que dans la stratégie nationale mer et littoral telle qu'elle vient de de paraître, c'est bien là déborde du ministère de l'Outre-mer, je le dis volontiers, je n'étais pas là aurait été inscrit le tourisme côtier avec une vision ultramarines spécifique koweïtien, ce qui le rôle des canaux et des mangroves, notamment pour le climat, la défense du climat côté inscrite le sujet de l'aquaculture donc sur votre réponse de participation, je dis, hein, on va diffuser l'étude prospective sur l'économie bleue et ça sera un des éléments de discussion dans les suites du 7 septembre et de l'appel de Fort de France 2 je veux le dire honnêtement, je suis pas très sûr qu'il faille associer toute la population à la présence d'un porte-avions de corvette ou de frégates dans les océans, par contre, par contre, les associés via responsabilisation différenciation ce qu'on est en train de démarrer, ça me semble une évidence si la stratégie bleu fait partie de la stratégie globale là-dessus vous pouvez compter sur moi. Merci monsieur le ministre, alors Madame Dindar dans c'était le tour de parole, a dû s'absenter, et elle a souhaité que ce soit monsieur Philippe Folliot, qui pose sa question et la parole. monsieur le monsieur le président, effectivement, notre collègue vous voulez vous interroger Monsieur le Ministre, sur un certain nombre de points et d'éléments et notamment sur une question qui est une crèche, une question essentielle qui est celle de l'ouverture des Outre- mer par rapport à leur environnement régional

les collectivités territoriales ultramarines dans le cadre de ces échanges régionaux dans le cadre de ces différentes instances, c'est un élément qui est un élément particulièrement important et parce que, somme toute, je crois qu'il y a un de vos prédécesseurs, monsieur le Ministre, qui a marqué l'histoire de la République, c'est Michel Rocard qui dans ses fonctions de ministre du Plan, à l'époque avait choisi de faire sortir les outre-mer de la notion d'exclusive avec la métropole et l'Hexagone et donc dans ce cadre, pouvez-vous nous rassurer sur l'implication donc et et le l'ouverture aux collectivités territoriales pour ses conférences régionales. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, et la France hexagonale et les territoires ultramarins, il n'y a pas de capacité à vivre éternellement comme ça les territoires ultramarins doivent vivre dans leur environnement, alors il y a des cas différents sur les pacifiques dans le Pacifique là. là. Denis et la Polynésie ont déjà capacité de nouer des accords notamment à chercher des accords de libre-échange, ce que je cherche, c'est à voir, dans le cadre des RUP, c'est d'une discussion qu'on doit avoir et sur lesquels les présidents de collectivités territoriales, avec lequel je suis en relation, le ministre de l'Intérieur et Madame la première ministre sont éminemment d'accord, il nous faut ouvrir. Les territoires nos îles. Alors en rendement régionale, y compris par des accords d'État à État y compris par un regard sur les échanges commerciaux qu'est-ce que ça peut changer, d'avoir un accord pour la France d'avoir un accord commercial de libre- échange avec Angela, par exemple, simplement c'est on est au milieu de l'environnement et il y a pas de solution des territoires ultramarins, s'ils ne sont pas dans leur environnement et tous les élus que je vois sont d'accord avec cela, c'est une discussion que j'ai avec Madame Colonna c'est une discussion que j'aurai, je crois que le rendez vous d'ailleurs pour demain 7 heures avec le ministre du commerce extérieur, hein, comment progresse sur ce sujet-là. J'ajoute : j'ai rencontré la CE PME au niveau national ce matin le président cela, ça se joue, pas simplement entre les élus des territoires et l'État, ça se joue, pour autant que les chefs d'entreprise, hein s'y mettent et s'ils mettent plein pot. C'était le sujet de la discussion, ils m'ont dit : vous venez à des problèmes de normes dire il faut importer et etc et donc je ramène à l'article 349 sur lequel on on travaille, c'est bien un sujet global, création de valeur insertion dans l'environnement.

D'élus, mais certains l'ont vu de la lettre de feuille de route que ma tracé, monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour être sûr que cette stratégie, on la partage bien tous les deux et qu'elle soit validée par Madame la première ministre, c'est le cas, c'est écrit, donc je vous adresserai cette feuille de route qui reprend à peu près ce que vous avez dit monsieur le député Folliot. Il est devenu sénateur. Vous avez 30 secondes chers collègues. Oui, monsieur le Ministre, et effectivement c'est un enjeu qui est un enjeu important, parce que les choses bougent dans l'environnement, quand on regarde le la question de et et l'environnement du sud de l'océan Indien, nous avons l'île Maurice, qui est un à un rapprochement avec l'Inde, la Chine, qui a des visées et qui interviennent sur les Seychelles et sur la Tanzanie nous avons Madagascar qui qui flirte avec la Russie et que donc dans ce cadre-là, il est important que nous puissions acté, dire le fait que les collectivités puissent être associés, par rapport à ces enjeux géostratégiques, mais aussi sur d'autres éléments, comment peut-on être crédible si nous n'avons pas une vision globale, je prends un exemple par rapport aux Comores, nous avons une aide aux de développement au niveau des Comores mais l'immigration amnistie n'est un enjeu essentiel pour les comment comme ça l'est aussi par rapport au Suriname et à d'autres pays vis-à-vis de la. d'autres aurait fait pareil que vous, mais là ça fait quand même 34 secondes je je. Je je termine pour dire simplement que si ce sont des enjeux qui sont des enjeux essentiels, merci de votre attention. La parole est à monsieur Chevreau. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nos outre-mer permet à la France de disposer d'une véritable richesse en matière de biodiversité marine comprise, elle représente ainsi 80 % de la biodiversité et englobe des enjeux particuliers comme la protection des coraux et des mangroves cette biodiversité pourtant plus que jamais menacé par le dérèglement climatique, ces dernières années, l'acidification des océans lié au réchauffement climatique, a engendré des épisodes de plus en plus importants et récurrents de blanchiment des coraux

ces écosystèmes joue un rôle essentiel de nurserie pour les poissons et leurs pertes provoque d'ores et déjà un véritable effondrement de la chaîne alimentaire qui se répercute sur l'accès à la nourriture ainsi que sur les activités économiques comme la pêche et le tourisme selon le GIEC, si le réchauffement climatique atteint plus 1 virgule 5 degrés 70 à 90 % des récifs coraliens pourraient disparaître et avec un plus de degrés ce risque monte à 99 notre pays dispose de la deuxième zone économique exclusive au monde, qui représente 8 % des mers du globe, à ce titre, il est de notre responsabilité d'agir en faveur de la protection de la biodiversité, de ces zones depuis 2010, la France a renforcé la création d'aires marines protégées qui ne représentaient que 0,8 % de la zone économique exclusive, en 2009 contre 24 %, 10 ans plus tard, néanmoins, le rapport de la mission d'information sénatoriale met en exergue le manque de moyens humains et matériels pour protéger de manière effective ces zones je souhaiterais donc connaître les actions menées par le gouvernement pour protéger cette biodiversité menacée quelles sont concrètement les moyens mis à disposition des aires marines protégées, en fait, il s'agit de garantir notre souveraineté sur nos espaces maritimes et sans donner les moyens, notamment avec les forces armées et aussi tous ceux qui agissent pour la préservation de la biodiversité, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, permettez-moi de vous saluer et je vais récupérer sur le temps qu'a dépassé le sénateur folie. La question que vous avez soulevées, a été, est au coeur de vos débats, hein, on a déjà essayé de réponse j'ai essayé d'amener quelques éléments voir quelques arguments supplémentaires oui exemplarité des Outre-mer en matière de protection de la biodiversité, je rappelle que l'objectif de classer 30 % des espaces terrestres et maritimes sous juridiction française en aires protégées et dépassé et déjà dépassé, alors après, il s'agit de savoir comment les surveille, mais il est dépassé, avec l'extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises qui devient la 2ème plus grande aire marine protégée au monde avec 1,5 millions de kilomètres carrés, un autre dossier est en cours pour la avec la protection des îles éparses, le parc naturel marin de Mayotte et le plus grand de France. La France entend poursuivre ses efforts en la matière, dans la perspective de la prochaine conférence des Nations-Unies sur les océans qu'organisera en France, en liaison avec le Costa-Rica, pays exemplaire en matière de, de, d'écologie et défense de l'environnement dans la dynamique du One Océan Summit organisé à Brest cette année je m'attacherai à ce que les outre-mer ils prennent toute leur place, Je voudrais citer deux 3 informations hein première, c'est que je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Françoise Gaill et avec Olivier Poivre d'Arvor pour essayer de travailler à la perspective d'une espèce de GIEC des océans, c'est très compliqué, ça fait 2 ans que j'ça mais je pense qu'on va progresser sur ce type de sujet, la 2ème, c'est que j'ai rencontré Monsieur Bougrain-Dubourg pour LPO protection des oiseaux, je l'ai dit, donnez-moi 10 actions exemplaires 10 actions exemplaires.

La parole est à madame Jasmin. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je remercie la délégation et particulièrement son président Stéphane Artano pour ce débat, monsieur le Ministre, à la suite du passage de la violente tempête Fiona en Guadeloupe les 23 et 24 septembre dernier, je souhaite vous interroger au sujet de la politique littéral littoral menée par votre gouvernement pour prendre en compte les effets du réchauffement climatique en outre-mer, en effet, le réchauffement climatique constitue un des défis fondamentaux de la stratégie maritime nationale et son impact sur l'habitat, le littoral est très important en outre-mer où les rives sont de plus en plus les les outre-mer sur les territoires, pour la plupart insulaire en proie à de violents risques naturels et particulièrement maritime désormais rendus plus fréquents et dévastateur, nous l'avons vu récemment avec le bouleversement climatique, c'est le cas de la tempête et avec cela ils s'ajoutent également les algues l'échouage des algues Sargasses face à cet enjeu climatique, il convient de revoir les orientations des documents stratégiques du bassin maritime pour y inclure une fiche sur l'habitat littoral cette bande littorale, héritage du passé colonial évidemment de la France fait encore partie du domaine maritime de l'État et bénéficie à ce site de garanties spécifiques qui font qu'elles ne peuvent être cédés sans une procédure de déclassement particulière les agences du du cinquante pas géométriques sont donc les acteurs essentiels, comme l'a souligné le rapport de la délégation sénatoriale sur le logement, mais aussi dans ce rapport il est aussi question de l'habitat indigne particulièrement aux Antilles, l'urgence c'est donc de reloger les familles sans droit licite exposées aux risques naturels majeurs prévisible, prévisible, de plus en plus, compte tenu des différents aléas, monsieur le ministre, je souhaite savoir qu'est-ce que vous, vous envisagez de faire pour clarifier et pérennisées à la fois les missions de l'agence de cinquante pas géométriques, mais aussi pour protéger les familles parce qu'il y a également le compte merci général de l'environnement qui demande développement

Madame la sénatrice Jacquemin, vous savez que je connais le sujet le 1er point c'est, je crois que c'est d'accord partie c'est de repousser à 2025, le transfert de la zone des cinquante pas géométriques aux collectivités territoriales, il est prévu, brillante que cette zone soit remise aux collectivités territoriales, on a le sujet à Saint-Martin aussi qui est un sujet très difficile d'ici là, il me semble qu'on a de choses à faire, c'est de finaliser la cartographie des zones ce qui nous permettra : premièrement d'engager le processus de régularisation, là où c'est possible, très clairement, hein, que lorsqu'il y a transfert on sache qui est régularisables au profit des habitants et deuxièmement d'engager les démarches de relogement pour les personnes situées en zone dangereuse, c'est ça les 2 perspectives : je m'en suis entretenu avec le président Mussington avec madame la sénatrice de de Saint-Martin Martin aussi, c'est ça que nous allons faire, je me rendrai à Martin pour commencer dès la semaine prochaine, d'ailleurs, sans passer par la Guadeloupe, je m'en excuse, mais je pense que c'est un respect pour les 100 Martinois et c'est ça qu'on veut faire et j'irai en Guadeloupe, je crois que c'est au mois de novembre avec le même message on délimite et après on transfert et on le fait d'accord partie et on délimite pour régulariser ou reloger. Madame Lana Téphany, vous avez la parole. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la délégation manteau jeté un salué les travaux de nos 3 collègues portant sur le sujet, constatant notamment la peine de la nation française à valoriser cet immense potentiel situé à 97 % dans ses outre-mer et je souscris pleinement aux recommandations de ce rapport pour faire face aux défis qui nous attendent demain. Mon maritime Mon maritime dans notre zone mon interrogation porte plus particulièrement sur la zone indopacifique au vu de l'actualité sur cette partie de la planète devenue le centre de gravité, stratégique, économique et financier, on ne peut que rappeler que la France détient un statut majeur de cet espace maritime grâce à ces territoires ultramarins et sa Z, aujourd'hui, les Américains se mobilisent fortement un nouveau dans la zone face à l'expansionnisme de la Chine ainsi la semaine dernière la Polynésie française, représentée par son président Édouard Fritch a été invité et a participé, en sa qualité de membre à part entière du Forum des îles du Pacifique audace au rassemblement organisé à Washington de tous les États insulaires de la zone, à l'invitation du président Biden en effet les États-Unis confirment leur appui et le soutien financier aux États insulaires pour faire face à l'heure de la vulnérabilité liée au réchauffement de la planète et pour une meilleure et plus grande coopération à leur développement durable vu l'Océanie convoité, vu l'accélération des enjeux actuels géostratégique est-il envisagé renforcement de nos bases militaires dans nos collectivités d'Outre-Mer, et plus particulièrement en Polynésie française où, depuis l'arrêt des essais nucléaires, les moyens maritimes de l'armée aurait été fortement redéployés hors de notre territoire. Merci, monsieur le Ministre. Un mot d'abord sur cette réunion à Washington, j'ai vu le président Fritsch pendant qu'il était à Washington, notre ambassadeur Philippe Étienne a travaillé, finalement, il est arrivé à un accord sur la participation de tout le monde, c'était la nécessité de la présence de la France, via ces territoires, être là en faisant attention quand même à ne pas ce que nos territoires ultramarins prenne parti sur le Detroit de Taïwan par exemple, même si la Chine est effectivement active voir fait d'un peu de d'activisme mais depuis le Brexit la France est la seule nation de l'Union européenne présente présente dans la région, on revient à cette coopération européenne. Je peux pas me prononcer à la place du ministre des armées, mais je rappelle qu'il y un renouvellement très conséquent des moyens, la marine nationale entre dix-sept et vingt-six, pas moins de 13 navires neufs auront été mis en service dans les territoires ultramarins dont 9 dans la zone indopacifique trois La Réunion, 3 en Polynésie 3 en Nouvelle-Calédonie, à ce jour, aujourd'hui pas moins de 4 frégates patrouille dans la zone et je ne compte pas l'émission effectuées dans les zones exclusives ultramarine par les bâtiments de la marine basée dans l'Hexagone, là c'était les bâtiments qui sont basés là-bas, au-delà de la question des moyens. Effectivement, je l'ai dit et je le redis, notre grand enjeu et de renforcer les coopérations avec avec nos partenaires, avec nos partenaires amicaux. Il faut multiplier les exercices militaires conjoints, lutter contre la pêche illégale, renforcer les moyens de réponse aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Stimuler la diplomatie économique essayer d'impliquer l'Europe, plus encore, et dans notre stratégie, l'Europe dans la région, chez le sujet UE péter OM le 22 novembre à Nouméa, si nous arrivons à faire en sorte que la commission accepte de le financer, ils ne reprennent pas les crédits qu'elle avait donné à l'association qui s'occupe de cela, on est en phase, c'est du temps, c'est de la coopération et c'est des moyens qui sont là, vous pouvez le constater au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure des bâtiments qui navigue dans la zone. Merci, la parole est maintenant madame Annick Petrus pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le secteur de la pêche ne constitue pas encore une véritable filière agricole à ce jour à Saint-Martin à la fin 2021 21 pêcheurs professionnels seulement exercent sur l'île, la pêche constitue une activité non régulière, dont une part significative est informel, environ un tiers Hélène Da leur traditionnelles et artisanales essentiellement lié aux loisirs ou à la subsistance l'possède le marché aux poissons qui fournit les restaurateurs et les habitants en produits locaux, une part importante de la consommation pour vient également d'Angela, il va voisine, l'absence d'équipements en procédant à la transformation du poisson ne permet malheureusement pas de répondre à une demande locale en croissance dans le cadre de l'économie bleue, la structuration du secteur de la pêche et de ses acteurs, le décret 2016, 781 du 10 juin 2016 offre un cadre réglementaire à la création de comité territorial des pêches à Saint-Martin en donnant notamment à la chambre consulaire interprofessionnel de Saint-Martin, la possibilité d'installer, d'animer et d'organiser cette structure si le comité n'existe pas, à ce jour, un processus de conventionnement est en cours et sa mise en oeuvre est attendue par les professionnels du secteur, notamment les syndicats de marins pêcheurs et les aquaculture de Lille, dans dans le but de développer le secteur du nautisme à Saint-Martin et toutes les activités qui sont liées, la collectivité termine au programme de formation liée à Homs liées aux métiers de la mer afin de sensibiliser, former nos jeunes Saint Martinois si les fonds européen pour les Affaires maritimes et la pêche, couvrant la période 2021 2027 pour permettent de dégager une enveloppe de 3 8 millions alloués au secteur, l'État pourrait-il nous accompagner financièrement, notamment pour l'aménagement de 2 points de débarquement de la mise en place d'une zone technique de pêche nous aider à l'installation de jeunes pêcheurs à Martin et en fait nous accompagner sur le renouvellement et la modernisation de la flotte, je vois merci. Oui, merci de l'avoir souligné. ça s'appelle le fonds européen pour les Affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, qui prend la suite du du pour l'ensemble de vos collègues pour la période 2021 2027 ce fonds passe de 700000 euros à 3 8 millions d'euros uniquement pour ça, Martin, il nous faut le mettre en oeuvre le mettre en oeuvre rapidement là-dessus, j'ai confiance, on va y arriver, après il y a un 2ème, sujet qui n'est pas fait et je vais le faire je pense avant la fin du mois. C'est lait de renouvellement de la flotte, on a parlé des problèmes qui étaient là, mais le régime d'aide concernant Saint-Martin n'avait pas été notifiée à Bruxelles n'avait pas été notifiée à Bruxelles et donc ça marche pas, donc on va le faire, je pense d'ici la fin du mois. Se posera le même problème de l'effectivité ah mais là, on sera dans la, dans le sujet global que je négocie avec Bruxelles donc hein oui ce fonds de 3 millions il faut s'y mettre, précisément avec le comité que vous avez évoqué de il faut que ça Martin rentre les le système d'aide au renouvellement de la pêche pour ça, la première étape c'est de notifier le régime d'aide pour qu'il s'applique à Saint-Martin et la 3ème étape, ça sera que ce système fonctionne mais ça, ça a été mon intervention de tout à l'heure. Merci, la parole est maintenant Madame Viviane Artigalas pour le groupe socialiste, écologiste et républicain, merci madame la présidente, monsieur le Ministre, les îles Eparses située dans le canal du Mozambique et dépendant de l'administration des Terres australes et antarctiques françaises représentent seulement 43 mètres carrés de surface terrestre cumulés, mais l'ensemble de leurs eaux sous juridiction rue juridictions françaises totalisent plus de 640000 kilomètres carrés, soit environ 6 % du territoire maritime français de par leur isolement, elles n'ont jamais été perturbées par l'activité humaine et sont de ce fait des sanctuaires pour une exceptionnelle biodiversité marine et l'étude d'écosystèmes encore fonctionnel les deux arrêter de 1975 et de 1994 les classes en réserve naturelle, il y a, interdisent toute pêche, cette zone est l'une des régions d'air primaire constituant l'avenir du Patrimoine mondial, marin, elle doit donc être protégé et préservé, ce que la France s'attache à faire grâce au déploiement d'une présence militaire permanente, or depuis 50 ans, les îles éparses font l'objet d'une double contestation territoriale de la part de Madagascar et de l'île Maurice, leurs ressources halieutiques énergétiques et minières que la France s'est attaché à ne pas exploiter suscite convoitises et dans revendications les îles éparses sont donc devenus pour la France, un enjeu de souveraineté, entendez-vous, Monsieur le Ministre, poursuivre les efforts initiés par le président François Hollande et son homologue malgache pour négocier une substitution équilibré répondant aux enjeux de sécurité de défense de la biodiversité et de lutte contre la pêche illicite dans cette zone. Monsieur le Ministre. Effectivement, l'ensemble des villes du canal de Mozambique sur l'objet d'abord sont une richesse extraordinaire et sont donc l'objet de contestations territoriales à l'encontre de la possession française. Je veux dire que j'ai cité le président François Hollande le président Macron est sur la même ligne, la défense clairement sur la même ligne, la défense de la souveraineté française sur ce

on va faire la guerre toute de suite, mais se réunira très prochainement pour ce sujet et parler ce différend territorial parallèlement une feuille de route sur la recherche avec l'ensemble des organismes de recherche sur la les îles Eparses sera signé très bientôt, vous l'avez souligné. L'armée française y est présente avec l'armée de terre, hein, et ils se relaient sur le sujet, donc il est pas du tout dans l'intention du président de la République de baisser la garde, bien au contraire, simplement, négociant avec Madagascar c'est l'objet de la commission mixte qui va se réunir et rendons utile saisi l'en matière de recherche cette là aussi la feuille de route qui sera signé.

vraiment les appétits des puissances étrangères touche directement la place stratégique de la de la France, donc je suis d'accord avec vous Monsieur le Ministre, nous devons vraiment être vigilant et poursuivre avec détermination cette gestion et réaffirmer la souveraineté de la France sur Cécile je vous remercie. La parole est maintenant Monsieur Dominique de Lège pour le groupe Les Républicains. La France est présente avec ses forces de souveraineté sur l'ensemble des océans et à cet instant, je tiens à rendre hommage aux 8500 personnels militaires qui assurent ces missions sur l'ensemble de des océans et au-delà à tous les personnels civils qui contribuent les zones de responsabilité permanente dont nous avons la charge concerne une quarantaine de pays avec lesquels nous entretenons des partenariats et coopération, ils sont souvent en voie de développement, ma question est la suivante : en quoi et comment l'AFD vient en soutien et coopère avec nos forces de souveraineté au profit des pays avec lesquels elles sont en relation et, ce faisant, facilite l'exercice de leur mission, par une meilleure acceptation et compréhension de leur président, je vous remercie. Monsieur le Ministre. Hein, je peux vous dire que je suis en relation fréquente avec l'AFD et son président, avec une priorité que je lui donne à son action dans les territoires ultramarins notamment des territoires dans le Pacifique, on a vraiment besoin de l'AFD de nous sommes convenus avec le président Rio. Et Madame la Ministre, Colonna, hein, de travailler, précisément sur ces coopérations sur comment on fait pour aider ces pays à peine, c'est un des sujets, c'est-à-dire de présence de la France, mais c'est un des sujets, immigration. Le SMIC à Madagascar, d'après mes informations, doit être à peu près à quarante euros chargé je sais même pas s'il existe, à à dans les îles des Comores. Le salaire chargé d'un travailleur du tourisme c'est 400 euros. En Guadeloupe, Monsieur monsieur le Sénateur Lionel, on en est un peu au-delà, heureusement, et donc nous avons tout intérêt, c'est l'intérêt de la France, de travailler avec ces pays pour qu'il se développe, que le salaire augmente, hein, que le salaire augmente, dès qu'on arrive.

Objectif de développement, c'est là l'accord que j'ai avec le président au. 2 perfectionner d'améliorer son action sur un certain nombre de sujets, j'ai un certain nombre de sujets. Dans les territoires eux-même, à ce propos là je vous donner une information, je suis en train d'essayer de travailler avec lui ce qu'il me reste qu'un second sur un système d'affacturage public qui permettrait aux petites entreprises de bénéficier de l'apport de trésorerie dans l'attente du paiement par les collectivités locales qui mettent sous un peu de temps, a payé en général elle paye simplement vous avez un gap de trésorerie qui est considérable et avec l'AFD, on essaye de travailler sur cette affacturage, il serait un bol d'air considérable aux économies ultramarines. Monsieur de Delage, il vous reste une minute 04. Merci madame la présidente, pour les zéro quatre, monsieur le Ministre, je me réjouis que vous soyez en relation avec l'AFD, pour autant, excusez moi, ça ne suffit pas, je me suis rendu il y a pas très longtemps à la Réunion, j'ai remis ce matin un rapport à la commission des finances sur l'engagement de nos forces de souveraineté, ce qui m'a été dit très clairement, c'est que les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos relations avec les pays voisins pourraient être largement atténué si s'de souveraineté et d'une façon plus générale, la présence française avait une meilleure coordination avec l'AFD et les moyens que nous mettons. En terme de coopération ces pays, alors je n'en dis pas plus j'entends votre engagement, mais je me permets de vous dire que, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et qu'il y a beaucoup de progrès à faire, je compte sur vous. aujourd'hui la mer ses richesses et les perspectives qui sont liés mérite de s'inscrire, profondément dans notre pays et la stratégie maritime 2023 2029 doit s'y employer, à cet égard je voudrais plus particulièrement m'attacher à la préconisation numéro 7 du rapport de la délégation outre-mer qui vise à développer les classes à enjeux maritimes dans les établissements scolaires par des partenariats avec les grandes fondations et des personnalités engagées dans le monde maritime, il serait judicieux en effet de pousser notre jeunesse vers le large à l'incitant par le biais de projet scolaire à s'inscrire dans des démarches de sensibilisation aux enjeux maritimes, ce sont souvent dans les jeunes vocations que les projets décisifs trouve naissance qui étaient très à la science à l'industrie, à l'aménagement du territoire ou encore à la Défense, je tiens d'ailleurs à saluer le commandant et son équipe page du Marion-Dufresne Dufresnes qui, en collaboration avec l'Ifremer on a âpres mener une centaine de jeunes de Mayotte et de la Réunion à bord pour mieux leur faire connaître la mer, les océans et les métiers qui s'y rattachent, et cela c'est a duré pendant un mois les classes à enjeux maritimes sont nés au lycée français de Barcelone de la rencontre de 2 femmes issues du monde de l'enseignement et de l'industrie navale, elles ont pour vocation de faire prendre conscience à des élèves de 4ème de 3ème et de seconde, qui sont les citoyens d'une grande puissance maritime, il s'agit également de leur donner les clés de lecture pour comprendre que les mers et les océans sont le théâtre de tous les défis de demain qui sont écologiques, économiques et géopolitiques, la mise en place de ces classes est très récente mais déjà 27 projets sont lancés à l'échelle nationale, à l'échelle de mon département, 3 écoles se sont engager mais je constate avec regret qu'une seule classe, ça peut être répertoriés

Anne Lopez le Vidourle est devenue un enjeu ultramarins c'est bien et et je m'en suis trouve satisfait juste les outre-mer montre la voie et c'est bien normal ce développement des classes enjeux maritimes dans les établissements scolaires, vous avez cité, vous y étiez, je vous en remercie l'initiative École bleu Outre-Mer permettez-moi de mettre une partie des remerciements sur le ministère de l'Outre-mer, puisque c'est lui qui l'a organisé de A à Z, bien sûr, avec tous les participants, nous allons essayer de recommencer parce que c'était vraiment bien et en plus, ça a été suivie d'une réunion des chefs de service. Divers et variés pour les sensibiliser aux affaires de l'outre-mer et en plus, c'était dans le canal de Mozambique qui des soucis pour beaucoup de gens ici, je voudrais vous signaler le projet de construction d'un lycée de la mer, à la Réunion, rentrer de à la rentrée 2027 projets, la construction d'un lycée professionnel maritime également en cours à Mayotte, prévue en 2028 ensuite, sur l'ensemble des associations, je veux vous dire que, on essaye de réformer notre système de subventions aux associations diverses, c'est ouvert, soit par un c'est ouvert ça mon cabinet, il suffit de téléphoner, vous demandez la directrice adjointe de cabinet qui a en charge tout ce sujet-là, éducatif et je peux vous dire qu'il y aura vraiment un bon accueil vraiment un bon accueil, moi je suis prêt à dans le Gard qui, vous le savez, une partie de mon coeur, hein, pour aller expliquer cela aux écoles. madame la présidente, monsieur ministre, mes chers collègues, en tant que dernier intervenant je vais faire le lien avec le projet de loi énergies renouvelables qui nous arrive dans quelques jours, ici au Sénat, dont je suis le rapporteur et et donc de face, je souhaite aborder la place des énergies marines renouvelables dans les territoires ultramarins manque de gisement foncier faible interconnexion au réseau électrique continentaux dépendance au jeu des énergies fossiles importés et une vulnérabilité face au changement climatique, tous ces facteurs rendent l'accélération de la transition énergétique plus urgente encore en outre-mer que dans l'Hexagone, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 inscrit un objectif d'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer, d'ici à 2030, j'ai une croissance rapide des énergies renouvelables, force est de constater que cet objectif ne sera pas atteint les énergies renouvelables représentent toujours moins de 30 pour 100 de mix électrique en moyenne dans ces territoires avec de fortes variations qui peuvent s'expliquer évidemment en Guyane, le mix électrique est composé à plus de 50 % d'énergies renouvelables, tandis qu'à Mayotte et à la Martinique, ce taux demeure inférieur à 10 selon une étude de l'Ademe de 2020, l'autonomie énergétique pourrait être atteignable dans nos outre-mer d'ici à 2035, à condition d'accompagner dans la durée le développement des énergies renouvelables, non seulement terrestres et maritimes, en particulier l'éolien Offshore énergie thermique des mers, selon cette étude au maximum de leur potentiel des énergies marines renouvelables pourraient représenter jusqu'à 30 % du mix électrique à Mayotte et en Guyane et 10 % la Réunion en Guadeloupe et à la Martinique, pour l'heure ces énergies occupe toujours une place très marginale dans nos territoires ultramarins, alors même que la France lors de la richesse de son domaine maritime, il existe pourtant un vaste potentiel qu'il s'agisse de l'Offshore posé comme je l'ai évoqué ou d'énergie plus émergentes comme l'éolien flottant l'énergie houlomotrice et hydroliennes ou l'énergie thermique des mers, des expériences novatrices existent mais elles sont rares et soeur ta difficultés techniques et financières, tandis que la la nécessité d'adapter les technologies ses spécificités de chaque territoire ralentit le développement de filières industrielles pérennes sur le ministre, alors où nous outre-mer peuvent oeuvre à la révision de leur programmation pluriannuelle de l'énergie que prévoit le gouvernement pour accentuer le développement des énergies marines renouvelables au-delà du texte qui s'avance dans l'ensemble de ces territoires, merci monsieur le Ministre.

une fois, c'est là une fois si, si, une fois c'est lui, c'est le 1er sujet : le 2ème sujet c'est que je veux dire ici, c'est dans les énergies renouvelables, auquel je suis extrêmement favorable, elles seront prises en compte dès lors qu'il y aura la PPE elle point être prise en compte de gré à gré ou sur des appels d'offres pour l'instant, les appels d'offres et je me suis fâché avec le ministère de la transition écologique et énergétique n'étaient pas lancé, donc on va lancer des appels d'offres sur les énergies renouvelables de mais ces appels d'offres ne doivent pas cacher l'absolue nécessité et l'absolue nécessité, quel que soit le développement des énergies renouvelables des énergies une énergie bio liquide Plensa bio liquide avec une grosse usine de manière à stabiliser à sécuriser, c'est tout le problème de la rivaux en Guyane, c'est le même problème en Corse dans les et Denis, il faut au delà des énergies renouvelables, accepter de payer et la creux le fait et le gouvernement le fait à travers la CSPE accepter de payer une usine qui fonctionne le minimum qui fonctionne au minimum, on fait une usine non pas pour qu'elle fonctionne, mais pour assurer la sécurité sur les énergies outre-mer Marine outre-mer hein, à ma demande lorsque j'étais président de l'des décisions ont été prises en comité interministériel de la mer pour que, dès lors qu'il y a une PPE toutes les études soit financé par la CSPE pour ses implantations d'éoliennes en mer, encore faut-il je le redis que le PPE soit votée par ailleurs les les régions ultramarines doivent être fiers de l'innovation en matière d'énergie, c'est le sujet des soit qu'à la Réunion, c'est le sujet de l'usine hydrogène à Saint-Laurent du Maroni et de tas d'autres sujets on ne mais il faut voilà à un moment donné, je sais pas l'état à un moment donné il y a des opérateurs, il faut que les PPE soit votée, sinon les opérateurs n'y vont pas donc petite. Expression d'humeur sur le fait qu'elle soit pas votre diminution depuis Gênes. Merci monsieur le ministre, et vous avez pu me faire partager au Sénat votre compétence dans les 2 minutes. Monsieur le président de la délégation. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous venons d'avoir un échange très riche, et je remercie chaleureusement le ministre chargé des Outre-Mer Jean-François Carenco mes collègues d'avoir aborder des problématiques qui ne concerne pas seulement l'outre-mer, mais là, en réalité, la place de la France dans le monde, je salue l'engagement remarquable de nos 3 rapporteur Annick Petrus Philippe Folliot et Marie-Laure Phinéra Horth qui ont fait à la fois un travail d'évaluation, mais également un travail de proposition à travers les 40 recommandations, l'ambition de la délégation que je leur présider et de replacer l'outre-mer au coeur de la stratégie maritime national ce qui me semble-t-il, a fait défaut en 2017 Monsieur le Ministre, nous appelions de nos voeux le débat que nous venons d'avoir enfin de donner un élan commun et coordonnée à la légitime ambition maritime de notre pays, nous espérons que vous ne vous arrêterez pas là et que le Parlement sera à l'avenir pleinement associés à l'élaboration de la prochaine stratégie maritime et que nos territoires ultramarins pourront y apporter leur contribution, indispensable, nous avons entendu hier lors du débat sur les fonds marins, le secrétaire d'État à la mer, évoqué le Conseil national de la mer et des littoraux comme un parlement de la mer, cette instance ne peut se substituer, comme l'a rappelé Annick Petrus ça la légitimité des assemblées parlementaires, le Sénat, l'Assemblée nationale pour se prononcer sur les orientations d'une politique déterminante pour notre avenir, notre conviction est aussi qu'il faut sans tarder, engager une évolution culturelle autour de l'océan, l'espace maritime ultramarins est en effet au confluent de tous les grands enjeux actuels les enjeux géopolitiques sécuritaire et diplomatique, on l'a dit, la France est en effet bordée de 23000 kilomètres de frontières maritimes avec près de 30 États une situation unique au monde, faut-il le rappeler, c'est aussi le seul pays présents sur les quatre océan Atlantique avec la Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'océan Indien avec la Réunion Mayotte l'océan Austral avec les Terres australes et antarctiques l'océan Pacifique, avec de la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et sans oublier de la passion qui partons cher à notre collègue Philippe Folliot, il faut aussi prendre en compte bien évidemment les enjeux de communication 90 % du commerce mondial est assurée par les voies maritimes les câbles numérique, câble sous-marin, en l'occurrence sur 95 % du trafic mondial des données, ce qui est phénoménal, les 11 énergétique avec l'objectif de développement des énergies marines renouvelables vous l'avez indiqué monsieur le Ministre, les enjeux scientifiques et de recherches avec notamment l'exploration des grands fonds encore largement méconnu, je vous renvoie à cet égard un autre débat d'hier sur les abysses et à l'excédent rapport de nos collègues Michel Canuet et Téva Rohfritsch enfin les enjeux climatiques et environnementaux bien évidemment qui ne sont pas les moins des Outre-Mer représentent, faut-il le rappeler 80 % de la biodiversité française, il est plus que jamais nécessaire d'encourager massivement l'acculturation fait maritime dans notre pays dans l'Hexagone comme dans nos outre-mer, c'est important de le souligner, pour y parvenir, 2 leviers sont indispensables : l'éducation et la formation, lesquels ont été insuffisamment mobilisés jusqu'à présent, notre collègue vive être Lopez que je salue, a insisté, à juste titre sur les classes à enjeux maritime mais notre rapport avance toute une série de propositions de bon sens sur ce sujet, comme par exemple le promouvoir le brevet d'initiation à la mer dans tous les collèges et lycées, en particulier dans les régions maritimes j'ai pas eu de gestion pour l'emploi et des compétences par territoire pour mieux orienter les jeunes vers les métiers de la mer enfin généralisé les plateformes des métiers avait du maritime dans les territoires ultramarins à cet égard l'année 2022 frais, a priori, un contexte exceptionnellement favorable pour promouvoir une ambition maritime plus conforme aux réalités géopolitiques géographique de notre pays, la conjonction inédite de la double présidence du Conseil de l'Union européenne et de la conférence des RUP par la Martinique devait permettre de mettre en avant les atouts que représente nos territoires pour l'Europe et défendre désorientation, tenant compte de leurs besoins et de la réalité, la présidence des RUP étant assurée jusqu'en novembre 2022 un bilan est prématurée, mais nous ne manquons pas de le dresser d'ici la fin de l'année on attendons et comme vous le savez les collectivités ultramarines souhaite notamment être mieux associés aux visites et réunions de haut niveau, organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères lorsqu'elles connaissent donc ça concerne ce serait déjà un grand pas pour l'efficacité de notre diplomatie si nous parvenions à cette approche coordonnée, je voudrais insister également sur l'opportunité de faire des outre-mer un levier pour la stratégie indo-Pacifique ça a déjà été dit ce soir, dont on a beaucoup parlé au cours du dernier quinquennat mais qui ne doit pas, selon nous, se limiter à une dimension militaire, je note le secrétaire d'État à la mer hier à utiliser le terme d'un d'Océanie, ce qui traduit peut-être une approche plus française des réalités géostratégiques dans cette région du monde, dont on peut se féliciter de cette région est présenté comme le le nouveau centre de gravité du monde et beaucoup d'indicateurs vont effectivement dans ce sens, elle concerne 60 % de la population mondiale, un tiers du commerce international et contribuera d'ici 2030 pour 60 % du PIB mondial, nous l'avons indiqué des responsables territoriaux lors de nos auditions pour la stratégie nationale reste aujourd'hui malheureusement 13 États tôt centré sont réel associations des collectivités ultramarines, ça a été demandée par plusieurs collègues, qu'elles soient, ce qui est vrai pour l'indo-Pacifique est également vrai pour la stratégie maritime dans son ensemble, monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre message est clair : il faut changer d'optique l'Outre-mers les outre-mer sont la clé de la réussite de la stratégie maritime française, je vous remercie. séance quelques instants pour effectuer des rotations nécessaires pour le poursuivre l'ordre du jour.

La séance est reprise à l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à actualiser le régime de réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, présenté par Madame Nathalie Goulet la procédure accélérée a été engagée sur ce texte dans l'addition générale, la parole est à monsieur Thani Mohamed Soihili, rapporteur de la commission des lois.

Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous examinons en urgence la proposition de loi déposée par notre collègue Nathalie Goulet que je tiens à remercier pour sa vigilance, il s'agit de régler diverses questions liées à l'éligibilité des juges consulaires des tribunaux de commerce avant les élections annuelles qui ont été décalés à dessein par le gouvernement à la fin du mois de novembre, c'est la 2ème fois et j'espère la dernière que notre collègue à à prendre une initiative en matière d'élection des juges consulaires des tribunaux de commerce, à l'Automne dernier, nous avions déjà adopté un texte pour régler les malfaçons hérité de la loi pacte la loi du 11 octobre 2021 voté conforme en première lecture dans les 2 chambres, a ainsi permis de réintégrer les membres un exercice et ancien membre des tribunaux de commerce dans le vivier des candidats aux élections des juges consulaires. Il s'agirait aujourd'hui de renouveler l'exercice car la conférence générale des juges consulaires de France et le ministère de la justice ont de nouveau relevé des difficultés relatives au régime de l'élection des juges consulaires, je tiens à vous rassurer tout de suite les travaux que j'ai menées n'ont pas mis en lumière de risque d'invalidation des mandats des juges consulaires ou de disparition des tribunaux de commerce, comme certains l'évoquent, il n'y a eu semble-t-il aucun contentieux, remettant en cause les élections organisées depuis 2019, l'enjeu est certes de corriger certaines erreurs de plumes, mais surtout d'élargir le vivier des candidats en permettant aux cadres dirigeants de se présenter aux futures élections avant l'adoption, à 2019 de la l'heure de la loi pacte les cadres dirigeants salariés faisaient partie du corps électoral des délégués consulaires, et à ce titre, étaient éligibles aux fonctions de juge consulaire la suppression et le remplacement des délégués consulaires par les membres élus des Chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat ont mis indirectement un terme à leur éligibilité or leurs compétences, spécialisé en droit bancaire ou Cambiaire par exemple, et leur disponibilité sont précieuses pour la résolution des litiges soumis aux juridictions commerciales à titre d'exemple, la conférence générale des juges consulaires de France estime que les cadres dirigeants salariés représentent actuellement plus de 40 pour 100 des juges consulaires, un exercice dans les tribunaux de commerce, de grande taille. La commission a trouvé opportun de rétablir l'éligibilité des cadres dirigeants salariés étant rappelé qu'ils seraient soumis aux mêmes règles déontologiques et disciplinaires, que l'ensemble des juges qui composent les tribunaux de commerce, elle a toutefois estimé que l'Arctique le 1er apporte une modification qui dépasse cet objectif puisqu'il vise à modifier le corps électoral des chambres de commerce et d'industrie, en permettant aux cadres dirigeants salariés de l'intégrer, c'est la raison pour laquelle elle a supprimé l'article 1er et modifier l'article 3 qui porte sur l'éligibilité des juges consulaires pour y intégrer les cadres dirigeants. L'article 2 de la proposition de loi à bord d'un tout autre sujet, il vise à créer une 5ème cause de cessation des fonctions des juges consulaires en cas de refus de siéger sans motif légitime, la commission a estimé que ce sujet n'était pas frappée du sceau de l'urgence par ailleurs dans un précédent rapport dont nous étions rapporteur François Bonhomme et moi-même l'année dernière nous avions relevé qu'une réponse disciplinaires pouvait être apportées à la situation du refus de siéger et avions recommandé que les chefs de cour se saisissent de leur pouvoir disciplinaire dans ces conditions, la commission a préféré limiter les débats à la problématique qui font d'urgence de la proposition de loi, à savoir le vivier des candidats aux élections des juges des tribunaux de commerce, l'article 2 a ainsi été supprimée dans le texte issu de ces travaux ce sujet mériterait plutôt d'être intégrés dans le projet de loi sur la justice du quotidien qui est envisagé en réponse au rapport du comité des états généraux de la justice. L'article 3 qui traite de conditions d'éligibilité aux fonctions de juge consulaire est vraiment le coeur de la proposition de loi, il vise à rectifier certaines malfaçons issu de la loi pacte, il s'agirait, en particulier de clarifier la question de l'inscription sur les listes électorales des Chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, le législateur de 2019 n'a pas souhaité qu'il s'agisse d'une obligation de double inscription, la commission a donc approuvé la modification de rédaction. L'article 3 vise également à permettre aux juges un exercice et aux anciens juges et en 6 ans d'ancienneté d'être réélu dans leur tribunal ou un tribunal limitrophes, sans condition de résidence, tout en prévoyant un régime dérogatoire spécial fixées par décret en Conseil d'État pour les tribunaux non limitrophes. Hein, l'état de la législation, les juges, un exercice et les anciens juges doivent justifier d'une domiciliation ou d'une résidence dans le ressort du tribunal où il candidate ou d'un tribunal limitrophes dans tous les cas sur cette dernière question, j'ai eu une hésitation, car les conditions actuelles résulte de la loi du 11 octobre 2021 et il pouvait paraître injustifiée de les retoucher aussi rapidement sans élément nouveau toutefois le ministère de la justice et la conférence générale des juges consulaires de France on fait voilà, on fait valoir que 307 juges consulaires pourrait ne plus se représenter aux élections si la règle était maintenu, il s'agit de personnes qui étaient domiciliés dans le ressort du tribunal dans lequel elles étaient élus en raison de leur activité professionnelle et qui, à la retraite ne dispose plus de 7 domiciliation, il leur serait donc désormais difficile de se porter candidat, sauf à se faire domicilier chez un tiers, compte tenu de cette information, la commission a choisi une solution d'équilibre la levée la condition de résidence lorsque le juge v se veut se représenter dans son tribunal d'origine ou un tribunal limitrophes, cependant, elle a maintenu cette condition pour les candidatures d'un des tribunaux non limitrophes il lui apparaît en effet nécessaire que le candidat conserve un lien géographique minimale avec le tissu économique local du tribunal dans lequel il souhaite exercer et mes chers collègues, le texte modifié que la commission vous invite à adopter, il permettra, je l'espère, aux juridictions commerciales de bénéficier d'un vivier élargi de candidats aux fonctions de juge consulaire. Merci, monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice Nathalie Goulet. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons ce soir afin de débattre ensemble la proposition de loi de votre excellente collègue de l'Orne Nathalie Goulet, qui porte sur un sujet important pour notre économie, dans le contexte que nous connaissons, je veux bien sûr parler de la justice commerciale. Les siècles d'existence de la justice commerciale sont une preuve irréfutable de son efficacité, mais aussi de son adaptabilité, ceux de justice a su se renouveler maintes et maintes fois pour relever sans cesse de nouveaux défis, jusqu'à aujourd'hui, et je vous en effet un rôle essentiel souligné avec insistance par le rapport du comité des états généraux de la justice auquel votre président de commission François-Noël Buffet a d'ailleurs grandement participé et je veux ici chaleureusement l'en remercier. Très concrètement, la présente proposition de loi vient donc tout d'abord élargir le vivier des candidatures des juges des tribunaux de commerce. Vous l'aurez compris le gouvernement, il y est très favorable, suivant la même logique d'élargissement du vivier des candidats juges consulaires la présente proposition de loi vise à supprimer la condition de résidence à l'égard des juges consulaires et des anciens juges présentant à leur propre réélection et s'il est indispensable que lors de la première élection les juges consulaires et leur entreprise au sein du ressort du tribunal de commerce,

En cours de mandat et ne possède plus d'entreprise ni de résidence dans le ressort duquel ils ont été élus, cette situation très fréquente dans les grandes régions par exemple en Île-de-France en Provence Alpes Côte d'Azur ou dans les Hauts de France. Ainsi, le D en l'état du droit actuel. Et son application aurait pour effet d'empêcher la réélection des juges les plus expérimentées sur un ressort dont ils connaissent pourtant toutes les spécificités ils ont exercé leur activité professionnelle depuis de nombreuses années et on connaissent parfaitement le tissu économique, or c'est précisément de ces juges dont nous avons grandement besoin ceux qui ont une expérience juridictionnel confirmé et qui connaissent charnellement, oserais-je dire leur ressort, ils y occupent fréquemment les postes stratégiques de présidents de tribunaux de commerce ou de président de chambre l'adoption de la proposition de loi, enrichi par les travaux de la commission des lois du Sénat dont je veux ici saluer le rapporteur Thani Mohamed Soihili et son excellent travail permettra de lever cet obstacle, permettez-moi d'insister, et je termine sur l'importance d'une adoption rapide de cette proposition de loi afin qu'elle s'applique aux prochaines élections prévues le 21 novembre et le 4 décembre 2022 acteurs de terrains indispensable. Les juges consulaires accompagne et soutiennent nos entreprises dans les périodes difficiles, c'est la raison pour laquelle au-delà de tout clivage partisan le gouvernement apporte son soutien plein et entier à la présente proposition de loi et permettez-moi, en conclusion de saluer également le travail de coconstruction réalisé avec le Conseil national des tribunaux de commerce, la conférence générale des juges consulaires de France, soit ils ont tous ici remercier. Merci, monsieur le Ministre, la parole, la discussion générale et maintenant monsieur Guy Bénard Roche pour l'Europe Écologie Solidarité territoire et pour une durée de 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, madame, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je commencerai par saluer le travail de notre collègue Nathalie Goulet qui grâce à son attention particulière à la situation des juges consulaires permet de veiller à la sécurité juridique à la sécurité juridique de leurs conditions d'exercice assis à leur pérennité, alors que l'ensemble de la justice et souffrante, il est heureux que le gouvernement puisse compter sur une telle alliés pour couvrir Sissonnais négligence du moins plusieurs oublie, en fait, oui, nous nous retrouvons ici car le temps presse, avec la tenue prochaine des nouvelles élections consulaires, plus de 130 tribunaux a la responsabilité d'étudier, près de 140000 affaires par an, outre les difficultés communes avec le système judiciaire, problème de moyens financiers recrutements nécessaires, notamment de greffes des tribunaux ont aussi subi des modifications importantes et successifs sous les derniers mandats par exemple au travers de la loi pacte cette loi pacte se voulant simplificatrice à réformer les modalités d'élection des juges consulaires qui seront désormais élus par les membres des de commerce et d'industrie CCI et des chambres de métiers de l'artisanat CMA, en plus des juges et ancien juge du tribunal, elle a donc eu des conséquences importantes sur le corps électoral dans celle d'écarter les cadres dirigeants salariés des entreprises aussi le présent texte sur lequel la commission s'est retrouvée propose de permettent de nouveau à ses cadres d'être et l'acteur Direct de ces formations juridictionnelle cette modification se justifie d'autant plus qu'il a été rappelé que 40 % des juges consulaires en exercice sont des cadres dirigeants salariés à l'heure où la participation citoyenne et démocratique est en grande difficulté dans notre pays, il apparaît plus que raisonnables de permettre une plus grande participation aux institutions de notre quotidien, ou plutôt dans ce cas, de permettre le matière de cette participation active aux tribunaux de commerce dans ce même esprit à la fois de bon sens, mais aussi, disons-le, à peu de bout de rustines face au manque de magistrats, la Commission a accepté de lever les conditions de résidence recours l'Euro relocalisation en cas de retraite aurait assécher le vivier que constitue les juges à la retraite qui peuvent vouloir continuer d'exercer dans juridiction d'origine ou limitrophes. Le choix de valoriser l'expérience des anciens juges ou des juges déjà en exercice reste équilibré mais nous devons néanmoins évité l'écueil d'une trop grande professionnalisation l'équilibre recherché difficile entre Real Application dans la vie locale et besoin de renouvellement, mais il ne doit pas être perdu de plusieurs rapports déjà mis en avant les difficultés de la justice commerciale dont a présenté il y a un an à peine, par notre rapporteur Thani Mohamed soit lit le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise en mai 2021 difficulté confirmée lors des travaux des états généraux de la justice si la confiance dans l'institution judiciaire, Monsieur le Ministre, vous est chère, vous comprendrez bien que cette proposition de loi n'est qu'une petite Pierre à l'édifice de travaux certes colossaux mais nécessaire, nous resterons attentifs à l'équilibre obtenu en commission mais surtout aux suites des efforts qui seront faits pour aller vers une confiance dans la justice et même, comme l'a dit Madame la première ministe vers l'amélioration de la justice du quotidien en attendant ces mesures et paroles et manquements des rédactions précédente et en conservant le vivier d'éligibilité des cadres dirigeants, constituent de premières mesures d'urgence équilibré permet donc au groupe écologiste de voter une telle proposition. Merci, la parole est maintenant à monsieur Gilbert Favreau pour le groupe, les républicains et pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le Ministre, Monsieur le, le rapporteur je crois que notre président de la commission des lois les tribunaux de commerce sont des institutions vénérables puisqu'elles ont été créées par un édit de 1563 du roi Charles IX leur statut d'origine a été souvent modifié au cours des siècles mais la proposition de loi qui nous occupe, vit simplement à actualiser le régime de réélection des juges consulaires, organisé par la loi, pacte du 22 mai 2019 qui avait réformer le système électoral des juges consulaires déjà la loi du 11 octobre 2021 avait apporter certaines corrections au texte de 2019, et celui-ci mérité qu'on lui en apporte encore quelques-unes d'abord en clarifiant les conditions d'éligibilité des juges pour faciliter le renouveau, le renouvellement de ces magistrats consulaires quelques fois en nombre insuffisant, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ensuite en créant une nouvelle cause de cessation des fonctions de ces juges enfin en corrigeant quelques erreurs commises dans les lois précédentes, cela étant précisé la proposition de loi qui nous occupe, a fait l'objet du dépôt de trois amendements, 2 amendements de suppression numéro un et 2, et un amendement, de modification donc 3 articles dans la PPL trois amendements, c'est un texte qui est court, qui est simple le je le précise les les articles de la proposition de loi étaient concernés par ces amendements, la cousine, la commission des lois, les a adopté tous les trois, l'adoption des 2 premiers amendements entraîne certes le rejet des mesures prévues par les articles 1 et 2 de la proposition de loi mais le rejet de l'article 1 est compensée par l'amendement numéro 3 le rejet de l'article de ne présente aucun caractère d'urgence et le problème du refus de siéger pourra être réglé comme il l'est actuellement devant le Conseil, les conseils des prud'hommes par une loi de justice ultérieures, c'est l'article 1442 tiré 12 du code du travail, en ce qui concerne l'amendement numéro 3 qui était un amendement, de modification, il vise utilement à permettre d'abord dire des juges ayant déjà exercé pendant au moins 6 ans et qui sont domiciliés dans le ressort du tribunal concerné ou dans le ressort des tribunaux limitrophes, mais également des cadres exerçant des fonctions de direction dans les entreprises situées dans le ressort du tribunal concerné ou des tribunaux limitrophes c'est c'est nouveau et ça mérite d'être souligné, en résumé, l'adoption de des 3 amendements déposés permet de façon pragmatique d'atteindre les objectifs visés par la proposition de loi d'abord avec les deux premiers amendements de suppression, le 1er qui supprime certes, l'article 1 de la proposition de loi mais avec une reprise du contenu de l'article supprimer dans l'amendement numéro 3, le deuxième, qui prévoit de régler ultérieurement le problème du refus de siéger comme il est actuellement devant les juridictions prud'homales enfin avec le 3ème, amendement qui, au-delà de quelques corrections de pure forme permet d'accueillir dans les tribunaux d'anciens membres du de tribunaux de commerce et des cadres d'entreprise, mais surtout, c'était l'objectif 1er de la proposition de loi. poules modifications intervenues permettront à la fois de conforter les tribunaux de commerce qui viendrait à manquer de juges et de tenir dans les délais, ça a été dit également tout à l'heure par monsieur le Ministre, les élections qui auront lieu le mois de au mois de décembre prochain, c'était le but de la proposition de quoi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a un an, nous avions approuvé un texte encadrant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce, il s'agissait de palier à certaines imperfections de la loi, pacte qui avait été adoptée de façon hâtive la proposition que nous examinons aujourd'hui vise à compléter la loi du 11 octobre 2021 on apportant de nouvelles modifications rectificative, c'est donc la deuxième fois que notre coeur leg Nathalie Goulet prend une initiative sur la question du renouvellement des juges consulaires des tribunaux de commerce et nous saluons son engagement, il s'agit d'un sujet capital dans notre économie, la justice commerciale où la justice consulaire est une institution dans notre système judiciaire vieille de 5 siècles en effet les juridictions consulaires ont été créés par un édit de 1563 du roi Charles IX pris à l'initiative de notre de chancelier Michel de l'hôpital, dont la statue domine cette tribune et et nos débats cette longévité des démontre toute l'importance de cette justice le texte qui nous est soumis en entend donc remédier aux insuffisances de la retouche législative que nous avions à l'année dernière, car les difficultés relatives au régime de de l'élection des juges consulaires ont été une nouvelle fois relevé l'article 1er clarifie ainsi certaines conditions de l'éligibilité des juges consulaires, l'article de entend régler la question du refus de siéger, on a six ans, en s'inspirant, donc d'une disposition déjà en vigueur devant les le conseil de prud'hommes et enfin l'article 3 qui traite de l'éligibilité des juges consulaires et apporte plusieurs corrections à la loi pacte et notamment la suppression de la condition de la double affiliation chambre au CCI et chambres de métiers pour être candidat pour une un 1er mandat de juge au tribunal de commerce, la commission a donc apporté plusieurs modifications et nous partageons donc sa position qui a consisté à se concentrer sur la problématique de l'éligibilité, l'urgence c'est et notamment donc dans l'article 3 je me réjouis qu'elle ait trouvé donc opportun de rétablir l'éligibilité des cadres dirigeants, aux fonctions de juge consulaire, élargissant ainsi le corps des candidats. Avant de conclure : je tiens donc à saluer le travail de du rapporteur de notre collègue Thani Mohamed Soly, monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc cette proposition de loi apporte de nouvelles réponses fort utile aux imperfections de la loi pacte donc le groupe, les indépendants votera bien évidemment cette proposition de loi. Le. La parole est maintenant Monsieur Stéphane Artano pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues m'comme l'avait très justement rappelé l'an dernier, notre collègue Maës Carrère lors de l'examen du précédent texte sur l'élection des juges consulaires, ce serait une erreur de considérer les dispositions techniques comme des choses de second nous observons très souvent, elles sont la condition du bon fonctionnement des systèmes entiers en ce qu'elle permette son accomplissement cohérent aussi je veux d'abord souligner le travail et la persévérance de notre collègue Nathalie Goulet qui porte ce sujet de l'élection des juges consulaires et travaillent en perfectionner les mécanismes je veux également saluer bien évidemment les travaux de notre commission des lois et de notre rapporteur Thani Mohamed qui a apporté un nombre important d'ajustement, voici donc la problématique qui peine une peine cela a déjà été dit par une première loi il y a un an, nous avions pu préciser les modalités de réélection de certains juges consulaires préciser également certaines inéligibilité à ses fonctions corriger d'une interprétation du du Conseil d'État, s'agissant du délai de viduité ou encore fixé des précisions quant aux conditions imposées par la loi pour faire partie du collège électoral des juges consulaires dans la continuité, le texte de la commission que nous discutons aujourd'hui vient revoir les conditions d'éligibilité des juges, l'exercice et ancien juge dans le tribunal de commerce d'origine ou un tribunal limitrophes, il n'y a pas lieu de s'opposer et bien évidemment aux dispositions qui vont être débattus, ceci étant entendu mes collègues du groupe RDSE et moi-même regrettons malgré tout cette répétition des textes bien sûr, elle est le symptôme d'un travail législatif, ces dernières années, trop hâtif et trop volumineux au regard du ton que dont nous disposons, inutile de redire tout ce que l'inflation législative a pu avoir nuisibles mais il a souvent été question de rustines durant les travaux préparant cet examen, la loi de l'an dernier d'ailleurs, on était une première, celles-ci sont serait presque une seconde et s'il fallait poursuivre cette métaphore, j'ajouterai que compte l'argent, tu es trop abîmé il faut souvent songer à la changer, alors j'espère évidemment Monsieur le Ministre, mes chers collègues, que nous n'aurons pas revenir une nouvelle fois sur cette problématique de l'élection des juges consulaires, ces observations est en fait le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, la parole est maintenant Monsieur Dominique Théophile pour le groupe RDPI et pour trois minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Nathalie Goulet d'avoir déposé cette proposition de loi, ce texte est évidemment très technique, il n'en revêt pas moins une importance particulière dans la mesure où il vise à faire en sorte que la loi dite l'une des lois majeures du Preez précédent quinquennat soit expurgé de ces dernières malfaçons et appliquées conformément à la volonté du législateur, ce texte se présente aussi le grand Avantage d'élargir le vivier des candidats aux fonctions de juge consulaire via le rétablissement de l'égalité des cadres dirigeants, un des pays ne peut que souscrire à ces objectifs dont la concrétisation est d'autant plus urgente que les prochaines élections consulaires doivent se tenir entre le 21 novembre et le 4 décembre dans quelques semaines, la réforme du collège électoral des juges des tribunaux de commerce, entrera en vigueur, ce dont je me félicite pour la première fois les juges consulaires seront élus par les membres des chambres de commerce et d'industrie et des membres des chambres de métiers de l'artisanat, en plus des juges en exercice et des anciens juges il faut espérer que la suppression du régime électoral à 2 degrés, conduira à une hausse du taux de participation après que la présente proposition de loi où a été définitivement adopté, il conviendra d'engager une réforme en profondeur de la justice commerciale depuis des années 2007 justice du quotidien et de proximité, parfois considéré à tort comme une justice périphérique a connu plusieurs améliorations, je pense notamment à l'extension de la compétence des tribunaux de commerce au litige entre artisans qui a été permise par la loi dite J 21 de 2016, nous devons suivent le mouvement de réforme à cet égard les propositions formulées par le comité des états généraux de la justice constitue une bonne base de travail, tout le monde s'accorde sur l'impérieuse nécessité de rang doit plus lisible l'organisation des juridictions commerciales ainsi je me réjouis que le comité et proposé d'expérimenter le remplacement de tribunaux de commerce par des tribunaux des affaires économiques dans la compétence, la compétence serait élargie aux agriculteurs, aux professions libérales et aux associations, je trouve particulièrement intéressante la proposition du comité consistant à créer un référé, sauvegarde de l'entreprise, sur le modèle du référé liberté des juridictions administratives, les juges consulaires serait ainsi dotée d'un outil leur permettant de répondre à des situations urgentes enfin une solution devra impérativement être proposé aux difficultés des tribunaux de commerce, la justice commerciale souffre d'un manque criant de moyens aussi, il faudra probablement poser la question du maintien de sa gratuité et étudier la possibilité de mettre en place un droit de timbre barémiser qui serait acquitté par la partie qui rentre à peine 10 recevabilité de l'instance toutes les pistes de réflexion qui ont été mises sur la table par le comité des états généraux de la justice sont très innovantes, nous aurons l'occasion d'un débat que l'an prochain dans le cadre d'un projet de loi en attendant ce cadre ce grand débat sur la réforme de la justice commerciale notre groupe votera pour la présente proposition de loi, je vous en remercie. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la justice consulaire n'est pas périphérique, elle ne l'a jamais été les gigas crises récentes, si vous me pardonnez ce néologisme, calquée sur les méga-feux et leurs implications la rendent de plus en plus central dans la vie économique dans la vie tout court, de nombreux de nos concitoyens lors de l'examen de la première proposition de loi vouée à pallier les dysfonctionnements identifiés dans la loi, pacte nous avions tous le Covid et la crise sanitaire en tête. Aujourd'hui, nous avons toujours le Covid beaucoup d'entre nous l'ont même contracté mais nous devons aussi composer avec l'instabilité internationale née de la guerre en Ukraine et la crise climatique et énergétique, les prêts garantis par l'État doivent être remboursés, même si certaines facilités peuvent être offertes dans certains cas, l'inflation est de retour, je n'irai pas plus loin sur les aspects conjoncturels, les laissant à nos collègues des finances et des affaires économiques bien plus disert que moi en la matière mais ce contexte il est présent dans la tête des dirigeants d'entreprise que nous rencontrons partout dans nos territoires, les difficultés sont là et l'intervention de la justice consulaire les accompagne parfois à l'approche des prochaines élections des juges consulaires des tribunaux de commerce, la proposition de loi de notre collègue Goulet rectifier favorablement par le rapporteur, que je veux féliciter pour son travail permettra de rétablir les cadres dirigeants salariés comme faisant partie intégrante du corps électoral des délégués consulaires et donc de les rendre pleinement éligibles aux fonctions de juge consulaire, les questions disciplinaires et des considérations plus générales sur la justice consulaire mérite sans doute d'être examiné dans le cadre du projet de loi faisant suite aux états généraux de la justice et dans un calendrier moins contraints, vous l'aurez compris mes chers collègues, le groupe socialiste, écologiste et républicain apportera son plein soutien à cette proposition de loi pour défendre la pérennité et l'efficacité de la justice consulaire. La parole est maintenant à la présidente Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste et pour trois minutes madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi de Madame Goulet dont nous discutons en cette fin d'après-midi, est une loi, cela a été dit d'actualisation de précision à la marge, elle vise donc à corriger des erreurs introduite par la loi, pacte et elle éclaircit les conditions de l'élection des juges consulaires dans les 3 tribunaux de commerce, cette proposition de loi et ce n'est pas son objectif ne bouleverse aucunement le fonctionnement des tribunaux de commerce, ce qui sur le fond et et d'ailleurs problématique pour nous, nous nous comptons non donc ici, à la forme, or c'est bien sur le fond qu'il serait pertinent d'intervenir car, de fait, c'est le trois confirme la volonté de sanctuariser la juridiction commerciale et ne prend pas en considération les critiques régulièrement émises quant à sa composition, puisque les salariés ne sont pas inclus inclus dans le processus des tribunaux commerciaux, les risques de conflits d'intérêts de mer o demeure aussi prégnant dans un microcosme où tout le monde se connaît et tout le monde fait des affaires, nous sommes ici en autarcie totale, nous continuons à adouber une juridiction non paritaire et je le répète : les salariés en sont écartés et non éclairés est l'idée que nous nous faisons de la justice et du principe même d'impartialité, je ne pense pas, nous en sommes malheureusement bien loin, on précise, mais on n'avance pas être modeste dans l'action, ce n'est pas être à la hauteur de notre mandat, et ce alors que la France est capable de proposer des Tribunaux paritaires efficace efficace et impartiaux tels les tribunaux prud'homaux alors malgré ces critiques, nous pouvons que nous pouvons formuler à l'égard de cette PPL je voudrais saluer le travail de notre collègue Nathalie Goulet et notre groupe votera ce ce ce ce texte en attendant un véritable débat de fond sur la composition des tribunaux de commerce en France une composition qui n'a d'équivalent nulle part en Europe, une composition qui ne saurait nous satisfaire. Merci madame la présidente, dernier orateur inscrit monsieur Philippe Bonnecarrère pour 3 minutes et pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai une appréciation très favorable des tribunaux de commerce de leur sérieux de leur implication de connaissance à la fois théorique et pratique, c'est un bon équilibre et je ne partage pas totalement, du moins en tant qu'ancien praticien les réserves qui viennent d'être formulées par la présidente, si nous avons 3 questions à évoquer la première question est celle de la composition du corps électoral, ceci a été largement évoqué se priver de 40 pour 100 de ce Didier électoral de cadres expérimentés qui sont pertinents dans la connaissance de la vie des entreprises serait regrettable de ne pouvons bien sûr qu'approuver la proposition faite par notre collègue Madame Goulet avec le travail de de perfectionnement assuré par la Commission sur le 2ème sujet : la question de la déchéance, je n'ai pas l'impression que ce sujet soit comme si pratique cela de magistrats qui refuseraient d'exécuter leurs activités il y a, à mon avis, d'autant moins de risques que s'il y avait un problème, il apparaîtrait assez vite, or les magistrats devant le très bien les commerces ont un système de mandat, 2 ans avant de pouvoir avoir un mandat complet, par ailleurs, comme nous avions un petit peu de temps, j'ai regardé rapidement à la bibliothèque, le code de commerce 724 1 et suivants, j'ai quand même été étonnée, chers collègues de l'importance du dispositif de déontologie pratiquée pour les tribunaux de, de, de commerce et au regard des atteintes possibles à la probité, et à mon avis là le Conseil national conférence nationale je me souviens plus que les termes exacts pour la la structure faîtière déontologique a largement les moyens de résoudre ce problème, j'ai même plutôt été impressionnant en sens inverse par l'étendue des obligations, et en particulier par les incompatibilités je vous monsieur le garde des Sceaux, que j'ignorais complètement que le mandat de ma juges consulaires, soit par exemple incompatible avec le mandat de conseiller municipal, ceci pour dire que le niveau d'incompatibilité, oui, oui, oui Monsieur le Conseiller, alors ne parlons pas de conseiller départemental la tout aussi listé dans dans le texte, les obligations déclaration d'intérêts dont ceux-ci, en résumé, pour dire que les obligations pesant sur les juges consulaires sont quand même très important, troisièmement, sur les questions de domiciliation, on comprend bien l'idée, l'idée, vous avez proposé de limiter à Despé limitrophes les chiffre que vous nous avez donné, je me suis rapporteur montre que là aussi, il serait dommage de se priver de magistrats compétents le groupe centriste votera bien sûr le texte proposé, ce qui bien sûr n'était pas en débat puisque celle qui a porté le texte parti en notre groupe, merci à toutes et tous. Merci la discussion générale est maintenant Close, nous allons passer la discussion du texte de la commission l'article et supprimer l'article 2 est supprimé, je vais mettre aux voix l'article 3 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, il y a,-t-il demande d'explications de vote, je n'en vois pas qui est pour, qui est contre qui s'abstient la proposition de loi et donc adopté je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 35 sur les conclusions pour le débat sur les conclusions du rapport 5 ans pour reconstruire la souveraineté économique et la séance est suspendue.